En application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi du 23 juillet 2010. Prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a émis un avis favorable à la nomination de Monsieur Gilles Leblanc, aux fonctions de président de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Lors du jour appelle le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 22 et 23 mars. La parole est de tabac DAB Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'écologie et des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes.

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, c'est un plaisir de vous retrouver ici pour préparer, avec vous, le Conseil européen des 22 3 mars prochain ce rendez-vous important donnera lieu en réalité à plusieurs réunions différentes que j'aborderai successivement le Conseil européen se déroulera jeudi après-midi, il reviendra sur plusieurs sujets assez classiques, qu'il s'agit du semestre européen ou du marché unique, notamment pour fixer l'objectif de faire adopter d'ici la fin de la législature, 2 priorités européennes le paquet numérique sur lesquels les travaux commencent à peine et le projet d'Union de l'énergie qui doit permettre d'atteindre les objectifs de transition énergétique très ambitieux que l'Union se fixer porte 1030, nous y reviendrons si vous le souhaitez, je voudrais surtout relevé que le Conseil européen devrait soutenir notre approche d'une Europe plus protectrice en abordant de façon positive, 3 domaines sensibles, dans lesquelles le point d'équilibre européen évolue progressivement en notre faveur. La mention d'une forte politique industrielle européenne qui est une priorité pour nous. Mais vous le savez, qui ne va jamais de soi au niveau de l'Union européenne sur le commerce, l'appel à ce que les co-législateur trouve un accord pour mieux contrôler les investissements. Un meilleur équilibre dans l'ouverture des marchés publics. Va clairement dans notre sens, nous souhaitons que la discussion permette aussi de parler de la mise en oeuvre des mesures de défense commerciale et rappelle la nécessité que les futurs accords commerciaux prennent pleinement en compte l'accord de Paris je relève que le Conseil européen devrait demander à la Commission de présenter une stratégie de réduction des gaz à effet de serre compatible avec cet accord, enfin 3ème. Sujet : le projet d'autorité européenne du travail proposée par le président Ion coeur vise à aller vers une plus grande convergence sociale par le haut dans l'esprit de la révision de la directive sur le détachement des travailleurs. Au-delà, le Conseil européen, reviendra sur la décision prise par les États-Unis, d'augmenter les droits sur leurs importations d'aluminium et d'acier. Pour des motifs allégués de sécurité nationale, au détriment notamment de l'industrie européenne, la commission travaille avec les États-Unis, avec l'appui des États-membres pour obtenir une exemption pour l'Union. Mais si nécessaire, elle se pressent prépare à prendre des mesures de sauvegarde de nos intérêts industriels et de rééquilibrage de nos échanges dans le respect des règles de l'OMC, c'est cet équilibre que le Conseil européen devrait refléter. Les chefs d'État et de gouvernement continueront leurs échanges réguliers sur la refondation de l'Europe, le thème choisi par le président, tout ce que pour ce conseil et celui de la fiscalité du numérique, la discussion portera sur la proposition que la commission rend public aujourd'hui même de taxer les GAFA en prenant une part limitée des revenus générés par leurs activités numériques en Europe. La France, vous le savez, portent fortement ce dossier avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Même si ces discussions sont toujours difficile. Et s'il faudra sans doute à terme un cadre international, chacun voit bien qu'il y a un vrai enjeu européen pour réguler un secteur d'activité nouveau. Vendredi matin, les 27 chefs d'État et de gouvernement se réuniront en format article 50. L'enjeu est double : il s'agira d'abord de faire un état des lieux sur les négociations de l'accord de retrait. Ce projet d'accord reprend les 3 questions prioritaires traités en décembre, les droits des citoyens, l'Irlande et le règlement financier mais aussi les questions de gouvernance et la transition. Michel Barnier a fait état lundi d'importants progrès. Mais a aussi souligné qu'il restait des points a tranché ou à préciser, c'est le cas par exemple des marchés publics de la gouvernance de l'accord ou encore de la question irlandaise sur ce dernier sujet, le principe d'un alignement réglementaire, comme le proposait l'Union européenne est posée. Mais il n'y a pas de vision commune sur ses modalités. Londres espère dans ce contexte, pouvoir faire état d'un accord au moins politique sur la transition. Afin, principalement, de rassurer les investisseurs. Nos grands principes sont respectés, notamment la limitation dans le temps, au 31 décembre 2020 la pleine application de l'acquis et l'impossibilité pour le Royaume-Uni de continuer à participer au processus de décision. Le Conseil européen devra cependant, tout en saluant les progrès rappelé fermement que rien n'est agréé tant que tout n'est pas agréé. Le 2ème objectif des 27 sera de se mettre d'accord sur des lignes directrices qui permettront à Michel Barnier de négocier le cadre général des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous devons préserver une approche d'ensemble cohérente. Nous préférerions que les Britanniques restent dans le marché unique, ou dans l'union douanière à l'issue de la période de transition. Mais s'ils ne peuvent accepter les quatre libertés et qu'ils veulent pouvoir passer librement leurs propres accords commerciaux, le seul modèle possible pour l'Union européenne et celui d'un accord de libre-échange avec un équilibre à respecter entre les droits et les obligations qui s'y rattachent, cela implique que certains domaines, comme les services financiers feront l'objet de mesures autonomes de l'Union. D'autres thèmes pourront donner lieu à des accords spécifiques comme la coopération policière et judiciaire ou la politique étrangère et de sécurité commune tout en insistant sur la nécessité de respecter entièrement l'autonomie du processus de décision de l'Union européenne. Le Conseil européen devrait enfin mentionné la pêche, compte tenu de son importance et de la nécessité de trouver un équilibre entre accès aux zones de pêche et possibilité de vendre les produits de la mer britannique dans le marché unique. Sur ce secteur, le principe de l'accès des pêcheurs européens aux zones de pêche britannique pendant la période de transition, a bien été clairement clairement Les chefs d'État et de gouvernement serait une iront ensuite à 19 ans, format Sommets, zone Euro, la France propose une approche ambitieuse, qui consiste à avancer, à court terme sur l'Union des marchés de capitaux et l'union bancaire y compris en mettant en place un filet de sécurité, mais aussi en allant vers la création, à plus long terme, d'une capacité budgétaire propres de la zone Euro. Il s'agit de contribuer à une véritable stabilisation macroéconomique et de pouvoir maintenir les investissements dans des politiques qui soutiennent la productivité, en particulier en matière de recherche et d'innovation. Nous travaillons étroitement sur ces questions sensibles avec le nouveau gouvernement allemand nous sommes déterminés à suivre le calendrier défini par le président de la République et la chancelière et repris par le Conseil européen de décembre aussi, le président et la chancelière, ont-ils rappelé vendredi dernier que nous travaillons en franco-allemand a une feuille de route dans la perspective du Conseil européen de juin. Un rendez-vous franco-allemand est envisagé dès le mois d'avril, sans doute un autre en mai, vous voyez que nous sommes déterminés à avancer. Les chefs d'État et de gouvernement évoqueront dîner les questions internationales les plus urgentes, ils marqueront leur totale solidarité avec le Royaume-Uni, après l'attaque de source dont tout conduit à penser que la Russie est responsable. Sur les Balkans occidentaux nous souhaitons bien distinguer ce qui relève du processus d'élargissement. Qui doit rester très exigeant et où les conditions pour progresser, ne semble pas encore rempli et l'appui qui peut et qui doit être à ces pays sous la forme d'un d'agenda positif pour les idées pour les aider dans leurs réformes, ce sera tout l'enjeu du sommet du 17 mai prochain à Sofia. Il est enfin possible qu'une discussion s'engage à nouveau sur les actions menées par la Turquie en mer Égée, tant vis-à-vis de la Grèce que de Chypre, je me tiens maintenant à votre disposition pour vous écouter, répondre à vos commentaires et à vos questions, je vous remercie. J'indique au Sénat que la conférence des présidents a décidé d'attribuer un temps de parole de 8 minutes aux orateurs de chaque groupe politique et de 5 minutes à la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées, la commission des affaires européennes et la commission des finances, interviendront ensuite durant 8000 minutes chacune le gouvernement répondra aux commissions et aux orateurs, puis nous aurons pour une durée d'une heure maximum une série de questions avec la réponse immédiate du gouvernement ou de la commission des affaires européennes, c'est-à-dire que tout sénateurs présents dans l'hémicycle, pourra intervenir s'il le souhaite, dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes

Monsieur le Président, Madame la ministre, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, nous sommes face à une actualité donc européenne et internationale extrêmement dense, je souhaiterais évoquer en préambule de fait qui rappelle combien même dans un monde devenu multipolaire, les agissements des États-Unis et de le la Russie nous préoccupe toujours au 1er plan, tout d'abord le président Donald Trump il vient d'exiger donc à l'Union européenne un abaissement des de des barrières douanières et réglementaires sur les produits américains et la taxation comme ça a été cité sur l'acier et l'aluminium en matière d'importation, j'espère que la commissaire Cécilia Malström donc actuellement à Washington, trouvera une issue favorable à ce dossier, ensuite je voulais également souligner la réélection donc du président Poutine une donnée, quoiqu'on en dise, et quoiqu'on en pense, avec lequel notre diplomatie doit travailler comme elle l'a déjà fait la Russie détient néanmoins, on le sait, une des clés de la résolution du conflit syrien l'actualité récente nous également évoquer la montée du populisme en Europe, les dernières élections italiennes confirment, hélas, un score du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue, c'est une réalité politique qui occulte cependant à tort les vrais attendu et les vrais attentes d'une majorité de citoyens européens, ce n'est pas moins d'Europe mais plus d'Europe qu'ils veulent pour faire face à des défis, dont on sait que la seule dimension nationale ne suffira pas à les résoudre, je pense en particulier au phénomène migratoire qui sont l'intention l'intervention de l'Union européenne aurait débouché et débordé surtout encore un peu plus les payer les États-membres en première ligne en première faut-il en effet rappeler à tous ces partis eurosceptiques que le repli sur soi, n'est pas la solution dans un monde telle qu'il est aujourd'hui, en réponse à la crise migratoire là l'Europe a mené un certain nombre de politiques qu'il faut poursuivre et approfondir, que ce soit donc le développement de la coopération avec les pays d'origine, où transitent. Le renforcement du contrôle aux frontières extérieures ou encore la gestion des des flux par des dispositifs quelques le tels que les accords de réadmission, je n'oublie pas la réforme, donc de la du régime d'asile européen sur lequel il faudra encore avancer le Conseil européen est censé pas parvenir à mettre au point une politique migratoire durable d'ici juin 2018, espérons qu'ils y parviennent à qu'il y parvienne, mais pour cela il faudra que les États-membres et la même vision de l'Europe, celle d'une communauté de destin et non pas celle d'un simple marché unique j'viens ainsi au Royaume-Uni, un pays qui a voulu jouer sa propre carte du destin mais qui essaie aujourd'hui de ne pas trop se couper de l'Europe. Il sera bien sûr largement question du Brexit au prochain conseil européen comme vous le savez, mes chers collègues, il me reste il nous reste, le traité de sortie un nouveau traité bilatéral et la période tranche de transition entre les 2 statuts, force est de constater que la marge de manoeuvre entre la ligne rouge britannique et les principes fondamentaux de l'Union européenne est extrêmement étroite 3 points sont essentiels et nous sommes nombreux à y à y tenir, je crois, je citerai la garantie des droits des citoyens européens résidant au Royaume-Uni, et des citoyens britanniques sur le territoire de l'Union. Ensuite, concernant la solution de la question irlandaise et enfin le règlement financier avant hier une étape, a néanmoins été franchi avec un accord entre Londres et Bruxelles, sur la période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni bénéficieraient des avantages du March est unique, nous pouvons y adhérer, car personne n'a au fond intérêt une relation déséquilibrée avec un pays qui reste malgré tout lié à l'histoire de l'Europe est un partenaire commercial important d'autres sujets majeurs que je souhaitais aborder la fiscalité donc numérique à ce jour, comme on le sait, de critères ont été arrêtés la taxe viserait les entreprises qui se présente comme un réseau social ou celle qui se présente comme une plateforme d'échanges, les rentrées annuelles devraient se pourrait donc atteindre entre 5 et 8 milliards d'euros par un parent à l'échelle de l'Union européenne, c'est une bonne chose au regard des enjeux budgétaires de l'Union européenne, au-delà de l'aspect financier, on ne peut que partager l'objectif qui consiste à envoyer un signal politique aux citoyens de l'Union européenne en leur prouvant la détermination de Bruxelles à lutter activement contre les le l'injustice fiscale je voudrais poursuivre mon intervention sur les perspectives de l'Union européenne, près de 60 ans après le traité de Rome. Profitant de l'amélioration de la conjoncture économique pour oser une véritable refondation de l'Union européenne, même si la fenêtre est limitée, compte tenu des élections prévues en 2019 la France et l'Allemagne ont promis une impulsion commune pour réformer la zone Euro est relancé, l'Union européenne, on ne peut que s'en réjouir, la grande coalition re nouvellement réinstallée autour de la chancelière Merkel pour nous y aider. Lors du discours de la Sorbonne en septembre dernier, le président de la République a affirmé que les défis lancés par l'Union européenne et à ses États-membres exigeait de faire revivre une ambition politique européenne sur le plan interne comme sur le plan externe, le groupe RDSE partagent cette volonté pour cela, il faut que soit défendu nos valeurs, nos préférences collectives nos intérêts communs, tant sur le plan géopolitique, économique, c'est le sens de la, de l'c'est le sens, donc de l'Europe souveraine défendre par le président de la République, cette défense de nos préférences collectives je souhaitais y revenir s'agissant en particulier de l'agriculture, comme vous le savez, madame, madame la ministre, les agriculteurs ont fermement exprimé des craintes quant à leur avenir lors du ce récent Salon de l'agriculture, le groupe RDSE restent très vigilants dans le cadre des accords de libre-échange que négocier absolument le l'Union européenne, le Sénat est d'ailleurs très mobilisée sur ces accords en prenant régulièrement l'initiative de propositions de rêve, solution européenne invitant à la protection de nos filières agricoles les plus fragiles, c'est le cas de celle du RDSE, porté par le président Ruquier concernant les échanges européens avec le maire Enfin, en tant que sénateur d'un territoire rural, je voudrais relayer les inquiétudes de nos agriculteurs sur la réforme de la PAC, même si cela n'est pas à l'ordre du jour du Conseil européen, les sénateurs du groupe air de se sont opposées à toute renationalisation la PAC ne doit pas être une variable d'ajustement budgétaire le C2 commun nous semble essentiel et non négociable le cadrage financier prévu en mai prochain nous permettra sûrement d'y voir plus clair et j'espère, de ne pas sacrifier ceux qui ont contribué à la richesse et au progrès de l'économie économique de l'Europe, pour conclure, je souhaitais donc rappeler que la construction européenne est consubstantielle au groupe RDSE et je réaffirme donc il faut plus d'Europe mieux d'Europe et c'est la solution à ce monde tourmenté, comme si on emploie très bien le président de la République à qui nous apportons notre soutien sur le projet européen je merci, je vous remercie de votre attention, merci. La parole est à madame Fabienne Keller pour le groupe. Les républicains pour une durée de 8 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues. Permettez-moi dans ce débat préalable au conseil européen qui aura lieu demain et vendredi d'aborder plus particulièrement 3 sujets : le 1er sera le Brexit le second, la zone Euro et le 3ème, les questions fiscales, avec un focus d'actualité sur les gaffes, le Brexit, vous l'avez rappelé : Madame la Ministre, ce sera dans point important abordé lors de ce Conseil européen, il y a beaucoup de discussions qui se déroulent dans les dernières semaines, vous avez rappelé le compromis qui vient d'être retrouvé autour de la date du 31 décembre 2020 pour la fin de la période de transition, l'Union européenne a obtenu gain de cause sur pas mal de d'éléments qu'elle défendait le droit des citoyens européens, mais aussi la non-participation du Royaume-Uni aux décisions politiques pendant la période de transition, mais l'Union a aussi fait des concessions concernant le règlement des différends qui, si j'ai bien compris sera renvoyé à un comité mixte et non à la Cour européenne de justice comme nous le souhaitions, le projet des lignes directrices pour définir le cap de la future relation entre l'UE et le Royaume-Uni annonce d'âpres négociations, vous l'avez rappelé.

elle pose des conditions, puis Donald que vous avez repris cette position, a affirmé que seul un accord de libre-échange était possible, un accord qui couvrirait les biens mais qui ne dit mot sur les services financiers, madame la ministre, est ce que vous pouvez nous indiquer ce qui s'est passé hier dans la réunion ministérielle concernant l'inclusion des services financiers au futur accord c'est évidemment un sujet important pour, en particulier le développement des services financiers à Paris et dans l'Europe des 27 à la suite de la sortie dès le Royaume-Uni 2ème point que je voudrais évoquer sur le Brexit, c'est ce sujet tellement délicat de l'Irlande du Nord, c'est un point sensible de la négociation, nous le savons tous, c'est la seule frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, l'objectif de base était d'éviter une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande pour maintenir l'accord du vendredi Saint, dont je rappelle que c'est le dernier accord de paix de l'Union européenne, il a à peine une vingtaine d'années, la conclusion qu'en ont tiré les négociateurs européens pour protéger l'intégrité du marché unique et la nécessité pour l'Irlande du Nord de ne pas s'éloigner du cadre réglementaire communautaire, or un important désaccord a vu le jour sur ce point lors du projet d'accord de retrait l'Union proposait de conserver l'Irlande du Nord dans l'union douanière, si les négociations n'aboutissaient pas à un accord, proposition initialement rejetée par le Royaume-Uni mais le 1er ministre semble évoluer sur ce point en acceptant peut-être cette solution comme dernier recours, madame la ministre est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette situation très délicate : les représentants britanniques, la future coopération en matière douanière puisse être suffisante et suffisamment puissante, pardon pour éviter le retour d'une frontière physique ou le déplacement de la frontière en mer d'Irlande, tout en préservant les intérêts européens, alors même que les Britanniques souhaitent quitter l'union douanière. Plus largement, quelle est la stratégie du gouvernement français en coopération avec les 26 autres États partenaires de manière plus générale, hein, dans ces négociations pour qu'elle progresse progresse de manière favorable, je voudrais ici souligner le rôle tout à fait remarquable que mais parfois difficile, assure le grand négociateur Michel Barnier 2ème sujet : la zone Euro, vous l'avez rappelé en raison des élections allemandes le projet franco-allemand pour la réforme de la zone Euro ne sera pas présenté lors de ce conseil, vous avez d'ailleurs indiqué qu'il y aura de sommet franco-allemand prochainement et je voudrais m'en réjouir, ils traiteront de cette question, mais peut-être plus largement de l'avenir de l'Union européenne sur la zone Euro, je voudrais insister sur 2 points : l'union bancaire et le parlement de la zone Euro le 1er l'union bancaire, je rappelle qu'il comporte 3 piliers qui ont pour but de limiter les risques de défaillance des banques européennes et de protéger les épargnants. Suite à la crise que nous avons connu ces points sont fondamentaux jour, or aujourd'hui, Madame la Ministre, il semblerait qu'un certain nombre de difficultés techniques, mais qui sont, nous savons bien technique cache toujours politique a plutôt des difficultés politiques semblent mettre en péril un accord est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus 2ème sujet : le parlement de la zone Euro, c'est un point qui me tient à titre personnel, très à coeur, avec le président Vincent et blé, président de la commission des finances, nous avons participé, le 19 et le 20 février dernier à la conférence, article 13 qui fait le point sur le semestre européen, je rappelle que cette conférence réunit des représentants des commissions des Finances des parlements nationaux, et aussi des parlementaires européens et des membres de la Commission européenne, donc c'est un lieu d'échanges particulièrement intéressant, les échanges sont sont riches utile on, cela permet de mieux comprendre les positions des différents États membres mais à ce stade, cela ne conduit à aucun avis concret à aucune prise prise de position, c'est pour cela, madame la ministre, je voudrais ici soutenir la création d'un parlement de la zone Euro n'ont pas de nouveaux élus mais des élus des parlements nationaux, du Parlement européen et la Commission aidés commissaire qui ainsi constituerait un lieu de dialogue, d'échanges au niveau européen et national et qui trouveraient naturellement son lieu de réunion à Strasbourg capitale européenne. L'objectif c'est bien sûr de mieux coordonner les politiques économiques et monétaires des pays de l'Union européenne et d'assurer la coordination des travaux à l'échelle nationale et européenne, que le représentant du Bundestag, présents à cette réunion, article 13 a salué cette idée et là clairement soutenu, madame la ministre est-ce que vous pourriez nous indiquer si ce projet progresse et plus globalement, quelle est la position du gouvernement français concernant le parlement de la zone Euro, dernier point, la fiscalité. Je voudrais traiter le sujet GAFAM mais surtout l'Axis l'Assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, ce projet d'assiette commune qui est en quelque sorte, préparatoire à la convergence des taux, hein, ça a été relancé en 2006 par la commission adopté au Parlement européen le 15 mars dernier suite au rapport de notre collègue député européen Alain Lamassoure laxistes, c'est un ensemble de règles communes en terme d'imposition pour les entreprises des 27 l'idée c'est de limiter l'intérêt à des délocalisations de résultats de valeur ajoutée de de marge d'un antre des pays de l'Union européenne, ça permettrait d'avoir un système unique et donc d'harmoniser l'assiette fiscale entre les États membres et d'éviter des niches, des exemples des exemptions, des avantages fiscaux, créant un différentiel entre les petits S'agissant plus particulièrement des GAFA donc le commissaire européen, Pierre Moscovici a annoncé tout-à-l'heure me semble-t-il, qu'il progressait, j'imagine que ce sera discuté au lors du conseil qu'il proposerait demain la taxation à 3 pourcent du chiffre d'affaires des entreprises à partir d'une certaine je rappelle qu'il est également proposé notamment par Alain Lamassoure, que le projet Axis intègre une disposition spécifique pour c'est gaffe de manière à pérenniser la possibilité de les fiscaliser, mais en tout cas cette fiscalité plus juste, plus équitable, être un sujet très sensible pour Nos concitoyens et une règle mieux respectée harmoniser être attendu par l'ensemble des Européens, Madame la Ministre, là aussi, est ce que vous pouvez nous faire un point sur ce dossier en tout cas je vous remercie tous pour votre écoute. La parole est à Monsieur André Gattolin pour le groupe, la République en marche, il a 8 minutes aussi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le Conseil européen qui se tiendra les 22 et 23 mars prochain restera peut-être dans les annales de l'institution, il est certes à ce jour, difficile de présumer que son caractère particulier dépendra de l'importance des décisions qui seront prises, mais une chose est certaine, c'est que ce conseil sera particulier au moins par sa forme et la nature des questions qu'il sera amené à soulever sa forme tout d'abord, il entérine, dans les faits, l'idée que l'Union ne peut, aujourd'hui avancer qu'à plusieurs vitesses, en effet, ce conseil débutera dans un format à 28 avant de passer rapidement dans un format à 27 sans le Royaume-Uni pour s'achever à 19 au format propres qui est celui de la zone Euro, nous faisons donc au niveau du conseil, ce que nous rechignent encore à faire, Clermont au niveau de la Commission et du Parlement européen, c'est-à-dire un processus de discussion et de décisions qui soient bien distinctes entre les États membres les plus intégrés et les autres, ce conseil sera aussi particulier dans sa forme en ce que son ordre du jour et pour une fois relativement restreint, en tout cas plus raisonnée et moins hétéroclites dans les sujets à aborder que lors des conseils passer la démocratie gagne toujours en clarté et en lisibilité de ses choix sur le fond, ce conseil ne pourra cependant pas manqué d'évoquer la soudaine et brusque tension diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie suite à la tentative d'empoisonnement à Salisbury, à l'endroit de Sergueï et lieu Ioulia Skripal la réaction britannique à cette énième tentative d'assassinat, laissant planer une intervention des services russes a été forte, très forte et d'une ampleur sans précédent depuis la fin de la guerre froide, le 14 mars la première ministre Madame Theresa May annoncé, en effet, l'expulsion de 23 diplomates russes le lendemain des gouvernements français, allemands et américains exprimaient leur c'est de solidarité avec Madame May dans la foulée, la ministre de l'intérieur britannique Madame Rambert relate. Accueillait favorablement la demande parlementaire de réouverture des enquêtes sur pas moins de 14 décès suspects survenus sur le territoire britannique au cours des 15 dernières années, dans ce contexte, nous ne pouvons pas nous empêcher d'en tirer 2 enseignements importants 1er renseignement malgré sa décision tonitruante de quitter l'Union, le Royaume-Uni n'est pas une île et il sur ce sujet d'ailleurs, comme sur bien d'autres besoin du soutien et de la coopération de ses alliés européens et chaque jour qui passe, ne manque pas de rappeler aux autorités britanniques, cette vérité qui dérange 2ème enseignement cette affaire à un site mon l'Avantage de ressouder un peu politiquement l'opinion britannique, mais aussi la majorité et le gouvernement de Madame Theresa May sérieusement mise à mal, il faut le dire par les divergences de plus en plus nombreuses quant à sa gestion post-référendaire du pays en creux l'affaire Skripal met cependant en lumière la mansuétude coupable dont les gouvernements britannique se ce successifs se sont rendus coupables, à une époque où leur objectif principal était d'attirer massivement sur son territoire, et en particulier sur la place de Londres, les investissements de quelques Ligue peu recommandables la réalité qui se fait jour aujourd'hui, c'est que le Royaume-Uni, contrairement à ce que disent ces médias et une grande partie de sa classe politique n'a pas souffert de trop d'Europe mais de son attitude de cavalier seul en Europe et de son manque absolu de vision sérieuse de sa place au sein de l'Union, car ce que l'aventure inédite du Brexit met en lumière, très concrètement, aujourd'hui c'est le coût réel de la non-Europe alors certes, l'Union européenne est loin d'être parfaite et nous sommes les premiers à appeler à sa refondation, certes, et du fait même de son caractère institutionnel et politique complexe et inachevée, elle a du mal à répondent simultanément à toutes ces crises qui la traverse et à relever tous les défis auxquels elle est confrontée aussi nombre de voix s'élèvent partout en Europe pour dire que l'Union européenne aurait finalement échoué à réaliser son credo fondateur, celui d'instaurer durablement un espace de paix et de prospérité sur le continent européen, c'est vrai, des tensions de plus en plus nombreuses émergent ou re-émerge ces dernières années au sein de l'Union entre certains de ses États-membres ou même à l'intérieur de-ci comme en Catalogne en Flandre ou en Ecosse, c'est vrai aussi que depuis la crise financière de 2008, la croissance dans l'Union européenne et là, dans la zone Euro demeure assez atone au regard de celles observées par ailleurs dans d'autres pays, notamment aux États-Unis et surtout dans les pays émergents, mais c'est oublier un peu vite le rôle majeur joué par l'Union, non seulement en matière de réconciliation franco-allemande, tout ça et de acquis mais aussi de consolidation démocratique de pays comme l'Espagne ou le Portugal, son rôle joué dans la réunification allemande dans la réconciliation entre l'Ouest et l'Est de l'Europe dans la pacification des des Balkans orientaux et Lens battre notre liste, la fin de la guerre civile en Irlande du Nord, sur ce dernier point, le blocage idéologique et souverainiste dont souffre encore le gouvernement britannique dans les négociations actuelles sur les questions de frontière irlandaise va à l'encontre de la réalité réalité historique, c'est-à-dire le poids et le rôle capital joué par l'Union dans le règlement de cette guerre civile au relent de guerre de religion en réalité, on peut le dire, cette réalité a été écrite, elle était écrite même noir sur blanc dans un très récent rapport de décembre 2016 rédigé par nos collègues de la Chambre des lords et qui soulignait, qui rappelait le rôle majeur de l'UE dans le processus de paix au vu notamment, je les cite des garanties apportées par l'Union dans l'application concrète des accords de belles phases de 1998 de son effet, l'effet de l'Union européenne sur la transformation des relations bilatérales entre les 2 Irlande et dans la présents au moment des tensions communautaires en Irlande du Nord et de l'impact distille considérable qu'ont eu, et que continuent d'avoir les financements européens en or en Irlande du Nord, alors oui c'est incontestable l'appartenance à l'Union est encore et toujours source de pacification, souhaitons que Madame May revienne vite à la raison et qu'elle accepte la proposition juste et mesurée, faites par les négociateurs européens sur la question irlandaise, l'Union, espace de paix donc, mais aussi et toujours espace de prospérité, certes il faut bien le dire, cette prospérité est à présent relative et assez fragile aussi la relancer est indispensable, c'est notamment pourquoi la France propose de renforcer la zone Euro d'harmoniser les politiques fiscales et industrielle de taxer les revenus des grands groupes du numérique, mais le coût d'une future non-appartenance à l'Europe s'observe aujourd'hui déjà très concrètement dans l'évolution récente et à venir de la croissance au Royaume-Uni, il avait en effet déjà loin le temps pas si lointain que ça ou en 2014, l'ex-1er ministre monsieur David Cameron plastronnait et promettait la tenue d'un référendum sur le maintien ou non dans l'Union, cette année là, en 2014, le Royaume Uni affichait une insolente croissance avec une progression de plus 3 virgule un pour 100 de son PIB quand la zone Euro n'était qu'à un virgule 3 et les cours ne cessent de se prolonger puisque aujourd'hui toutes les prévisions pour les années à venir, monde qu'il y aura un différentiel important au bénéfice de la zone Euro, j'espère, Madame la Ministre, qu'à l'occasion de ce Conseil européen, la France et ses partenaires auront de ramener nos amis britanniques à plus de rap de raisons en le rappelant peut-être cette belle formule du grand écrivain anglo-australien Arthur au fil de ce que l'on croit n'a aucune importance, seuls les faits comptent, je vous remercie. La parole est à monsieur Pierre Ouzoulias ce pour le groupe CRCE il à 8 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, au 1er temps de la République romaine au début du Ve siècle avant notre ère, à plusieurs reprises la plèbe décida et organisa sa sécession en se rassemblant hors de la ville pour protester contre les abus de pouvoir des patriciens le poids des dettes qui pesaient sur elle et son exclusion des magistrature en s'insurgeant de la sorte elle voulu montrer son opposition à une forme de gouvernement qu'il excluait et qu'il ignorait son souhait d'être mieux associés à la vie politique de la cité, vous me permettrez de considérer que les électeurs italiens viennent de manifester par la radicalité de leur vote, une forme moderne de retirement. à l'occasion de ce débat, il nous incombe de comprendre pourquoi le rejet de l'Europe est devenue dans ce pays fondateurs de l'Union, le socle commun des extrémismes et de la xénophobie, d'autant plus que le séisme politique qui vient de toucher l'Italie s'ajoutent à ceux qui ont déjà ébranlé l'Allemagne, l'Autriche, la Léttonie, la Hongrie, le Danemark, la Suède, la Slovaquie dans tous ces pays, une extrême droite résolument racistes et anti-européenne s'est solidement installé dans les parlements et parfois dans les gouvernements au délitement de l'eau, de l'idée européenne fondée sur la démocratie, la paix, les droits de l'homme et la solidarité, elle oppose la fermeture des comptes des frontières, la chasse aux étrangers le repli identitaire et souvent la volonté de constituer de nouvelles entités nationales au-delà ou en deçà des limites actuelles des États, des élections européennes se dérouleront dans un peu moins d'un an en mai 2019 chers collègues tremblons à l'idée de moins en moins invraisemblable que ses forces puisse devenir la principale composante du futur Parlement européen comment en est-on arrivé là, comment l'Italie, pays connu depuis toujours comme l'un des plus actifs partisans la construction s'en éloigne aujourd'hui avec tant de violence, d'aucuns ont estimé, non sans raison que l'afflux de réfugiés dans la péninsule, avait contribué à déstabiliser une société déjà fragilisée par la crise, il est vrai que l'Italie, comme la Grèce, ont dû gérer cet accueil sans grande aide de l'Union européenne, dont la plupart des membres leur ont refusé toute forme de solidarité. Les organisations non gouvernementales évaluent à plus de 10000 le nombre de réfugiés qui vivent en Italie dans des campements de fortune, sans aucune aide, malgré les appels du pape, François, qui exhorte les Italiens allaient recevoir dignement, parce que je le cite : les pauvres sont notre trésor, la peur de l'étranger est devenue la manifestation d'une opposition radicale à la globalisation dans sa variante européenne et de ses conséquences toujours plus destructrices parcouraient l'Italie du sud de la Sicile et comprenez à la vue de leurs innombrables friche industrielle que le mal est là, dans ces tissus économique totalement déstructuré par 30 années d'une crise sans fin, la carte électorale de l'Italie et aujourd'hui celle de la pauvreté : celle des régions en voie de sous-développement, celle de l'exode des jeunes diplômés vers le nord dans un mouvement similaire à celui qui avait poussé hors du pays, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents, au-delà de ces Terres du Sud partout en Europe, vous trouverez des régions entières, subissant le même déclin et manifestants vis-à-vis de l'Union, le même dédain ainsi, pour les mêmes raisons, les mines lance britannique accablé par la perte de leur industrie ont voté massivement en faveur du Brexit dans le Royaume-Uni, la production manufacturière ne représente plus que 9 pourcent et son recul a été le plus dévastateur dans ces régions qui constituait jadis le coeur historique de la révolution industrielle pour leurs chômeurs ce déclin est associé à la construction européenne et il aurait parfaitement indifférent que la City perde son passeport financier à la suite du Brexit tant le destin de cet îlot de richesse l'est devenue, aujourd'hui, étrangers en France des processus similaires sont à l'oeuvre et je vous rappellerai que depuis 40 ans, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière dans l'économie a été divisé par 2, ce reflux général à vider de leur substance, nombre d'anciens bassins industriels ces déclassements de régions entières sont les conséquences d'une redistribution géographique majeur de la production industrielle qui se réalise maintenant à l'échelle européenne de nombreux emplois parmi les moins qualifiés, ont migré vers l'Est de l'Europe et les productions à haute valeur ajoutée sont maintenant concentrés dans un petit nombre de pays de l'Europe du Nord qui ont maintenu puis renforcer leurs capacités dans ces domaines, ces emplois perdus ont rarement été remplacés par de nouveaux créés dans d'autres secteurs économiques, il en résulte de fortes disparités géographiques de la richesse qui ne cesse de s'accroître et qui mine les fondements d'une Europe qui ne peut se perpétuer sans être solidaire, l'Allemagne est souvent considérée comme la responsable de ces déséquilibres économiques parce qu'elle n'aurait parce qu'elle aurait imposé une politique économique et monétaire favorable à ses seuls intérêts la critique est en partie injuste car son gouvernement a soumis son pour son propre peuple au même ordolibéralisme avec les mêmes conséquences sociales dans son rapport du 7 mars dernier la Commission européenne, note ainsi que la faiblesse de la demande intérieure et la stabilité des salaires, associée à une production économique inférieure à celle de 2009 ont eu pour conséquence d'accroître considérablement les inégalités sociales et la pauvreté en Allemagne des riches, des richesses de ce pays sont détenus par 10 pourcent de la population, alors que la moitié des ménages, les poules Pauvre n'en détient plus que 1 pourcent l'emploi à temps partiel a beaucoup progressé et surtout près de 3 millions de travailleurs sont obligés d'exercer un second emploi pour vivre de façon synthétique, le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités de traitement place l'Allemagne au sommet des pays les plus inégalitaires de l'Europe face à cette crise de l'Europe, une nouvelle fois le renforcement de la relation franco-allemande nous est proposé comme la seule solution possible, elle est sans espoir, sans analyse radicale de l'ordolibéralisme instituer comme principe régulateur de l'Espace économique européen, cette doctrine impose l'équilibre budgétaire, l'indépendance monétaire, il y a un un niveau élevé de concurrence pour mettre l'entreprise au service de la société et aux Frères et offrir soi-disant ainsi à chacun de ses membres, la faculté d'y prospérer, alors que le 21ème siècle nous est présenté comme celui d'une aire sans idéologie, il est urgent d'abandonner ce dogme dans l'état social de l'Europe monte qui nous conduit aujourd'hui à l'abîme notre union n'a pas besoin de grandes déclamations depuis la colline de la technique s'ou l'amphithéâtre de la Sorbonne pour convoquer les mânes des pères fondateurs de l'Europe, si nous sommes incapables de comprendre qu'il nous faut trouver d'abord dans l'urgence de la taille de la catastrophe qui vient des moyens pour soulager le quotidien de millions d'Européens qui vivent dans ces territoires de relégation condamné par déçus des processus économiques qui les exclut, ayons l'audace salvatrice d'affirmer dans les discussions à venir que le seul horizon pour sauver l'Europe est celui de la réduction des inégalités, des politiques en rupture avec les dogmes de l'ordolibéralisme sont expérimentés en ce moment, elles prouvent par leur succès, qu'il est possible de concilier le développement, la redistribution de la richesse et l'indispensable solidarité entre les individus et les territoires j'achève sortons de la pensée unique pour poser les bases d'une analyse rigoureuse des camps social des politiques économiques replaçons maintenant l'humain et la société au coeur de nos préoccupations, soyons humaniste pour tenter d'éviter que l'Europe de demain ne soit plus qu'un espace dédié à la libre circulation des marchandises et livré aux forces anti-démocratiques, La parole est maintenant à monsieur Philippe Bohn Carrère pour l'Union centriste. Il a 8 minutes. Oui, Monsieur le Président, Madame la ministre mais, chers collègues, le président de la République a demandé et obtenu la confiance des Français sur un programme faisant une large place à la construction européenne à l'affirmation de notre communauté de destin, il a, à plusieurs reprises exprimé l'ambition européenne de notre pays, une exigence Ilana présenté les fondements intellectuels historique, mais aussi en a tracé des perspectives lors de son discours de la Sorbonne, auquel vous avez fait là référence à la veille du Conseil européen, le soutien à l'action européenne du président de la République est plus que jamais nécessaire, mon propos n'est pas simplement l'expression d'un soutien au président de la République, même si je l'assume volontiers, il est aussi l'expression des intérêts de notre pays, nous pouvons chers collègues aisément mesurer l'imbrication des enjeux français et des enjeux européens par le nombre, la diversité, l'importance des sujets que vous avez évoqué les gens et les autres à l'issue de l'intervention de Madame la Ministre, ceci illustre assez bien vos attentes, ce que vous avez appelé suivant des formules différentes, le coût de la non-Europe l'espoir d'un plus d'Europe ou d'une autre Europe, quelle que soit, en tout cas les points de vue qui ont été exprimées, suivant les les bancs ainsi le rouge, me semble-t-il, dans vos interventions, une forme de gravité de gravité peut-être un petit peu plus lourde que ce que nous avions pu entendre lors des débats de ce type, la République romaine, voir l'empire Romain, puis les mythes lance du 19ème de la 2ème moitié du XIXe siècles ont été rappelés à notre attention et je partage, chers collègues, l'intérêt de cette mise en perspective historique, je dois crever même indispensable, j'aurais quand même tendance à y rajouter que c'est tout à l'honneur du travail qui a été fait depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a été fait par les gouvernements successifs de de l'Europe, quelle a été l'ampleur des chantiers et quelles en sont fort heureusement les résultats, il est important de conserver cette perspective historique, y compris sur le couple franco-allemand dont on nous disait il y a quelques secondes qu'il était sans reste foire, j'aurais tendance à considérer qu'il est justement plein d'espoir et en tout cas, il est de nouveau opérationnel avec un axe européen marqué dans le contrat de grande coalition, mais aussi des prudences rédactionnelle qui font que, entre ambition européenne et prudence rédactionnel, il peut y avoir quelques inquiétudes sur les risques de statu quo et d'une certaine manière, je crois qu'il faut faire attention à passer au-dessus des formules de Style compte au couple franco-allemand, c'est bien sûr un élément essentiel, mais au-delà de la formule, il convient de souhaiter, de faire en sorte que le contenu soit à la hauteur des enjeux dans les mois qui viennent, le thème même du conseil autour de l'emploi, de la croissance et de la compétitivité pourrait inciter à une forme de statu quo quelques craintes à cet égard, tant pour certains et notamment pour les pays du nord de l'Europe dans la durée, l'Union européenne apparaît comme une forme d'îlot de stabilité et de prospérité, du moins par rapport au malheur du monde, mais rien n'est acquis, vous le savez, en particulier pour notre pays qu'il a devant lui de nombreuses réformes à mener et nos partenaires, nous le rappellent régulièrement pour regagner une position de leader économique en Europe, que nous n'aurions jamais dû quitter et réduire notre taux de chômage comme l'ont fait avec succès plusieurs de nos voisins, c'est dire, chers collègues, que la politique économique de la zone Euro, sa gouvernance l'union bancaire le marché unique des capitaux Santana tente de décisions que la convergence fiscale sur laquelle plusieurs d'entre vous avez insisté État mettra 9 depuis les taux de l'impôt sur les sociétés en passant par les rescrit fiscaux, sans oublier la fiscalité du numérique qui faut confine à la caricature pour Google qui paieraient un impôt 9 pourcent de son chiffre d'affaires hors de l'Union européenne, à comparer avec un minuscule 1 pourcent 0 92 pourcent, paraît-il, dans l'Union européenne là où Facebook réussirait la performance de descendre à moins de 0,10 la question des droits de douane est venu se rajouter à ces difficultés avec les initiatives individuelles des USA qui sont graves par leurs conséquences européennes et qui sont surtout grave

plus stratégique, avec en particulier la question de l'accord sur le nucléaire autour de l'Iran et la Deadline, qu'il y a au 12 mai à cet égard, vous comprendrez madame la ministre que pour mes collègues, comme pour moi-même la voix de l'Europe et particulièrement attendu sur ces différents sujets c'est dire aussi que le contexte géopolitique est très lourd du Moyen-Orient à la Russie de l'Ukraine à la mer de Chine et même pour ceux qui ont la foi européenne chevillée au corps, le découplage entre les enjeux géostratégiques, la montée en puissance militaire d'état continent et les précautions oratoires ou les pudeurs qui peuvent exister, Anne Europe autour de la politique par exemple de défense peuvent quelque peu agacé, mes chers collègues, finalement, à côté des enjeux économiques que j'évoquais rapidement, il y a quelques secondes des enjeux géostratégiques, l'Europe a des défis particuliers en matière de sécurité en matière d'immigration en matière de gouvernance économique en matière de sécurité beaucoup beaucoup de risques, que ça soit bien les questions défense ou les questions de lutte contre les terrorismes trouve maintenant leur véritable horizon de lutte ou de traitement au niveau de l'Europe et si on avait un seul doute je dirais l'obsession de nos amis britanniques à rester dans le cercle européen de la défense ou le cercle européen de la lutte contre le terrorisme est exemplaire, même chose bien sûr sur les enjeux en matière d'immigration, plusieurs d'entre vous avez rappelé qu'à ne pas traiter correctement ces questions ce qui se posait à des risques tels que ceux qui viennent d'être matérialisés électoralement en Italie cette situation n'est peut-être pas unique et nous la retrouverons d'une certaine manière, dans quelques semaines sur la réforme du droit de Gilles, qui fait l'objet de beaucoup de débats dans notre pays, bon, je dois dire que même encore une fois pour des observateur bienveillant vis-à-vis du gouvernement, elle peut paraître quelque peu surprenante, tant cette question du droit d'asile n'est plus une question franco-française et tente sa véritable place, être au niveau européen, vous avez évoqué la gouvernance économique démocratique j'aurais je souhaitais évoquer des consultations citoyennes comme l'importance de la conservation D vidéo D vidéo mais je dois désert la conclusion, conclusion qui ne conduira en tout cas Madame administre a souhaité que demain et après-demain, le Conseil puisse prendre dès décision le plus grave est aujourd'hui la des dunes d'être dans des situations de non-décision alors sans se désintéresser des des contenus, c'est vraiment une aspiration à ce qu'il y ait des décisions lorsqu'une feuille de route soit fixé, ce qui permet de répondre favorablement à la juste préoccupation me président de séance. Merci, la parole est à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le Conseil européen des 22 et 23 mars prochain se déroule dans un contexte où l'instabilité et les inquiétudes s'intensifie, la position de droite douane sur les importations d'aluminium a des été d'acier aux États-Unis ainsi que les tensions accrues avec la Russie tente encore davantage les relations diplomatiques en interne, l'Union européenne doit avancer tangibles ment sur des dossiers cruciaux qui détermineront son avenir à moyen terme, parmi lesquels, bien sûr, la question de son budget après 2020 la sortie du Royaume-Uni ou encore l'amélioration du dialogue social, ce conseil a donc un rôle majeur à jouer, en terme d'impulsion politique d'autant plus qu'il est situé à un an des élections européennes, il sera l'occasion de vérifier ni plus ni moins l'ambition des chefs d'État pour l'Europe, à un moment où il se révèle impérieux de conforter le pôle de stabilité, de solidarité et de protection qu'à l'Union européenne dans cette perspective, le profil du futur cadre financier pluriannuel de l'Union sera signe essentiel, en effet, le Brexit va créer un manque à gagner estimé entre 12 et 15 milliards d'euros par an, soit 10 à 15 pourcent des ressources propres de l'Union, en parallèle, la Commission et les dirigeants des États-membres n'ont de cesse d'exprimer leur volonté de voir l'UE monter en puissance sur un certain nombre de missions pour le moins non négligeables, c'est le cas, par exemple, nous le savons, en matière d'asile et de gestion des flux migratoires mais aussi de défense, de sécurité européenne de soutien à l'industrie, à l'innovation, autrement dit le CHP Post 20 20 est une équation : comment répondre à l'ensemble des défis toujours plus nombreux qui se posent à l'Union européenne sans la contribution du Royaume-Uni, la réponse logique voudrait qu'il faille augmenter le montant du budget actuel à cet égard, le Parlement européen vient de démontrer dans sa position adoptée très largement que pour remplir à minima, ses missions actuelles, de le de l'UE devrait être portée à 1,3 du PIB européen pour rappel, il est actuellement à 1 pourcent quand il représentait 1,25 pourcent du PIB de l'Union en 1999, or la Commission européenne sample aujourd'hui s'orienter vers un plafond maintenu à 1, voire 1,1 pourcent du PIB européen tandis que les États-membres à l'occasion du conseil européen informel de février dernier paraissait avoir acté une baisse des ressources du budget pour cause de Brexit qu'on ne peut pas faire plus avec moins, avoir une réelle ambition pour l'Europe aujourd'hui oblige à élargir les ressources propres de plus par delà les éventuelles hausses de contribution des États-membres, qui sont certes un signal, mais aucunement une solution pérenne, nous ne pouvons pas reporté, encore une fois les négociations sur cette thématique, c'est le moment idoine, par conséquent, Madame la Ministre, le gouvernement est-il prêt à appuyer l'idée du d'augmentation des ressources propres de l'UE, sans cela, ce sont les politiques européennes essentielles à la matérialisation du principe de solidarité qui risquent d'en subir les conséquences, la PAC et les politiques de cohésion au 1er chef et ce serait une erreur colossale, vous connaissez ici notre attachement au Sénat assez de politiques structurelles qui permet d'établir un lien Direct entre Bruxelles et tous les territoires de lutter contre le sentiment d'éloignement que peuvent ressentir les citoyens européens à l'égard de l'UE de tout simplement rendre concrète les valeurs, les avancées si nombreuses que favorise l'Union. Dans le climat actuel, caractérisé par une montée généralisée du populisme, ainsi que par une critique facile à l'encontre des institutions européennes, la PAC et les politiques de cohésion sont précieuses, il convient de les préserver à tout prix, tout en assurant à l'UE d'avoir les moyens de répondre aux nouveaux enjeux, il convient de ne pas oublier que le budget européen n'est pas uniquement un instrument financier, il est l'expression de choix politiques qui traduisent une ambition : nous avons besoin d'avoir des preuves de cette ambition et il est temps de convaincre, d'autre part, la réforme de la zone Euro, dont la feuille de route doit être adopté en juin prochain et l'occasion de marquer une ambition pour l'Europe, or, eu égard aux dernières réunions au niveau ministériel, les inquiétudes de taille peuvent poindre l'achèvement de l'union bancaire semble être en difficulté, en particulier sur la question clé du Fonds européen de garantie des dépôts, la réforme du semestres européen risque quant à elle, d'aboutir l'adresse, l'attribution des fonds de cohésion à la à l'aboutissement de réformes structurelles, les collectivités ne doivent surtout pas être tenus responsables des choix budgétaires des gouvernements alors avoir une ambition pour l'Europe c'est aussi regarder vers l'avenir, donc vers la jeunesse, le programme Erasmus, peut-être davantage que tout autre que de l'Union européenne a fait ses preuves et est reconnu de nombreux étudiants ont bénéficié bénéficie encore de cette ouverture à l'Europe de la richesse d'un séjour dans un autre pays membre et au retour de leur expérience, ils deviennent en quelque sorte des ambassadeurs de l'Europe et ils incarnent concrètement cette idée d'Union des peuples européens, ainsi il est heureux que les ministre de l'éducation et annoncé unanimement leur volonté de renforcer considérablement Erasmus, certains prônent un doublement de la dotation fixée à 14,7 milliards d'euros pour la période 2014, 2020, d'autres un triplement néanmoins au-delà de la problématique afférentes au montant du programme, il est intéressant de s'interroger sur l'ouverture d'Erasmus à alors 50 voire même je dirais au secondaire ou aux jeunes diplômés comme quelques États-membres le recommande surtout nous nous inquiétons du risque de substitution d'un système de bourses, un système de prêts individuels afin de tenir l'objectif d'un doublement d'Erasmus, nous aimerions avoir des précisions et des garanties du gouvernement sur ce point madame la Ministre car Erasmus Erasmus doit pouvoir profiter à l'ensemble des jeunes et non à certains et non à certains à quelques-uns qui aura un capital financier de départ plus substantiel enfin dans nos rangs, vous le savez, notre ambition a toujours été social, Jacques Delors a lancé ce mouvement indispensable car le marché unique sur le bien-être social des citoyens européens n'a que peu d'intérêt, et pourtant ce dialogue social européen cette amplement essoufflée ces 2 dernières décennies, c'est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir des récentes avancées qui consolide le pilier social européen, la proposition de la commission concernant la création d'une autorité européenne du travail était attendue, elle ne sera pas la résultant d'une fusion entre les agences existantes et aura comme principale tâche en tout cas dans l'immédiat, de garantir la libre circulation des travailleurs dans le respect des règles européennes en matière de détachement, dont la réforme, vous le savez, vient justement d'aboutir, la proposition sur la coordination des systèmes de sécurité sociale visant à améliorer l'accès à la protection sociale en élargissant l'ouverture à tous les travailleurs et en rendant plus effectif les droits sociaux des citoyens sont des objectifs qui donne tout son sens à l'Union européenne, protéger et améliorer le quotidien de chacun, les 20 principe du socle européen des droits sociaux programmés l'Automne dernier à soi cette finalité sociale de l'UE, sans attendre les actes juridiques européens qui donneront corps à ses principes, la commission a encouragé les États membres à les traduire une concrète au dans leur ordre interne, il en va de l'égalité entre les femmes et les hommes de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du dialogue social dans l'entreprise, en somme, 2 thèmes sociaux majeurs à l'actualité si contemporaine et aux incidences si multiple, je ne vous parle pas du congé de paternité, égalité salariale, rôle de l'entreprise, mais vous le savez, où en est le gouvernement dans la traduction nationale de ce socle européen enfin, mes chers collègues, ce Conseil européen n'est pas anodin, il permettra de jauger de l'ambition des États membres pour l'Europe et nous espérons que le président de la République sera mettre en conformité ses déclarations avec des engagements tangibles et élevé au service de l'UE et surtout au service de ses citoyens, je vous remercie. La parole est à madame Colette Mélot pour le groupe, les indépendants 8 minutes aussi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le Conseil européen des 22 et 23 mars sera d'une grande importance pour l'Europe économique et pour l'Europe sociale, il sera d'abord l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de lancer le fameux semestre européen en adoptant les priorités économiques de l'Union, fondé sur l'examen annuel de la croissance, le semestre européen est le principal outil de convergence des économies européennes et s'articule autour de 3 axes de coordination premièrement, les réformes structurelles qui vise principalement à promouvoir la croissance et l'emploi conformément à la stratégie Europe 2020, deuxièmement les politiques budgétaires dans le but d'assurer la viabilité des finances publiques, conformément au pacte de stabilité et de croissance, enfin, la prévention des déséquilibres macroéconomiques excessifs, sur ce point, je me réjouis de la récente décision de la Commission européenne de sortir la France de la catégorie des pays à déséquilibres macroéconomiques excessifs pour la première fois depuis 10 ans, le 6 mars dernier la commission a en effet publié son diagnostic annuel sur la santé des pays européens et la France a recueilli un satisfecit pour les réformes entreprises, cette nouvelle est encourageante. Mais, fait peser une responsabilité accrue sur le président de la République et sur le gouvernement pour poursuivre l'assainissement des finances publiques et les réformes de structure, par exemple, le niveau de notre dette publique l'aggravation continuelle de notre déficit commercial depuis plusieurs années, sont des points très préoccupant, qui devront faire l'objet d'action extrêmement ferme à court terme, lors de l'examen des lois financière de l'Automne, notre groupe a défendu cette logique de responsabilité budgétaire et de réformes structurelles ambitieuses, elle est pour nous, crucial pour retrouver notre crédibilité Anne Europe et la capacité d'entraînement politique qui nous a fait défaut ces dernières années ce Conseil européen sera donc éminemment économique mais son ordre du jour apporte également beaucoup d'espoir aux tenants d'une Europe plus sociale, plus juste et plus solidaire, je crois, un effet que ces 2 aspects de la construction européenne vont de Pair et que l'Europe sociale a trop longtemps été négligé au profit du marché unique, le primat du grand marché, a sans doute été une cause du désenchantement chante Mandé peuple que nous observons depuis plusieurs années, il est heureux que l'Union européenne tentent enfin de marcher sur les 2 jambes de l'efficacité économique et de la justice sociale l'une ne peut aller sans l'autre, un discours du pape Benoît XVI ce grand européen m'a beaucoup marqué en 2017 à Vienne devant le corps diplomatique, il évoquait avec attachement notre maison Europe notre modèle européen qui qu'il qualifiait d'ordre social qui conjugue efficacité économique avec justice sociale pluralité politique avec tolérance libéralités et ouverture, il a affirmé que ce modèle était menacée par une mondialisation qu'il ne s'agissait pas de combattre, c'est une illusion populiste mais de canaliser, de réguler pour préserver l'autonomie des plus fragiles et de bien-être des générations futures, je crois qu'il exprimait ainsi le sens profond du projet européen et le rôle historique de ces institutions, aussi je me félicite que l'ordre du jour social de ce Conseil européen soit fournie et ambitieux, la mise en oeuvre concrète du socle de droits sociaux et par exemple, une nécessité pour harmoniser les conditions de vie des travailleurs s'européen, la proposition de création d'une autorité européenne du travail et pour l'accès à la protection sociale est également une bonne initiative de la Commission, elle permettra de remédier aux failles du marché unique, tout un exploitant tout son potentiel pour la mobilité des travailleurs, sa mission sera d'encourager la coopération des États-membres en matière réglementaire d'échange d'informations et de médiation dans la continuité de l'initiative du président de la République sur le travail, détaché, la France devra soutenir la création d'une institution puissante et efficace au mandat élargi en matière de fiscalité numérique c'est toujours cette idée d'un équilibre entre l'efficacité économique et la justice fiscale qui devra présider aux mesures qui seront présentées lors du prochain conseil européen ce dossier complexe, il inclut de nombreux facteurs dans un environnement technologique changeant, il impose de trouver un équilibre politique entre encouragement de l'innovation et juste contribution aux charges communes les plus grands économistes du monde dont le prix Nobel français Jean Tirole ont admis que la fiscalité de l'économie numérique est un grand défi contemporain, il s'agit bien ici de prendre en compte des modèles économiques en réseau qui échappe par nature à la territorialité de l'impôt et qui profite de surcroît de la concurrence fiscale entre les États membres de l'Union, cette question est l'exemple parfait de pourquoi nous avons besoin de plus d'Europe, seule une Union européenne unie, solidaire et parlant d'une seule voix sera capable de peser face aux géants du numérique américain et demain chinois je terminerai donc par ce dernier point. L'Europe doit être plus efficace, je l'ai dit, elle doit être plus plus juste, je l'ai rappelé mais celle doit être également plus unie et plus forte pour défendre ses valeurs et ses oeufs et ses intérêts dans le monde, avec le départ du Royaume-Uni, la France se doit plus que jamais entraîné l'Union européenne vers un avenir de puissance notamment avec nos partenaires et amis allemands, le 55ème anniversaire du traité de l'Élysée, que nous avons fêté il y a 2 mois, a d'ailleurs démontré la volonté du président de la République et de la chancelière allemande de relancer le projet européen grâce à la force motrice indiscutable du couple franco-allemand, pour autant, l'Union européenne compte 28 bientôt 27 États-membres membres et chacun aura alors un rôle essentiel à jouer afin que nous puissions incarner une véritable Europe puissance cette Europe-puissance défenseur de ses intérêts et protectrice de ces valeurs ne peut néanmoins fonctionner que si tous ses États-membres et institutions jouent le jeu, j'en veux pour preuve la récente nomination de Martin Selmayr au poste de secrétaire général de la Commission européenne dans des conditions inacceptables qui jette une ombre sur le projet européen, le président du groupe, les indépendants, Claude Malhuret, là d'ailleurs parfaitement expliqué lors de sa question au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la semaine dernière à l'aube des élections européennes, cette nomination dans des conditions obscures, est un cadeau aux europhobes qui vont dénoncer l'opacité les manoeuvres internes et le manque de démocratie qu'il reproche à l'Europe, il est absolument nécessaire que la France conteste cette nomination lors du prochain conseil européen en dénonçant le manque de transparence de la procédure, ainsi que la sur-représentation de l'Allemagne au sein des postes clés des institutions de l'Union. Sans hurler avec les loups, populiste et eurosceptique, les partisans de la construction européenne doivent avoir le courage de critiquer ce qu'ils aiment et qu'ils défendent, non pas dans une critique abrasive destructrice et ne celle des europhobes, mais dans une critique constructive et bienveillante avec l'idée de rebâtir la maison Europe sur des fondations plus ferme et plus durable, remercie. La parole est à monsieur Stéphane Ravier pour les non inscrits pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, les sujets abordés lors de ce Conseil européen sont multiples : je me concentre donc sur un seul point et non des moindres, celui de l'adhésion possible de la Turquie à l'Union européenne, car au-delà de l'enfumage médiatique et les déclarations d'un certain nombre de nos collègues parlementaires nationaux la vérité que nous devons aux français veut que les négociations entre la Turquie, les mondialistes de l'Union européiste vont bon train, j'en veux pour preuve une réunion prévue le 26 mars à Varna, en Bulgarie, où les dirigeants de l'Union, rencontreront le président turc Erdogan pour faire le point sur les relations entre l'Union européenne à la Turquie, nous devons normaliser les relations avec la Turquie, a soutenu le 1er ministre bulgare lors d'une réunion avec Monsieur Junker le 12 janvier à Sofia, le président de la Commission européenne avait pour sa part déploré la détérioration des relations avec Ankara, je le cite, la Turquie s'éloigner d'elle même à grands pas de l'Europe, cette rencontre nord ne veut permettre de renouer le dialogue, personne ne s'en cache, elle doit nous permettre de partager nos points de vue sur la façon de faire avancer notre relation sur la base du respect mutuel et de l'intérêt commun, ont insisté messieurs Junker dans leur lettre au président Erdogan alors nous le disons, nous, au Front national et nous sommes les seuls, nous ne voulons pas renouer le dialogue avec la Turquie : nous demandons et ce depuis le début des négociations, l'arrêt définitif du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne pourquoi car Mircher collègues l'histoire, c'est avant tout la géographie, prenez une carte du monde, vous aurez beau la présenter dans tous les sens, a secoué la roulé en boule déployées là, la Turquie ne fera toujours pas et ne fera jamais partie du continent européen, pourquoi car la Turquie islamique ne fait pas partie culturellement de l'Europe chrétienne, n'en déplaise aux talibans de la laïcité aux marchands du temple, l'Europe, c'est avant tout un héritage et les non-judéo-chrétien, pourquoi, parce que la Turquie dictatorial d'Erdogan ne fait pas partie de l'Europe démocratique depuis la tentative de pu-putsch de l'été 2016, l'état d'urgence perdure en Turquie et il est bien évidemment un prétexte pour étendre la répression bien au-delà de la mouvance, accusé d'avoir fomenté le coup d'État, un rapport du Haut Commissariat de l'ONU en date du 20 mars dernier dénonce des arrestations arbitraires et le renvoi des fonctionnaires, les chiffres donnent en effet le vertige à 50000 arrestations, dont 160 journalistes 150 ans, universitaires, 150000 fonctionnaires ont été suspendus ou radiés, on ne compte plus les remises en cause de l'état de droit et de l'indépendance de la justice, un siècle après le terrible génocide arménien, les Turcs continue de persécuter les quelques communautés chrétiennes qui subsistent dans ce pays en pleine réislamisation délaissant le Patrimoine chrétien pourtant multiséculaire avec ses 80 millions d'habitants, l'adhésion de la Turquie fera de l'Europe, une autre petite nièce de l'Islam est une cible de l'islamisme comme pourrait le craindre certains intellectuels français cela aussi, je tiens à le dénoncer, réduction du rôle du Parlement et concentration de ses pouvoirs entre les mains du président presse aux ordres justice sous pression, opposition muselée islamisme conquérant décidément la Turquie ressemblent de plus en plus à la macronie c'est la raison peut-être pour laquelle Emmanuel Macron recevait en grande pompe en janvier dernier à l'Élysée, le président turc, alors de grâce, mes chers collègues, finissons-en avec cette hypocrisie, car l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne est un processus qui avance masqué mais qui a avancé à marche forcée, contre l'avis des peuples contre l'avis des Français avec le soutien zélé de nos collègues socialistes et les républicains au Parlement européen, la Turquie, qui après avoir reçu 7 milliards d'euros de l'Europe doit en recevoir 6 de plus dans les 3 ans à venir, et ce en échange de la maîtrise des flux migratoires, comme le veut un accord funeste signé en mars 2016 insupportable chantage du président Erdogan

de clandestins et qui ont déferlé sur l'Europe entre 2011 et 2017 et la Turquie continue d'être une terre de passage, alors que le nombre de traversées de la mer Égée continue d'avoisiner les 5000 mensuel ministe, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vous le dis, pour des raisons géographiques, historiques, culturelle, politique et démocratique non, définitivement non à la Turquie en Europe. la parole et Tamas Adam la ministre pour une première salle de réponse. Non, non, non, non, excusez-moi, où va, j'ai oublié les rapporteurs. Je m'étais après oui oui. Donc dans la suite du débat, la parole est à monsieur Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces warm. Retrouvant Retrouvant l'esprit de Rome plaider en février 2007, le rapport du Sénat sur l'état de l'Europe, le Brexit, tout autant que les doutes de nos concitoyens exigent que l'on refondu une Europe déjà en crise, c'est cette priorité qu'ont réaffirmé le président de la République et la chancelière à Paris vendredi dernier, notre rapport du Sénat, disait qu'il fallait retrouver un Leadership, le couple franco-allemand est désormais à nouveau sur pied, alors halte aux dérives bureaucratiques repoussoir du projet européen recentrons-nous sur l'essentiel, une Europe offensive centrée sur ses vraies priorités mon collègue bonne car les a rappelé la sécurité, l'emploi, l'immigration, les investissements d'avenir, l'alternative, mes chers collègues, elle éclaire le sursaut ou la sortie de l'histoire en 2050 aucun État européen ne pèsera plus pèsera pèsera moins de 1 pourcent de la population mondiale, seule l'Allemagne fera encore partie des 10 premières puissances économiques mondiales, c'est donc à travers l'Union européenne et elle seule, que les États européens pourront continuer à vivre, c'est aussi en regroupant ses forces que l'Europe pourra préserver son modèle de société et défendre ses valeurs portées par les États-Nations le projet européen doit être renouvelée, le Sénat avait tracé la feuille de route de ce nouveau départ largement repris dans le discours de la Sorbonne, par le président de la République, nous ferons mi-avril avec mon collègue et ami le président Bizet au sein de notre groupe de suivi du Brexit, un point sur la mise en oeuvre de cette feuille de route que nous proposerons à l'exécutif, en quoi l'ordre du jour du prochain conseil européen nous rapproche-t-il de cette exigence de refondation, je laisse à Jean Bizet, le soin de s'exprimer en notre nom à tous les 2 sur la renégociation du Brexit à proprement parler et ne voudrait faire que 2 remarques qui recouvre mais différemment les propos de l'orateur précédent, tout d'abord les Balkans occidentaux dans l'ordre du jour, on trouve en effet un point concernant les négociations d'adhésion qui sont en cours avec la Serbie et le Monténégro, l'ouverture prochaine de négociations avec l'Albanie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine est envisagée, tandis que la perspective européenne semble plus éloignée pour la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, bien sûr, personne ne peut nier la dimension historique et géopolitique de ce processus dans une région longtemps qualifiée de poudrière où les rivalités stratégiques ont toujours été forte avec les jeux d'influence russe turc élargie maintenant jusqu'à la Chine, c'est dans cette région que la première guerre mondiale dont nous commémorons cette année le centenaire a démarré, c'est également là que s'est déroulé le 1er et dernier conflit majeur qui est connu : l'Europe à ce jour, depuis la Seconde Guerre mondiale, si l'Union européenne devait s'élargir aux Balkans occidentaux se veut ce devrait être plutôt pour consolider l'ensemble européen et non pas pour le déstabiliser, or, franchement Madame la Mini, je vous le demande, la relance de l'élargissement est-elle vraiment souhaitable au moment même où l'Europe doit se concentrer sur ça refondation et alors que nos capacités financières vont être réduites par le Brexit évidemment le processus d'adhésion est un puissant levier de réformes dans les pays candidats dans des domaines essentiels tels que l'état de droit, la sécurité, l'émigration, ainsi que pour la pacification des relations à l'intérieur des Balkans, mais je le dis fortement à la lumière des précédents élargissements, il ne faudra frère preuve d'aucun laxisme et les pays candidats devront, le moment venu, être parfaitement prêts, notre conviction est que l'Union, l'Union européenne devra l'être également, ce qui sous-entend qu'elle ait pu elle-même mener les réformes institutionnelles et financières nécessaires à sa relance est-il raisonnable d'envisager les premières adhésions, celle de la Serbie et du Monténégro à l'horizon 2025, pourquoi se fixer ainsi une échéance au risque de décevoir des opinions des pays concernés, alors nous appelons le gouvernement à la plus grande prudence tirons donc les enseignements du référendum britannique sur le Brexit en reconnaissant que l'Europe doit d'abord se consolider elles-mêmes avant de poursuivre un processus d'élargissement qui contribue à la défiance des opinions publiques européennes à son égard. 2ème remarque parlons-en la Turquie candidate à l'adhésion depuis 1999, elle risque de percevoir l'accélération du processus d'élargissement des Balkans comme un affront pour elles-mêmes, c'est vrai, un sommet Union européenne-Turquie doit avoir lieu le 26 mars prochain à valeur à Varna, en Bulgarie, la Turquie souhaite en effet une accélération de son processus d'adhésion, comme nous l'a indiqué récemment encore son ambassadeur à Paris, nous savons tous, et je le dit à l'orateur précédent nous savons tous que cette perspective n'est pas crédible, ne serait-ce qu'en raison de la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, actuellement en Turquie si une réaction des autorités était légitime après la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, le régime d'état d'urgence entraîne des atteintes manifestement disproportionnée à la liberté d'expression et une remise en cause de l'indépendance de la justice, d'autre part, nous le regrettons, la Turquie est à nouveau à l'origine d'une montée des tensions en Méditerranée orientale, où elle a encore récemment bloqué une plateforme de forage italienne, tout près de chips et a été à l'origine de plusieurs incidents avec la Grèce à ceci s'ajoute bien évidemment, mes chers collègues, les préoccupations liées à l'intervention turque en Syrie dans la zone d'Afrine, où la situation humanitaire est absolument catastrophique. Mais à la différence de l'orateur précédent, il est clair que la Turquie demeure un partenaire stratégique majeur, membre de l'Otan, avec qui nous devons dialoguer malgré son éloignement constant et croissant du camp occidental

et la Turquie, dans lequel la Turquie s'engageait à bloquer le flux d'immigration clandestine, cet accord est scrupuleusement respecté de la même manière, nos relations économiques sont eux absolument essentiel et la société civile turque qui souffrent actuellement nous demande constamment de ne pas rompre un dialogue qui demeure un instrument en faveur de transformation interne, le président de la République s'est prononcé lors de son entretien de janvier avec le président Erdogan pour une reformulation du dialogue Union européenne-Turquie : nous pensons que c'est la bonne voie et je pense, Madame la Ministre, que vous aurez l'opportunité de nous préciser quelles sont les modalités de ce dialogue nouveau nous avons d'autres exemples le statut avancé du Maroc avec l'Union européenne en étant c'était une des possibilités alors, mes chers collègues, nous le voyons bien la France est de retour en Europe à vous au gouvernement d'utiliser cette force pour créer une dynamique pour relancer le projet européen car, croyez bien, c'est bien la tante de tous les peuples d'Europe, je vous remercie. La parole est à monsieur Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes. La 8 minutes aussi. Monsieur le Président, Madame le Ministre, monsieur le président de la commission de la défense, messieurs, mes chers collègues, 22 et 23 mars prochain un Conseil européen de printemps particulièrement riche avec en 1er lieu une nouvelle étape importante pour ce qui concerne l'Europe. Près du Royaume-Uni, un projet d'accord de retrait, paru le 28 février à transcrit en terme juridique, le rapport conjoint des négociateurs du 8 décembre 2017, il doit permettre d'aboutir à un accord final d'ici octobre 2018, cet accord devra résoudre les 3 questions clés qui portent à la fois sur le droit des citoyens le règlement financier et la délicate question de l'Irlande, cette dernière question demeure la plus complexe et la plus lourde de conséquences potentielles, comment ne pas reconstituer une nouvelle frontière entre l'Irlande si le Royaume-Uni renonce au marché unique et l'union douanière, comment éviter de faire renaître des tensions qui avaient été apaisé avec l'accord du vendredi Saint, nous prenons acte de l'annonce faite par les négociateurs d'un accord autour de la mise en place d'un espace réglementaire commun incluant l'Union élu Irlande du Nord sans frontières intérieures, j'oserais dire, sans provocation, que c'est en pointillé, une réunification de l'Irlande, qui se profile toujours en pointillés. En l'absence d'une autre alternative, c'est probablement la solution la plus sage, pouvez-vous nous en dire plus Madame la Ministre, c'est aussi l'occasion pour moi de saluer une nouvelle fois l'excellent travail effectué par le négociateur de l'Union. Notre compatriote et ancien collègue Michel Barnier pour la relation future Madame mais a désormais clarifier la position britannique, c'est la solution d'un accord de libre-échange qui est la seule voie possible, soyons clairs, il en résultera des complications et un coût élevé pour les entreprises, mais c'est la conséquence du choix britannique, il ne saurait non plus y avoir un marché unique à la carte, l'intégrité de celui-ci doit être préservé les services financiers seraient soumis à un dispositif d'équivalence, enfin la coopération avec le Royaume-Uni devra demeurer étroite dans des domaines comme la défense ou la sécurité intérieure, je salue d'ailleurs la dernière proposition du président task. Annonçant qu'il n'y aurait pas de barrières tarifaires quelle serait symbolique, par contre, il n'a rien dit sur les barrières non tarifaires et on sait que le coût des barrières tarifaires sont quelquefois beaucoup plus élevé, voire représente 15 pourcent du coût d'une transaction en moyenne une période de transition paraît inévitable, mais elle sera conditionné à un accord sur les modalités de retrait. Nous approuvons les principes posés par l'Union cette période ne doit pas aller au-delà du cas de financier pluriannuel en cours, soit le 31 décembre 2020, ne doit pas être reconductible également le Royaume-Uni devra respecter l'ensemble de l'acquis communautaire, mais il ne sera plus partie au processus de décision puisqu'il sera désormais années les 4 libertés, en particulier la liberté de circulation devront être main. Nous, nous prenons bonne note d'un accord trouvé par les négociateurs sur cette transition, pouvez-vous, Madame la Ministre, apporter plus de précisions, au Sénat, sur ce point, pendant que le Royaume Uni organise son isolement, parce que je crois qu'il faut le dire ainsi, l'Europe doit continuer à avancer, en affirmant son unité, le Conseil européen de juin devra marquer une étape importante pour la relance européenne. Mais dès sa réunion de mars. Le Conseil européen abordera des questions cruciales, je pense à la stratégie du marché unique au marché unique du numérique à l'Union des marchés de copies. Taux et à l'union de l'énergie d'ici décembre, la commission devrait faire un point sur la mise en oeuvre de la législation existante, l'Union doit aussi se doter d'une stratégie industrielle forte, c'est un enjeu majeur en s'appuyant sur l'atout que constitue son. Marché unique véritable joyau, fruit de. Plus de 50 ans de travail en commun : l'Europe doit organiser une véritable reconquête industrielle, le défi du numérique est maintenant de latin, jeunes gens s'artificiel doit être relevé, l'Europe ne peut être simplement consommatrice, elle doit être aussi productrice pour cela, nous devons faire émerger champions européens, on le dit souvent et depuis plusieurs années, ici au Sénat, la politique de la concurrence a été conçu dans un contexte je dirais d'autrefois, il y a plus d'un demi-siècle, qui n'a plus rien à voir avec les enjeux d'aujourd'hui, le monde a changé la politique de l'autorité de la concurrence doit elle aussi changer, elle doit être réformé pour mettra l'union de rôle revêt relevé, pardon, le défi de la reconquête industrielle, la fiscalité du numérique est aussi un enjeu important, que peut-on attendent du Conseil européen sur cette épineuse question entre les propositions de la commission, les propositions également et les réflexions de l'OCDE en la matière, le Conseil européen devra affirmer également son engagement pour un multi-latéralisme commercial réguler avec l'Organisation mondiale du commerce en son centre, il devrait aussi soutenir les négociations en cours d'accord de libre-échange le système multilatéral est malheureusement en crise les États-Unis ne sont pas je dirais étranger à tout cela, refusant depuis plusieurs mois, voire quelques années, je dirais le bon fond. Seulement de l'organe de règlement du différend, le tribunal commercial international en refusant la nomination de 3 juges par. C'est précisément à la retraite, mais l'Union européenne doit jouer un rôle actif pour tenter de redresser ce multilatéralisme et dans ce contexte des accords commerciaux bilatéraux peuvent être bénéfiques pour l'Union, mais ceci doit défendre fermement ses intérêts exiger la réciprocité, le Sénat a fait valoir cette position lorsqu'il a débattu de la résolution européenne sur les directives de négociations en vue d'accord avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, notre commission examinera dans quelques instants à l'issue de ce débat, le rapport de Pascal Alizart et Didier Marie, sur la proposition de notre collègue Jean-Claude Requier sur les négociations avec le Mercosur, nous pourrons ainsi réaffirmer avec beaucoup de clarté ses positions, enfin, le Conseil européen devrait évoquer les relations avec les Balkans occidentaux, le président, bon, on a évoqué tout à l'heure. Tout ceci, quelques semaines avant le sommet qui se tiendra à Sofia, le 17 mai non rapporteur Claude Kearney Simon ensuite. Pour se rendront en Sibérie, pardon en Serbie. Et ils en reviendront, j'en suis persuadé en Serbie et en Monténégro qui négocient précisément leur adhésion, nous sommes favorables. Aux initiatives qui permettront de renforcer la connaissions la connexion de cette région avec l'Union ou de prévoir un engagement commun sur des défis tels que la sécurité ou l'émigration mais nous devons aussi veiller à prendre en compte l'état de nos opinions publiques à l'égard d'une procédure d'élargissement qui a paru aller un peu trop vite, et donc le courage de dire qu'il faut assumer et confirmer le moratoire sur l'élargissement pour conforter l'acquis communautaire, je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre, monsieur le président, Mesdames, messieurs les présidents Jacques collègues au cours de ces derniers mois, le contexte économique au Royaume-Uni, le contexte économique en Allemagne ou encore en Italie, ainsi que les divergences toujours aussi profonde entre les États membres sur l'avenir de la zone Euro ont pu éloigner la perspective d'un Conseil européen ambitieux néanmoins concernant le Brexit l'accord trouvé lundi dernier sur la période de transition va pas maître d'enrichir considérablement les échanges entre les États membres et d'ouvrir le débat, le début des discussions relatives aux relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, quelques mots d'abord concernant précisément le Brexit après ouvert avoir ouvert la seconde phase de négociations en décembre dernier les 27 États-membres devront adopter les orientations présentées par le plan Tusk, début du mois concernant le cadre de relations futures avec le Royaume-Uni, la question de l'inclusion des services financiers dans le futur accord de libre-échange cristallise les tensions, le projet d'orientation qui devait être initialement présenté au Conseil européen, les écarter de la discussion d'un futur accord de libre-échange, toutefois, les ministres des Affaires étrangères des affaires européennes des 27 États-membres ont approuvé hier vous le savez, je l'avais dit un projet incluant les services financiers dans une annexe, comme je l'avais déjà rappelé en décembre, notre commission des finances, a estimé que dans le cadre de nos travaux sur la compétitivité des places financières, a estimé qu'un accord couvrant l'ensemble des services financiers ne s'imposait pas le ministre de l'économie, Bruno Lemaire, a évoqué la mobilisation des régimes d'équivalence et qui d'équivalence existants, notre commission des finances, a souhaité attirer votre attention, la dernière sur la nécessité de rendre plus exigeants, ces régimes d'équivalence, afin d'éviter les risques de divergence réglementaire, ceci pourrait se traduire par l'introduction d'un mécanisme de réexamen régulier des décisions d'équivalence a qu'ici qu'une obligation de réciprocité, alors j'ai une question madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer que les services financiers seront bien inclus dans les négociations à venir sur l'accord de libre-échange avec le Royaume-Uni et, bien sûr, si telle est le cas Compte-tenu des risques que je viens de rappeler je souhaiterai souligner qu'il est préférable que les services financiers soient soumis à des régimes d'équivalence renforcer plutôt qu'un régime Haddock propre au Royaume-Uni. Enfin, concernant l'accord de transition, l'impasse politique semble résolu en achevant la période de transition, le 31 décembre 2020 la question de la participation du Royaume-Uni au prochain cadre financier pluriannuel et donc tranché Madame ministre, bien que ce point ne soit pas spécifiquement à ce qu'Elor du jour du Conseil européen, je me permets de souligner que les discussions concernant le prochain cadre financier pluriannuel soulève des inquiétudes quant à l'avenir des politiques communes, nous souhaiterions donc une clarification de la position française, notamment au sujet du financement de la politique agricole commune, dans un contexte où le retrait du Royaume-Uni devrait se traduire par une perte d'au moins 10 milliards d'euros pour le budget de l'Union européenne, je reviens alors du jour du Conseil européen, car d'autres points, et ils sont nombreux, mais d'autres points intéresse notre commission des finances s'agissant tout particulièrement du sommet de la zone Euro, les propositions avancées par la Commission européenne en décembre dernier s'avérait plus pragmatique que celle défendue par le président de la République, toutefois, aucune mise en oeuvre concrète est envisagée et les blocages politiques demeurent, comme l'a souligné le refus de 8 pays d'Europe du Nord, y compris les Pays-Bas, pays refus de mener des réformes ambitieuses,

je me réjouis de cette avancée, mais je tiens également nécessité réaffirmer la nécessité pour le futur Fonds monétaire européen de voir sa responsabilité engagée devant les Parlements nationaux, dans ce contexte, il semble que la consolidation de la zone Euro, devra encore attendre le sommet de juin, la publication d'une feuille de route franco-allemande sera nécessaire sans doute nécessaire pour avancer, certes nous sommes a priori moins pressé contenu de l'embellie économique avancé dans la zone Euro mais contesté dans la zone Euro, néanmoins, il semble plus opportun plus que jamais de renforcer la résilience de notre système bancaire et la convergence des économies nationales, enfin j'aborderai la question de la fiscalité du numérique qui vous savez, intéresse particulièrement à la commission des finances concernant la fiscalité du numérique, la Commission européenne a présenté, ce matin, 3 textes différents, pour mettre en oeuvre une taxation des entreprises du secteur numérique dans les pays où il réalise des activités à court terme, il s'agirait d'instaurer, vous le savez, une taxe de 3 pourcent sur les recettes brutes de certaines activités numériques dans une perspective de plus long terme, la Commission présentera une proposition de directive visant Wax non plus, le chiffre d'affaires mais à taxer les bénéfices, le bénéfice d'entreprise grâce à la notion de présence numérique significative, une notion qui serait appréhendé par des critères tels que l'utilisation des données personnelles, je tiens à saluer ses propositions, ce qui s'inscrivent dans le sillage de recommandations de la France et qui vont évidemment dans le bon sens, comme vous le savez, la commission des finances du Sénat, travaille depuis plusieurs années sur la fiscalité numérique et ce dans le cadre d'un groupe de travail,

à cet égard, je rappelle que notre commission des finances avait déjà regretté cette approche graduée de la Commission européenne, notamment en matière d'accès, de consolider l'impôt sur les sociétés, plus communément appelé Axis et on a vu aujourd'hui les limites de cette approche madame le ministre j'espère que la France encouragera ses partenaires européens à une prise de décision en matière de taxation des entreprises du secteur numérique pour prolonger l'initiative à laquelle j'avais pas, il avait participé à la dernière, c'est un enjeu absolument majeur quand on voit aujourd'hui le faible taux d'imposition payées par l'entreprise, plus communément appelé GAFA et les enjeux que cela représente, vous avez encore une table ronde ce matin par la commission des finances, merci de votre attention sur ce sujet, nombreux et variés qui retiennent partiront à l'attention de votre commission des finances. finances. Maintenant, donc c'est bien madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes. Répond pour un temps.

permettez-moi d'essayer de me concentrer sur les remarques qui relève de l'ordre du jour du conseil, je reviendrai. Tout de même rapidement après avoir entendu Monsieur le Sénateur, mais non vide, Monsieur le Sénateur Ouzoulias sur la lecture que l'on peut faire du résultat des élections italiennes, je partage le point de vue exprimés selon Le Caire électeurs italiens n'ont pas regretté trop d'Europe mais plutôt pas assez d'Europe au moment où l'Italie avait le plus besoin que l'on exprime notre solidarité à son endroit, qu'il s'agisse des conséquences de la crise financière ou de l'afflux massif de migrants auxquels elle a eu à faire face devant l'avoir à l'esprit, au moment où nous travaillons sur la réforme, la réforme de l'Union européenne, nous l'avons pleinement à l'esprit, au moment où nous travaillons sur la réforme du régime de l'asile et d'émigration, y compris au plan national, puisque le projet de loi asile immigration vise précisément à pouvoir davantage harmoniser l'examen des demandes d'asile à travers l'Union européenne et c'est pleinement inspiré des pratiques, notamment de nos voisins allemands, je reviens sur l'ordre du jour du conseil et vous avez été nombreux à évoquer le Brexit monsieur le Président, Bizet, monsieur le Montgolfier Madame Keller messieurs Catelin monsieur Menonville je vous en remercie car vous me donnez l'occasion de revenir sur ce sujet important, oui monsieur Gattolin oui Monsieur le Président, Bizet, le mode de règlement de la question irlandaise est encore floue, je vous le concède bien volontiers et cela constitue un objet de préoccupation pour nous éclaircir cette question avant octobre une priorité, il reste malgré tout que l'accord exprimé par les Britanniques sur ce qu'on appelle le Back, Stop, ce qui revient à ce que, faute de mieux, l'Irlande du Nord reste de fait dans l'union douanière constitue un petit progrès, s'agissant des services financiers. Nous avons rappelé que le Royaume-Uni ne pouvait plus bénéficier passeports financer la première ministre britannique l'a elle-même reconnu et nous avons insisté pour que les services financiers soient traités en dehors de l'accord de libre-échange, par des mécanismes d'équivalence définie unilatéralement par l'Union européenne, j'espère avoir répondu à votre préoccupation, monsieur le rapporteur général. Sur sa Bery. Monsieur le sénateur Gattolin a rappelé la gravité de ce qui vient de se passer au au Royaume-Uni, nous avons exprimé notre totale solidarité vis-à-vis de notre voisin, partenaire et allié britannique. Qu'il reste. Donc, il quitte l'Union européenne ne change rien à ce voisinage à ce partenariat, et à cette alliance, le Conseil européen reviendra sur cette question jeudi soir et s'exprimera sans doute fortement. La double tentative d'assassinat intervenu à Strasbourg, il est en effet le premier example depuis 1945 d'utilisation sur le sol européen d'un agent neurotoxique prohibée, c'est donc une affaire particulièrement sérieuse. Plusieurs d'entre vous ont également souhaité revenir sur le sujet relatif à la zone Euro, monsieur de Montgolfier Madame Keller Madame Mellow. Croyez bien que nous sommes pleinement mobilisés à travailler au renforcement de la zone Euro à la finalisation de l'union bancaire au renforcement du mécanisme européen de stabilité ou bien encore à la création d'une capacité budgétaire de la zone Euro, afin de faire face, au prochain choc vous économique et de pouvoir maintenir le niveau d'investissement c'est précisément au moment où la croissance est revenue dans la zone Euro, que nous sommes en situation de travailler à ses sujets. Il y a évidemment des nuances, tant les positions des différents États-membres, il y a évidemment des sujets techniques qu'il faut surmonter les Pras les les nous progressons, je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes engagés à présenter conjointement une feuille de route avec l'Allemagne pour le prochain conseil européen de juin, j'ai bien noté, madame la sénatrice quelle heure votre intérêt pour un contrôle parlementaire accru l'intérêt que je ne saurais contester ici en ces lieux et que nous partageons. voudrais tout de même dire qu'aujourd'hui une priorité, elle est à la finalisation de l'union bancaire. à l'Union des marchés de capitaux et à la mise en place d'une capacité budgétaire c'est petit à petit que nous progresserons dans le renfoncement de de la zone Euro, vous l'avez signalé s'agissant du semestre européen Madame la sénatrice mélo. La sortie de la France de la catégorie des déséquilibres excessifs est une bonne nouvelle, mais nous ne nous tous vont pas pour autant relâcher nos efforts, la reprise est là, elle doit encore être soutenue notamment par des refus réformes structurelles c'est également indispensable pour garantir la soutenabilité de nos finances publiques, nous serons à ce titre pour la première fois en 2017 depuis 10 ans sous la barre des 3 pourcent du PIB le déficit public.

Nous devons aborder la négociation du prochain cadre financier pluriannuel en étant cohérent avec nos ambitions pour l'Union européenne. Il y a un consensus pour considérer que de nouvelles priorités doivent être traités au niveau de l'Union européenne, il y a également un consensus pour ne pas sacrifier les politiques traditionnelles, de ce point de vue-là. Notre détermination à poursuivre. Les politiques historiques en priorité la PAC est totale, nous sommes d'ailleurs clairement opposées à toute renationalisation de la PAC, et donc à tout cofinancement national du 1er pilier je vous rassure Monsieur ça signifie, il faut d'abord fixer nos priorités avant de définir l'enveloppe. Du budget européen, je partage Madame Robert votre encouragement à explorer de nouvelles ressources propres pour que de travail a été accompli. Pour réfléchir à de nouvelles ressources propres, je pense en particulier au groupe de haut niveau, présidée par Mario Monti n'est plus temps d'en faire l'objet de colloques et de discussions intellectuelles mais de traduire dans les faits ce que ce sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord en matière de nouvelles ressources propres pour le budget de l'Union européenne, j'ajouterai qu'au moment où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il est temps de mettre fin à toutes les formes de rabais qui avaient été négociés et adoptés au fur et à mesure et qui n'ont plus leur place aujourd'hui dans le budget européen s'agissant de la politique de cohésion, je voudrais aussi vous dire dans quel état d'esprit, nous abordons cette négociation, nous pensons qu'elle doit être conditionnée, mais qu'elle doit être conditionnée au respect des valeurs de l'Union européenne et donc en particulier de l'État de droit et aux efforts de convergence fiscale et sociale, qui sont le gage de la cohésion. Vous avez été aussi nombreux à parler de fiscalité du numérique, monsieur le rapporteur général, monsieur Menonville Madame Keller Madame Mellow, il s'agit d'un des défis majeurs de notre temps, nous sommes à ce titre, déterminé à aboutir à une juste taxation des géants du numérique au niveau européen sans attendre. Qu'un accord soit trouvé au niveau international, nous voulons une Europe de l'équité de la justice fiscale, bien entendu, le sujet est complexe, mais le statu quo ne peut perdurer nos concitoyens attendent des résultats, nous sommes de ce point de vue pleinement en phase avec la proposition présentée aujourd'hui par la Commission et qu'il fera demain l'objet d'un débat lors du dîner du Conseil, vous avez également mentionné madame la sénatrice Keller et monsieur le rapporteur général, les discussions sur l'ça vous le savez. Au conseil cette discussion ne progresse pas, nous le regrettons et nous sommes déterminés à avancer sur une harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en franco-allemand et de ce point de vue, le travail a repris avec la nomination d'un nouveau gouvernement allemand et nous allons essayer d'aller de l'avant en bilatéral entre la France et l'Allemagne, et je dirais, de ce point de vue de donner l'exemple pour faire en sorte que ce qui est faisable entre Paris et Berlin se s'largesses à l'ensemble de de l'Union européenne en matière d'Europe sociale, la commission Madame Mellow Madame Robert vient de présenter son projet d'autorité européenne du travail, nous sommes en train de l'examiner en détail, mais l'enjeu est important puisqu'il s'agit de lutter contre les fraudes et ce de de se donner les moyens collectivement de faire respecter nos règles du jeu communes l'absence d'autorité du travail, explique une partie des fraudes au détachement des travailleurs sur ce dernier sujet, vous l'avez évoqué l'accord intervenu permet d'encourager la mobilité des travailleurs tout en convergeant vers le haut, en avançant vers une Europe qui protège mieux ses citoyens. Sur les Balkans occidentaux mais. C'est président encombrant Monsieur le Président, Bizet je partage votre point de vue fixer une échéance théorique pour l'adhésion de nouveaux membres de l'Union européenne est artificiel et n'a pas de sens en soi. à sa décharge, ce n'est pas vraiment pas exactement ce que fait la Commission, le président Junker a été très clair publiquement sur le caractère impératif des critères à remplir pour les pays candidats. Nous serons fermes sur le respect de ces critères, y compris pour l'Albanie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui de notre point de vue ne paraissent pas aujourd'hui en situation de les remplir, dans un délai rapproché, ce qui ne permet pas d'ouvrir les négociations, il était également indispensable et vous le soulignez, à raison, Monsieur le Président, Bizet, de continuer à travailler étroitement avec ces pays, en particulier dans le domaine de l'état de droit, où il reste encore beaucoup à faire, mais aussi pour la jeunesse, pour la sécurité ou pour une intégration plus forte dans le secteur des transports ou des télécommunications par exemple c'est ce c'est là l'objet du sommet de Sofia, du 17 mai mais aussi des échanges bilatéraux que nous avons avec ces pays, l'Union européenne doit impérativement en enforcer son partenariat vis-à-vis des Balkans pour ne pas laisser le Champ libre à la Turquie à la Chine à la Russie ou à d'autres dans les logiques et les intérêts diffère des nôtres. Enfin, bon nombre d'entre vous êtes revenu sur l'actualité avec les États-Unis à travers les annonces du président Trump en matière commerciale, nous le savons tous une guerre commerciale avec les États-Unis sur l'acier sur l'aluminium ne ferait que des victimes et des victimes très concrètes, puisqu'il s'agirait des producteurs européens. Face à ces mesures américaines Monsieur von l'Union européenne doit donc réagir dans l'unité, nous recherchons en priorité une exemption de ces mesures américaines, le temps presse, en cas d'échec, notre réaction devrait être forte et respectueuse du multilatéralisme, nous nous y préparons, c'est ce que la commission fait avec notre appui, je voudrais pour terminer dire un mot de la Turquie Monsieur Cambon Monsieur Je vous confirme que nous trouvons parfaitement naturel de dialoguer avec la Turquie voisine géographiques de l'Union européenne partenaire difficile mais essentiel dans la lutte contre le terrorisme ou dans la réponse au défi migratoire qui vous préoccupe tant sur aviez. Mais nul ne songe à poursuivre les négociations d'adhésion avec la Turquie. Nous constatons. Le blocage du à des choix politiques opérés par Ankara qui l'éloigne chaque jour davantage, des valeurs de l'Union européenne, je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au débat interactif et spontané, dont la durée a été fixée à une heure par les la conférence des présidents une heure maximum. Et pas obligé Chaque sénateur peut intervenir pour 2 minutes maximum s'il se manifeste, s'ils sont sollicités, la commission des affaires européennes ou le gouvernement pour rire pourront répondre, s'ils sont sollicités, donc qui veut prendre la parole pour prendre les dernières inscriptions. En espérant que cela va tenir dans une heure maximum. bien. Et donc on va commencer par monsieur Alizart. Pour 2 minutes Monsieur le président merci madame la ministre, mais chers collègues sur l'agenda même Nice vous l'avez précisé tout à l'heure de ce prochain conseil, les sujets ne manquent pas et il s'ouvrira une nouvelle fois sur une Europe en crise aux prises avec des menaces intérieures comme extérieures qui mettent en péril son avenir parmi les plus grands dangers, je pense au populisme à la division et au final, au risque de la désintégration de l'Union européenne Royaume-Uni a déjà un pied dehors, les pays du groupe de grade marque souvent leur différence, voire leur défiance et l'Italie, ça a été rappelé aussi vient d'envoyer un message politique très clairement cette montée des populismes à laquelle la France n'échappe pas, n'est pas apparu ex nihilo, elle a des causes profondes et multiple, il y a évidemment le terrorisme qui continue d'inquiéter sur le vieux continent, l'avenir de la zone Euro, les tensions toujours fortes avec la Russie, la concurrence économique mondiale exacerbée mais je crois que le point de jonction de tous les eurosceptiques, et sans doute la crise migratoire, celle que l'Union européenne a géré maladroitement dans l'urgence et en laissant notamment l'Italie, en première ligne trop longtemps, on en mesure aujourd'hui les conséquences, en déplacement à Bruxelles il y a quelques jours, sur la politique migratoire, j'ai été particulièrement choqué par ce verbiage technocratique et condescendant de fonctionnaires européens vis-à-vis de ceux qui pensent mal ou de ceux qui ne comprennent rien, ces citoyens européens en plein désarroi auquel nous sénateur nous adressons au quotidien dans nos territoires, ils ont besoin d'action d'explication de geste qui rassure et pas de stigmatisation des toujours plus commode de montrer du doigt de soi-disant égaré que de s'attaquer réellement au problème contexte que j'estime dangereux, quelle leçon la France tirera-t-elle du scrutin italien et quelle politique migratoire défendra-t-elle auprès des instances européennes, je vous remercie. Merci madame la ministre vous répond. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Alizart, je l'ai dit tout à l'heure, nous considérons que les électeurs italiens ont adressé un message clair : l'Europe n'a pas été assez présente pour les aider à faire face au défi migratoire qu'il devait relever, c'est la raison pour laquelle, depuis l'été dernier, la France s'est beaucoup engagé à traiter tout d'abord la dimension externe de la crise migratoire en travaillant davantage avec les pays d'origine d'migrations en orientant mieux et de manière plus systématique, l'aide au développement en faveur de la formation et de l'emploi des jeunes, en particulier en Afrique subsaharienne en travaillant à la stabilisation des pays de transit et nous avons tous en mémoire les horreurs que subissent les candidats aux migrations lorsqu'il traverse, la Libye, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous travaillons à la fois la stabilisation de la Libye, mais aussi à faire en sorte que l'examen des demandes de d'asile puisse être fait des, des pays comme le Niger ou le Tchad et nous encourageons les autres pays européens à faire la même chose que ce que nous avons commencé à faire sur la réforme du régime européen du de l'asile, nous n'avons pas beaucoup avancé, nous avons avancé sur certains aspects, mais pas tous, il faudra à l'évidence, disposer d'un gouvernement italien issu des élections pour pouvoir dialoguer avec ce partenaire important puisqu'il a été particulièrement impactés, je dirais que, évitons de blâmer la technocratie de Bruxelles, là où ce dont l'Italie a le plus souffert, c'est du manque de solidarité de certains États-membres qui ont considéré que la solidarité c'était recevoir des crédits européens mais pas recevoir des demandeurs d'asile. La parole est à monsieur le pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaitais commencer ma question par de de conviction, la 1ère c'est qu'on ne peut pas opposer l'élargissement de l'Union européenne et son approfondissement. On a toujours dans l'histoire, eu le courage de faire l'un et l'autre en même temps, ou de ne faire ni l'un et l'autre par manque de courage, la 2ème conviction c'est que si l'Union préfère la stabilité à la défense de ses valeurs, elle perdra sa stabilité et n'aura plus de valeur et c'est la raison pour laquelle lorsque je constate l'évolution du président Junker sur la question des Balkans, je dois saluer en 2014 au moment de sa prise de fonction, il disait souvent mandat pas d'élargissement en 2017, il parlait de l'âge de, de, d'offrir une feuille de route, crédible et en 2018 le 2 février il a offert cette feuille de route, elle était effectivement indispensable Karl les conséquences des fausses négociations actuelles qui ont transformé finalement une perspective européenne en état de négociations sont dramatiques, une un état de droit préoccupant dans la plupart de ces pays, un développement des trafics criminels, une situation économique et sociale qui incite à à l'immigration massive et qui n'est pas du tout similaire à ce qu'on constate en Europe centrale, où il y a plutôt une embellie économique enfin des accords d'investissement avec les Émirats, l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou la Chine, à des conditions extraterritoriales dans la plupart de ces pays qui sont de plus en plus préoccupante cette en laissant finalement prospérer à nos frontières, cette instabilité et ses menaces, c'est l'ensemble de l'Union européenne que nous menaçons l'Allemagne a bien compris ces enjeux et la position de la France par contre malheureusement est beaucoup plus ambigu et vos réponses comme la l'intervention du président de la commission des Affaires étrangères, le thème en témoigne : il est triste, madame la ministre, que dans cette région, 100 ans après le Front d'Orient qui a été essentiel pour notre présence de la France et et l'image de la France dans cette région que le rôle de la France aujourd'hui s'inscrivent et se place plutôt sur l'étagère de la l'Ostalgie quelles initiatives la France entend-elle avoir pour ne pas être à leur remorque de l'Allemagne sur cette question majeure de l'élargissement aux Balkans, je vous remercie. Madame la Ministre.

nous avons une histoire commune, nous avons une géographie commune et nous avons donc un destin commun et si l'Union européenne ne s'intéressent pas aux Balkans, d'autres le feront et le font déjà, c'est la raison pour laquelle, à l'occasion du sommet de Sofia, du 17 mai nous poussons pour un agenda positif, à destination des pays des Balkans, qu'il s'agisse de venir en aide à leur jeunesse, notamment en poussant à des mobilité étudiante vers les universités de l'Union européenne en prenant garde toutefois à ne pas alimenter la fuite des cerveaux dont ces pays sont déjà les victimes et puis aussi en soutenant la mise en place d'infrastructures de transport de télécommunication qui leur permettent à la fois d'être mieux équipés d'être mieux intégrées sur le plan régional, ceci étant tendre la main à aux Balkans, c'est aussi rendre service aux réformistes et aux progressistes de ces pays en les aidant à pousser un agenda de réformes indispensables de réformes à adopter, mais surtout de réformes à mettre en oeuvre, qu'il s'agisse de l'étape droit qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption, qu'il s'agisse de la lutte qu'il s'agisse de la lutte contre le Crime organisé, ces pays ont encore beaucoup à faire, nous sommes prêts à Alesi mais il serait irresponsable de faire miroiter à ces pays une adhésion à l'Union européenne, tant qu'ils ne se sont pas davantage rapproché de ses valeurs. Merci, la parole ta Madame Goulet 2 minutes. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, comme le dit très bien notre ancien collègue Jean Arthuis, l'Europe ne parle pas aux Européens, et j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, les priorités sont aux marchés financiers, moi je voudrais. Parler de l'Europe, qui est un peu inaudibles Kemal inaudible face au au barbarie, on a vu le Yézédis on a vu les Syriens et je voudrais vous parler du Yémen, je vais vous parliez du Yémen, parce que ce pays traverse une crise ancienne depuis 2015, l'Europe a contribué à hauteur de 200 millions d'euros pour l'aide aux populations et et je pense que l'Europe doit pro doit procurer aux populations une aide technique pour recevoir les aides, notamment de la dernière conférence des donateurs à à Genève, l'Arabie Saoudite propose plus d'un milliard d'euros, et a déjà versé un autre milliard les Émirats et d'autres pays sont venus pour aider les populations yéménite, le problème c'est que l'aide n'arrive jamais à l'endroit où elle est supposée arriver et donc on a un problème, puisque de toute façon, cet argent pourrait très bien servir aux adversaires des pays voisins et même tomber en des mains mauvaise ou en tous les cas pas auxquels sont destinées, donc je pense que l'Europe qui a quand même une technocratie, que le monde entier lui envient pourrait aider et assister ces pays à pouvoir diriger à la fois l'aide humanitaire à la fois l'aide alimentaire mais aussi l'aide médicale et l'aide financière donc ma question est assez simple : pensez-vous que l'Europe puisse aussi proposer une aide technique au Yémen, de façon à assurer l'aide financière et sa bonne arrivée à destination de ces populations qui sont dramatiquement touché, je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le président, madame la sénatrice Goulet, le Yémen d'une tragédie, une tragédie, vous n'en avait pas véritablement fait état mais une tragédie qui tient au fait que un conflit dure depuis des années dans ce pays et que, à ce stade, ce que nous réclamons, c'est la possibilité pour l'aide humanitaire d'entrer dans un pays où les aéroports sont détruits ou les installations portuaires sont occupés et où les convois humanitaires ne peuvent pas circuler, vous le savez, des médecins de Médecins sans frontières ont même été pris pour cibles l'urgence c'est de mettre fin aux activités militaires, c'est de trouver une forme de règlement politique évidemment de travailler à destination des populations et de travailler à une reconstruction du Yémen, il n'est pas anormal que les pays du Golfe, compte tenu de la responsabilité qui est la leur dans la situation actuelle du Yémen soit loin devant ceux qui doivent participer à sa reconstruction, ce n'est pas nous qui avons participé à sa destruction. alors la parole est à monsieur Richard. C'est le président, M. la ministre, mes chers collègues, l'approfondissement de l'Union européenne et monétaire sera donc au menu du sommet de la zone Euro de vendredi. En la matière, la proposition phare d'Emmanuel Macron, le président et la création d'un parlement de la zone Euro qui aurait vocation à contrôler l'exécution d'un budget autonome devant atteindre plusieurs points de PIB, soit un montant se chiffre en centaines de milliards d'euros d'ores et déjà l'idée d'un Parlement spécifique semble devoir connaître le même sort que la proposition de listes transnationales pour les élections européennes qui, comme vous le savez, a été enterré le mois dernier par le Parlement européen et par les chefs d'État et de gouvernement quant au budget de la zone Euro, la réalité politique rattrape ce projet du président de la République la Commission européenne n'a pas jugé bon d'aller au-delà de la proposition d'une simple ligne budgétaire intégré au budget général de l'Union, par ailleurs, les pays d'Europe du Nord, ont adressé, le 6 mars une fin de non-recevoir catégorique à cette idée, arguant à mon sens, non sans raison, que l'avenir de la zone Euro passe avant tout par la remise en ordre des politiques économiques et budgétaires nationales quant au partenaire allemand, il risque bien d'être difficile à convaincre l'accord de coalition conclu entre la CDU, CSU et le SPD qui placent l'Europe au coeur de son projet ignore comme vous le savez, totalement cette proposition madame le Ministre dans ces conditions, ma question est simple : la création d'un budget autonome de la zone Euro est-elle vraiment encore une proposition officiellement soutenu par la France et parce l'de la feuille de route que la France discutera prochainement avec Berlin en vue du Conseil européen de juin, si c'est le cas, pouvez-vous nous en dire plus sur le montant et l'affectation défendue par la France sur ce budget je vous remercie. Merci madame la ministre, votre réponse. constitue le gouvernement allemand figure précisément le renforcement de la zone Euro, alors il peut être facile de signer une lettre à quelques-uns dans un journal, quand tout va bien, quand la zone Euro est en croissance pour considérer que on se préoccupera de son renforcement plus tard plus tard quand, quand tout ira mal quand on devra, comme on a dû le faire il y a quelques années, agir dans la précipitation, quand il faudra rendre des comptes aux populations, ce qu'on n'a guère fait pendant la gestion de la crise financière s'il faut un contrôle démocratique aux décisions prises dans la zone Euro, c'est que c'est ce qui a cruellement manqué compte on a par exemple le traité du cas de de la crise grecque c'est ce qui explique aujourd'hui le désamour vis-à-vis de l'Union européenne dans une partie de l'Europe du Sud, qui pourtant était la zone en Europe la plus favorable à la construction européenne, alors on peut décider de ne rien faire et d'attendre que tout aille encore plus mal que les populistes, avance encore davantage à chaque échéance électorale où on peut décider qu'on prend ses responsabilités, que, il ne suffit pas d'appeler à davantage de rigueur et à faire le ménage chez soi, là, la prévention des risques, c'est : c'est bien le partage des risques, c'est important aussi cela et la conséquence normale du fait que nous avons une monnaie commune que nous avons besoin d'avoir une union bancaire, une union des marchés de capitaux, parce que c'est ce qui est favorable à la croissance et à l'emploi dans l'Union européenne, c'est pourquoi nous travaillons notamment avec l'Allemagne, vous l'avez très justement rappelé pour rédiger une feuille de route d'ici le mois de juin, vous me permettrez à quelques jours après la constitution du gouvernement allemand de ne pas vous donner les résultats des tous premiers entretiens que nous avons eu le président de la République avec Madame Merkel, Bruno Lemaire avec son homologue, Jean-Yves Le Drian, avec le sien et moi-même, avec le ministre des affaires européennes allemand. Merci, la parole est à monsieur Didier Marie. Il n'est pas là donc à Madame Robert. Oui, merci Monsieur le Président, en fait, je vais poser la question, que devait poser monsieur Vaugrenard qui malheureusement ne peut pas être là cet après-midi, il a, il y eu a un souci, donc si vous me permettez, je vais poser la question, qu'il souhaitait, vous posez, Madame la Ministre, cet après-midi, je souhaiterais aborder la question des droits sociaux et notamment les dernières propositions de la Commission européenne sur la mise en oeuvre du socle européen des droits sociaux, il s'agit du projet de création d'une autorité européenne du travail ainsi qu'une initiative visant à garantir l'accès à une protection sociale pour tous les travailleurs salariés et non salariés aujourd'hui ceux qui travaillent à temps partiel dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou ceux travaillant sans être salariés représentent près de 40 pourcent de ceux qui occupent un emploi, ces personnes n'ont toujours pas une bonne couverture sociale ne bénéficiera pas systématiquement d'une assurance chômage et non pas obligatoirement accès à des droits à pension, la proposition de la Commission vise donc à fixer un cap aux États-membres afin de favoriser l'accès à la protection sociale pour tous les travailleurs, salariés ou non, il est également prévu de publier une analyse des mesures prises et des progrès réalisés au niveau national en matière d'emploi ainsi que dans le domaine social,

les discussions à 27 sont en effet particulièrement complexe, ne serait-il pas temps de modifier la lourdeur des procédures européennes et de rendent possibles des prises de décisions à la majorité, voire à moi dans le contexte international que nous traversons, l'Europe ne pourra peser que si elle accepte d'agir sans être obligatoirement et systématiquement d'accord à l'unanimité, il s'avère donc nécessaire et urgent de réfléchir à la remise en cause de la règle absolue de l'unanimité, pouvez-vous, Madame la Ministre, mais donner la position du gouvernement sur cette ambition de décisions à géométrie variable selon les sujets à évoquer et notamment sociaux je vous remercie. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Robert en matière d'Europe sociale se Göteborg a été un moment important parce qu'il a permis de proclamer un socle de droits sociaux dans l'Union européenne, maintenant il nous faut passer au concret, la traduction des déclarations d'intention en projet législatif européen, nous y sommes attachés je je parlais tout à l'heure de notre soutien de principe à la création d'une autorité européenne du travail, je ne vous cache pas que le climat n'est pas simple pour une raison qui, elle, est assez facile à comprendre, vous avez d'une part des pays du nord de l'Europe qui ont peur que tout travail d'harmonisation sociale dans l'Union européenne se fasse en en dégradant leur modèle social et vous avez de l'autre côté des pays du de l'Est de l'Europe, qui considèrent que leur croissance économique repose sur le dumping social aujourd'hui pour pouvoir avancer, nous avons mis en avant la nécessité que dans le prochain budget européen les fonds et notamment les fonds de la cohésion soit conditionnée à la convergence sociale qu'on ne puisse pas en même temps temps maintenir une politique de l'eau costaud de travailleurs de 2ème classe et financer cette politique par des fonds européens, il nous paraît essentiel de nous faire entendre sur ce point, s'agissant du mode de décision éventuellement de recourir à une Europe différenciée je nous met en garde, s'agissant de l'Europe sociale, il est possible qu'une avant garde puisse avoir des projets plus ambitieux mais nous risquons d'entretenir une concurrence interne à l'Union européenne entre États-membres, alors même que nous le voyons dans le climat économique et commerciale du moment nos concurrents à travers le monde ils sont surtout en dehors de l'Union européenne et nous devons renforcer notre cohésion entre États-membres et donc travailler à une plus grande convergence sociale. Merci, la parole : thème Madame Saint-Pé.

ont avancé des propositions pour un pacte finance-climat ambitieux dans un contexte international ou le ou les États-Unis se désengage de l'accord de Paris et laissent entendre un éventuel retour négocié dans l'accord, l'Union européenne doit afficher une volonté ferme de conduire la transition énergétique et de sauver le climat alors Madame la Ministre, dans la perspective du cadre financier pluriannuel post-2020 l'énergie sera-t-elle une priorité politique, la France va-t-elle impulser une dynamique auprès de l'Union pour faire reprendre le Leadership à l'Europe en matière de finances climat s'achemine-t-on vers la création d'un vrai budget climat au niveau européen permettant d'investir massivement dans la recherche dans la transition énergétique de financer le développement durable des continents voisins avant que les migrations climatiques ne secouent l'Europe encore davantage, oui, l'enjeu est grand, telle que l'a déclaré le président de la République et le défi reste à relever, je vous remercie. Madame la Ministre votre réponse. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Saint-Pé. Nous avons défini un ambitieux cadre énergie-climat pour 2030 dans l'Union européenne, qui repose sur 3 grands objectifs : au moins 40 pourcent de réduction des gaz à effet de serre comparé à notre nos émissions de 1990 au moins 27 pourcent de renouvelable dans le mix énergétique européen, et au moins 30 pourcent d'efficacité énergétique, nous sommes en train de négocier les législations qui décline ses objectifs de manière opérationnelle, on peut dire que le travail est déjà accomplie au 2 tiers et non peut espérer qu'il sera totalement terminé à la fin de cette année côté climat nous venons de réviser le rénover le marché du carbone et les politiques de réduction des émissions hors marché hors marché du carbone, du côté de l'énergie, nous achevons la négociation du paquet qu'on appelle pour une jeune énergie propre pour tous les Européens de novembre 2016, composée de huit directives et de règlements sur l'énergie, il y a 2 enjeux majeurs, mettre en place une gouvernance européenne des politiques énergétiques en demandant à chaque État-membre de se doter d'un plan national énergie-climat qui s'inscrivent dans l'atteinte des objectifs européens et adopté le fonctionnement du marché de l'électricité au caractère raciste pardon particulière des nouvelles sources d'énergie renouvelables dont on sait qu'elles sont souvent intermittente pour leur permettre progressivement de trouver à se financer sur sur le marché.

il n'en demeure pas moins qu'il reste encore un certain nombre de difficultés, je vais parler elle des territoires et en particulier du secteur primaire pour constater d'une part dans des secteurs où la politique européenne est importante, que l'on constate un certain nombre de conditions de distorsion de concurrence, je pense au secteur affecté affecté en dans notre pays pour lesquels le gouvernement est en train de se chercher des solutions permettant de bien rémunérés et les producteurs, il s'agit du porc et du et du lait dans le domaine porcin, par exemple, on s'aperçoit qu'en Allemagne les exploitations sont indument accompagné aidés financièrement par les pouvoirs publics, ce qui conduit à des distorsions de concurrence aux Pays-Bas, on s'aperçoit que qu'un certain nombre d'exploitations fantômes sont identifiés, et on s'étonne après qu'il y a 360000 tonnes de l'de stocks de poudre de lait au niveau de l'Europe qu'il faudrait aussi pouvoir évacuer au plus tôt, donc il est important que le gouvernement puisse faire en sorte que les conditions de concurrence sur l'ensemble du territoire européen puisse être les mêmes de façon à ne pas désavantager nos producteurs de la même façon, on peut se réjouir qu'au niveau de du Brexit, un accord puisse être trouvé, je voudrais là aussi appelé l'attention du gouvernement sur la situation de nos marins pêcheurs puisque la France est la 2ème puissance maritime du monde, au plan de l'étendue du domaine maritime et on sait que les zones de pêche sont pour l'essentiel dans les britanniques donc il importe là aussi que ne soient pas laissés pour compte, ces professionnels, mais que dans l'accord avec les Britanniques que le gouvernement prenne bien en compte cette dimension de pêche qui est de zones de pêche qui est importante pour l'ensemble de nos pêcheurs. Merci, la parole à Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur qu'à Nevers, vous avez raison, la politique agricole commune et historiquement l'une des premières politique intégrée de l'Union européenne, l'une des plus importantes et pas, pas seulement en termes de crédits alloués, mais parce qu'elle permet l'autonomie, la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, cette politique souffre de défauts et lorsque nous appelons à la réforme et à la rénovation de la politique agricole commune, c'est pour mieux traiter les sujets que vous avez mentionné en particulier pour pour mieux encourager l'organisation et je dirais la durabilité de nos filières pour éviter évidemment tout risque de distorsion c'est ce pour éviter ce risque de distorsion que nous sommes défavorables à la renationalisation de la politique agricole commune, sans quoi les modèles agricoles risqueraient de de de diverger bien davantage, vous avez nous sommes aussi très attentifs à ce que la politique agricole commune puisse mieux et la gestion, la prévention et la gestion des crises auxquelles les filières agricoles sont confrontés, vous avez parlé de la situation des marins-pêcheurs, dans le contexte du Brexit je disais tout à l'heure que nous avons obtenu, contrairement à beaucoup de déclarations politiques un peu rapide de certains hommes politiques britanniques, l'accès aux eaux britanniques pour les marins pêcheurs européens soient maintenus dans la période de transition, et il est évident que l'accès des produits de la mer pour les marins pêcheurs les marins pêcheurs britanniques au marché unique européen ne se fera pas sans conditions, ça serait un aspect important de la négociation de la relation future et je tiens à vous dire ici à quel point le négociateur européen, Michel Barnier et sensibilisé à cette question particulière. Merci, la parole est à monsieur Huré. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le projet des pères fondateurs de l'Europe et d'enjeux au Mans fragilisé. Pourtant, il a permis, entre autres, de vivre en paix pendant plus de 70 ans, du jamais vu sur ce continent pour relancer ce projet d'Union sur le continent européen, il faut renforcer les coopérations économiques, sociales, diplomatique et militaire, en y mettant les moyens nécessaires. Les autorités européennes doivent être ferme sur le respect des conditions de coopération. Mais elles ne doivent pas ni donner l'impression. Ni vouloir en régime montée, les pays membres, en les privant, ou en leur donnant l'impression de vouloir les priver de toute expression particulièrement sur ce qui constitue les aspects spécifiques de leur identité. Et manière de vivre ensemble l'union dans ces domaines ne peut se s'imposer Nice décrété il faut laisser au temps le temps et je pense que les générations Erasmus vont y contribuer efficacement les pays de l'Union doivent plus et mieux se parler, s'expliquer, se rassurer les échanges entre les parlements nationaux peuvent y contribuer, mais il faut les amplifier ces démarches initiative parlementaire doit s'inscrire dans toutes les autres actions visant à combattre l'euroscepticisme, voire l'europhobie, le temps presse 2019, 2020 vont être déterminantes et notre responsabilité. à l'égard des générations suivantes comme du monde est grande. Merci madame la ministre. On doit être attentif à entendre les préoccupations des États-membres, c'est ce que fait le président de la République depuis son élection, c'est ce que je fais à ses côtés, nous nous sommes rendus dans un très grand nombre d'États membres de l'Union européenne, nous avons reçu au-delà des contacts que nous avons à Bruxelles l'ensemble de nos homologues nous dialoguons avec tous ferme sur nos convictions, mais dans le respect des préoccupations de nos partenaires, nous n'aurions pas pu. Réussir à renouveler à réviser la directive sur les travailleurs détachés dont on nous avait annoncé qu'elle serait emblématique d'une division entre l'Est et l'ouest de l'Europe, si nous n'avions pas eu cette démarche dans le même temps. Il y a des éléments communs aux États membres de l'Union européenne, l'union n'est pas seulement un marché unique je rajouterais que ça n'est pas non plus seulement un carnet tchèque lorsqu'on adhère à l'Union européenne, c'est qu'on adhère à ces valeurs fondamentales, notamment en matière d'état de droit, de séparation des pouvoirs et ces valeurs démocratiques et on sait que, au-delà d'et membre fondateur de l'Union européenne, les pays qui ont rejoint l'Union par la suite l'ont fait en sortant de dictature ou en sortant d'années de joug soviétique et que c'est justement parce qu'ils aspiraient à rejoindre ses valeurs que ils sont venus dans l'Union européenne, nous, nous le payons pas et ne doivent pas l'oublier non plus, s'agissant des progrès que nous pouvons faire aujourd'hui dans l'Union européenne, nous considérons que l'Europe différenciée, n'est pas un gros mot que sur certains sujets. Ceux qui veulent aller de l'avant, doivent pouvoir le faire sans forcer ceux qui ne sont pas prêts ou qui n'en ont pas la volonté, mais sans être bloqués par eux non plus. Merci, la parole à Madame Jourdas. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues j'aborderai ici le volet du Brexit concernant la politique de sécurité de l'Union européenne et particulièrement du répercussion en matière de coopération policière policière et judiciaire, que le retrait du Royaume-Uni va entraîner la nécessité de promouvoir la sécurité au sein de l'Union européenne a toujours été d'une importance cruciale, le traité de Lisbonne à donner un nouveau souffle à ce combat en octroyant de nouvelles compétences à Eurojust et Europol, ce sont donc des acteurs clés non seulement pour la sécurité intérieure, mais aussi pour la sécurité extérieure, puisque ces agences coopèrent au-delà des frontières de l'Union avec Frontex des partenaires extérieurs et des États tiers ce n'est un secret pour personne, nous vivons dans un monde globalisé, où les activités criminelles ne se limite pas aux frontières ni à un territoire de l'Union, terrorisme, trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic d'être s'humains, contrefaçon et j'en passe, ce sont autant de menaces criminelles qui se jouent en dehors des frontières étatiques. Aussi, malgré son retrait, il est essentiel que le Royaume-Uni puisse continuer à coopérer avec Europol et Eurojust, agence pour lesquels il a eu un rôle déterminant actuellement le le directeur d'Europol est anglais ce pays 8 contribue ardemment à la base de données d'Europol de plus sa sortie d'Eurojust et porteuse de conséquences lourdes, notamment en matière de reconnaissance des décisions de justice et de sortie du mandat d'arrêt européennes le Brexit constitue donc un challenge majeur pour Europol et Eurojust dans le même temps qu'une réduction de la sécurité des citoyens de l'Union est inenvisageable, dès lors, Madame la Ministre, j'aimerais connaître les modalités de coopération qui peuvent être développés entre le Royaume-Uni et ces agences afin de continuer à l'avenir le travail entrepris et à et savoir seront les négociations d'un se nomme domaine. Merci madame la ministre. C'est le président, Madame la sénatrice Jourdas, je partage votre analyse sur le fait que on matière de criminalité en matière de lutte contre le terrorisme, les frontières n'existent pas, on ne peut, de ce point de vue que regretter le départ du Royaume-Uni, parce que si il a jusqu'à présent largement contribué à Europol, dont je précise, la nouvelle directrice exécutive et belge, je viens de la rencontrer, il en a aussi énormément bénéficié cette absence de respect des frontières des réseaux criminels ou des réseaux Trigny terroriste est une autre raison pour renforcer notre partenariat avec les Balkans, dont je parlais tout à l'heure, puisque ces enjeux plus de contrôler le terrorisme et lutte contre la criminalité organisée et intéresse aussi ces États tiers mais qui sont des états proches s'agissant du Royaume-Uni, il est évident que les 27 sont déterminés à maintenir un partenariat étroit avec les Britanniques en matière de justice et et d'affaires intérieures qu'il s'agisse de coopération judiciaire ou de coopération policière, ces aspects seront traitées dans la la manière dont nous allons concevoir la relation future avec le Royaume-Uni ces aspects sont d'ailleurs clairement mentionné dans les directives de négociations qui vont être données à Michel Barnier après le Conseil européen de demain et après-demain. Merci monsieur Cadic pour 2 minutes. Si Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues Madame amis j'ai été quand même un peu surpris par vos réserves concernant les Balkans sur la date objectif puisque s'il me semblait que monsieur Macron dans son discours à la Sorbonne nous permettait de penser qu'on aurait dans un horizon proche une adhésion : par exemple, la Serbie et du Monténégro, David Davis et Michel Barnier, se félicite de cette sur la question des citoyens, lundi dernier, je suis heureux, j'en fait partie et j'ai dans la main, un livre de témoignages qui sont poignants, donc sur les Européens qui vivent au Royaume-Uni et j'espère, Monsieur le Président, que nous aurons l'opportunité de recevoir un jour dans notre commission ses représentants, selon la formule de Donald Tusk, il est utilisé hier dans sa lettre au Conseil, les 3 millions de ressortissants européens au Royaume-Uni et le 1000000 de Britanniques dans les autres pays membres pourront continuer de vivre sans ressentir les effets du Brexit les personnes concernées ne partage pas cet optimisme, j'étais lundi à une journée de conférence à Londres, intitulée Shue Da IST auch ou Daillebaud. J'ai longuement parlé avec les 3 millions et British finira, les associations de citoyens ont l'impression d'un accord qui se fait sur leur dos pour les ressortissants européens au Royaume-Uni, ils devront se soumettre à une procédure de demande de statut migratoire pour remplacer leur statut actuel dérivée du droit européen, ils n'ont pas de certitude de succès car la procédure n'est pas déclaratoire comme à présent. Et certains droits sont perdus la jeunesse européenne en fera les frais, par exemple, la jeune Français de Londres ne pourra pas ramener sa future femme sous les règles du regroupement familial, passée une date butoir. Pour les Britanniques, en France et dans les autres pays membres, le problème est différent, ils perdront leur liberté de circulation et seront obligés de rester dans leur pays d'accueil actuelles. ça semble être encore une discrimination. Est ce que la France est prête à soulever ces questions et exiger que les réserves des associations de citoyens soient prises en compte, je vous remercie. Merci madame la ministre, Monsieur le président, Monsieur le Sénateur Cadic l'accord auquel l'Union européenne, les 27 et le Royaume-Uni sont parvenus au mois de décembre qui est traduit aujourd'hui dans le projet d'accord de retrait, c'est un accord qui prend en compte la situation des citoyens européens au Royaume-Uni, de même que celles des citoyens britanniques résidant dans l'Union européenne, cet accord permet que les Européens au Royaume-Uni continue à travailler, a redit à résider à étudier au Royaume-Uni dans les mêmes conditions qu'actuellement, qu'ils continuent à bénéficier de la même protection sociale mais par exemple du même accès aux soins, c'est un élément essentiel auquel nous avons été extrêmement attentifs et nous avons également obtenu que les citoyens arrivant au Royaume-Uni pendant la période de transition ne soient pas discriminés par rapport à ce qui s'y trouvaient avant le 29 mars 2019 ce n'était pas acquis au départ cette un succès de la négociation qui est menée par Michel Barnier, nous allons continuer à être extrêmement attentifs à la situation des Européens, en particulier de no 300000 compatriotes notre consulat à Londres, être en contact étroit avec les associations qui les représentent, les autorités britanniques multiplient les réunions d'information concernant la situation future des ressortissants européens alors malgré tout, je dois, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que devenant États tiers le Royaume-Uni n'accordera pas à ceux qui rejoindront le Royaume-Uni, après la fin de la période de transition, les mêmes avantages que à des ressortissants de l'Union européenne, c'est une des raisons qui nous fait regretter la décision du Brexit mais c'est une décision souveraine du peuple britannique et nous avons réussi à en accompagner les effets de la meilleure manière possible mais resteront de toute façon, très attentifs à la situation de nos compatriotes. Dernière question de ce débat monsieur me rend pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, juste retour aux remarques comme mon collègue, une heure et je suis effectivement très inquiet moi du devenir de l'Union européenne, il me semble que j'ai posée rapidement 3 questions, c'est que l'Europe, de quoi parlons-nous quelle identité européenne Europe elle est perçue par les peuples comme étant très très éloigné de préoccupation et au fur et à mesure des élections, nous voyons monter Les mais europhobe, on va les appeler comme ça, pour simplifier, on se pose la question du jour des frontières ou est-ce que s'arrête cette Europe et a je voudrais poser 3 questions : la première concerne la Turquie, quel est ce drôle d'allié qui occupe depuis plus de 40 ans qui se permet aujourd'hui d'occuper une partie de la Syrie qui massacrent nos alliés objectifs

à travers les siècles, l'Angleterre, l'Angleterre aujourd'hui, on peut se rappeler ce que disait le général de Gaulle, de l'Angleterre choisira toujours le grand large, et en fait, l'Angleterre a gagné l'Europe est un continent qui s'exilent s'exacerbe réellement la divergence sociales et fiscales, quoi de rapports entre des taxations, à 16 pourcent en Irlande, au sein du Bénélux de Holding qui permettre les optimisations fiscales ou les travailleurs français et la France et les entreprises françaises sont les premières victimes, tout ça, et dernier point très rapidement, Schengen, Schengen, il y a eu une commission des Affaires européennes, qui annonçait la décision du Conseil et qui a émis un texte que je vous invite mes chers collègues, allez voir c'est le texte E 12 809 concernant les acquis Schengen et notamment concernant la France, la France en 2016 madame la Ministre, hé bien loin de ce que souhaitaient l'Europe qui souhaitait déjà pas grand-chose concernant Schengen, elle est déjà incapables notamment sur tout ce qui est sécurité intérieure concernant voici les entrées des du territoire, d'assurer la sécurité correctement, donc une réponse qu'elle est, les mesures, quelles sont les mesures prises par la France pour respecter je mets entre pointillés les acquitte Schengen. Merci madame la ministre, votre réponse. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur me en ce sont série de remarques plus que que des questions, donc je vais essayer d'aller vite, la Turquie, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est un partenaire indispensable dans la lutte contre le terrorisme, nous lui devons pouvoir identifier et notamment les apprentis djihadistes français qui se rendent en Syrie ou en Irak, en passant par son sol, ne l'oublions pas

nous le comprenons que la Turquie pénètrent profondément dans le territoire syrien et cause des déplacements de population et une aggravation d'une situation humanitaire qui est déjà dramatique, nous lui demandons de permettre l'aide humanitaire et de permettre aux citoyens syriens de de revenir chez eux, vous avez parlé de du Royaume-Uni, vous avez parlé de des divergences fiscales, sociales que l'on constate constate au sein de l'Union européenne, c'est exactement la position du président de la République de considérer qu'aujourd'hui le projet européen ne peut continuer, ne peut s'approfondir qu'à condition de travailler à plus de convergences sociales et fiscales, sans quoi le fait d'avoir une monnaie unique ne suffira pas à renforcer l'Europe comme puissance économique, c'est la raison pour laquelle, par exemple en matière fiscale, nous plaidons pour la mise en place d'un corridor d'sur d'sur l'impôt sur les sociétés et c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, nous sommes favorables à conditionner le versement de certains fonds européens au respect de la convergence, fiscale et de la convergence sociale s'agissant de Schengen, nous considérons aujourd'hui que il ne l'heure n'est pas venu d'élargir Schengen, même si certains États membres sont candidats à l'adhésion à Schengen, tant que nous n'avons pas réformer et renforcer Schengen en travaillant, en particulier un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne pour cela, il faut davantage de moyens, davantage d'effectifs, nous nous y sommes zinc engagé, nous travaillons aussi à une meilleure interopérabilité de nos systèmes d'information entre États-membres de l'Union européenne, ce sont des enjeux que nous prenons très au sérieux. Merci madame la ministre, le rapporteur, le président de la commission des Affaires européennes, veut prendre la parole. Ce qui n'est pas prévu. pour répondre à essayer collectivement avec beaucoup de d'humilité sur ce point, j'ai senti au travers des différentes questions je dirais la transcription de l'inquiétude que ressentent nos concitoyens au travers des questions des différents collègues nous vivons un monde qui n'a jamais été aussi incertain et le souhait de Françaises et des Français, c'est d'avoir une Europe qui protège, je n'ai pas d'une Europe protectionnisme l'Europe qui protège, elle n'avait pas été spécialement conçu, si vous voulez, avec la vague migratrices que nous avons connu l'espace Schengen où où où je dirais l'agence Frontex n'avait pas été dimensionné pour l'ampleur de cette vague de migration et les réactions de l'Europe, hé bien, elles se font à la vitesse à sa vitesse et sa vitesse et celle des 27 États-membres notre collègue Madame Robert a a a souligné pourquoi toujours avoir des règles à l'unanimité l'unanimité c'est souvent sur les questions je dirais financières mais souvent dans d'autres domaines se sondés majorité qualifiée et là rassemblé 27 États-membres sur une majorité qualifiée, ce n'est pas toujours si vous voulez, extrêmement évident donc une Europe qui protège en fin de compte, quand on regarde ça avec le temps, regardez ce qui s'est passé après Lehman Brothers 2008, l'Union européenne a fini par constituer si vous voulez un corpus réglementaire qui sur le plan de l'Union des marchés de capitaux qui sur le plan de l'union bancaire a fini par obtenir quelque chose de très solides, mais ça a mis du temps, une Europe qui protège, c'est aussi une Europe qui, au travers de la coopération structurée permanente élabore tout doucement une défense européenne, mais elle a aussi sa demande je dirais du temps et une Europe qui protège, c'est aussi une Europe qui essaie de corriger ce qui a été votée, évoqués par notre collègue qui en avait sur je dirais les fraudes, les dérives de certains États parmi les plus je dirais les États fondateurs travers de la fraude à la TVA sur la filière porcine, on l'a dénoncé l'Europe va corriger va sanctionner, de même que sur les Pays-Bas madame la minute a reçu un courrier de ma part sur ce point précis, il n'est pas normal si vous voulez qu'au sein même de l'Europe, nous aurons, nous ayons des distorsions je dirais sur ces problématiques, mais c'est pas ça l'Europe, chacun peut diverger peut je dirais s'emballer, entre guillemets, là ça va être corrigé, c'est comme ça aussi que fonctionne l'Europe je crois ce qu'il faut retenir et ce sera ma conclusion, c'est que, il faut trouver un juste équilibre entre l'Europe des coopérations renforcées, qui nous permet d'aller plus vite, sans avoir une Europe à double vitesse, peut-être une Europe avec des premiers de cordée et puis une Europe si vous voulez qui assurent une cohésion de l'ensemble des 27 c'est l'Europe des valeurs telles que a décrit ou à souhaiter encore une fois, notre collègue Benoît Huré, donc l'Europe, hé bien, si vous voulez, c'est une construction qui je dirai n'a jamais de fin, parce qu'elle est toujours à parfaire, merci.

et puis nous allons reprendre avec l'examen du projet de loi relative à la protection des données personnelles, enfin, à la suite de l'examen de cette loi.

cette loi. Séance et reprises lors du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relative à la protection des données personnelles dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 46 rectifier au sein de l'article 12. Il y a 14 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur patients. Monsieur oui, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Georges Patient nous propose là de rétablir la ligne 5 dans sa rédaction d'origine telle qu'été présenté par le gouvernement, il rappelle que l'article 89 du RGPD permet des dérogations en dans le domaine des archives et l'argument de manière très précise son son point de vue dans un amendement dont la clarté n'a échappé à personne, lors de sa lecture attentive, je vous remercie,

Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues de l'introduction d'un droit de rectification des archives en apparence anodine pose plusieurs questions qui méritent d'être débattus ici, je me réjouis qu'elles aient trouvé tant d'échos dans notre chambre, il y a d'abord la question de l'authenticité des archives qui pose un problème scientifique, le droit de rectification de nos contemporains en mémoire de leurs aïeuls au prétexte de telle ou telle arguments justifient d'altérer des documents à valeur historique ne s'agit-il pas là d'une pratique qui risque de nuire au débat scientifique de chercheurs visant à déterminer des vérités historiques ou sociales seront selon des règles déontologiques qui leur sont propres, même les erreurs une révèle une part de vérité en outre des rectifications sont déjà possibles par le biais de publication, commentant ces archives, il y a également la question plus prosaïques de la charge de travail que ces modifications impliqueront pour les archivistes largement sous-estimé ici, madame la rapporteur nous soulignons votre effort de compromis, mais nous considérons que la rédaction que vous proposez reste insuffisamment protectrice, le principe d'authenticité des archives ne peut s'accommoder de nuances, je vous remercie. Oui, Monsieur le Président merci madame le Garde des Sceaux juste donc reprendre un petit peu les arguments bien entendu qui viennent défendue par notre collègue on en précisant qu'il est nécessaire que les traitements mis en 9 par les services publics d'archives déroge au droit de rectification, les traitements visés par la suite, le 12 ne porte que sur les archives définitives archives historiques et en aucun cas sur les archives courantes et intermédiaires, également appelé archi-vivante qui sont, quant à elle bel et bien soumis au droit de rectification, alors les 2 principes importants c'est intégrité et authenticité, les informations que comportent les archives historiques sont souvent périmés incomplètes du seul fait de leur ancienneté, elle comporte parfois des inexactitudes et des erreurs volontaires accorder un droit de rectification sur ces archives historiques reviendrait à porter atteinte à leur authenticité, qui est à distinguer de la notion de véracité, or la mission de l'archiviste, bien entendu, c'est la garantie de l'authenticité des documents et puis comme vient de le dire, notre collègue ce droit rectification sur des archives historiques générer de surcroît une charge de travail extrêmement lourde quand on songe au kilomètre de linéaire que ça peut représenter au niveau des archives, qu'elles soient nationales, départementales ou communales. Si pour l'amendement 53 identique de Monsieur Loïc Hervé défendu de Monsieur Mazuz hier, il n'est pas là donc saute. Et l'amendement présenté par le gouvernement numéro 90 Madame la ministre Je suis président, mesdames les sénatrices messieurs sénateurs, donc, cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 12 du projet de loi qui prévoyait une dérogation au droit de rectification pour les traitements à des fins archiviste hic dans l'intérêt public, cette dérogation ne vise que les jardins que les archives dites historiques qui sont déjà anciennes et conservés par les services publics d'archives et non les archives vivantes effectivement soumises, quant à elle, au droit de rectification, elle garantit leur intégrité et leur authenticité au regard de l'histoire, s'agissant des archives historiques, il convient de distinguer le caractère original et authentique des documents de la véracité de l'information qu'ils contiennent les services d'archives ont pour mission de conserver des documents citant authentique et c'est aux chercheurs, aux historiens de les apprécier pour éventuellement apporter un regard sur la véracité des informations qu'ils contiennent par ailleurs la rectification de documents qui sont vieux de 20, 30, 40 ans ou plus, constituerait une charge démesuré, me semble-t-il, pour les services publics d'archives qui conserve, nous le savons, des kilomètres d'archives et des centaines de de téraoctets de données cet exercice de ce droit s'avérait en réalité impossible en raison de l'extrême difficulté pour ses services de vérifier l'exactitude des informations demandées. Merci madame Sylvie Robert pour le 136. Défendue. Amendements sont 49 rectifier monsieur Delcros. Toujours eu. Oui s'inscrit bien sûr dans la continuité des des précédents et moi, je veux dire, c'est que ça me paraît extrêmement important de rétablir cette dérogation au droit rectification qui bien entendu reste valable, comme ça a été dit, pour les archives vivantes, c'est, c'est c'est très important parce que je pense qu'il faut protéger ses articles historiques, elles contiennent des données qui sont exacts au regard de la réalité des faits de l'époque, d'autres qui sont inexactes, parfois 2, parfois de façon involontaire, parfois de façon volontaire, avec des objectifs très précis, on a tous en tête et des exemples dans l'année dernière dans ces dernières périodes tragiques de notre histoire du XXe siècle et c'est extrêmement important que les historiens que les chercheurs comme ça a été dit, puisse disposer de toutes les données qu'elles soient exactes, qu'elle soit inexacte parce qu'elles permettent de comprendre ce qui s'est passé et donc elles permettent au final d'écrire l'histoire d'analyser l'histoire d'écrire l'histoire et de la faire comprendre à la population, donc je pense qu'on est sur un sujet qui est extrêmement important et je pense que ce serait une erreur

Si vous m'y autorisez monsieur le président, pour la clarté de la discussion, je vais défendre l'amendement tout en présentant l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements, discussions communes. C'est un peu compliqué puisqu'il y a des amendements, discussions communes qui ne sont pas encore défendu donc vous donner un avis avant même qu'il soit présenté. moins pour ceux qui ont été présentés, oui, très bien, très bien, très bien. Depuis la fin des années 70 l'articulation entre les principes régissant respectivement la conservation des archives, l'accès aux documents administratifs et la protection des données à caractère personnel Africom fréquemment soulevé des difficultés, je tiens d'abord à dissiper quelques malentendus le droit en vigueur ne prévoit aucune dérogation au droit de rectifier des données personnelles inexactes au bénéfice des services publics d'archives, il prévoit seulement une dérogation à la durée normale de conservation des données une dérogation aux obligations de confidentialité une dérogation au droit d'accès des personnes physiques aux données personnelles qui les concernent telle qu'il est défini par la loi Informatique et Libertés, une dérogation au droit d'opposition à voir ces données traitées le droit de rectification est strictement encadré par le droit français communautaire, comme l'a confirmé le contrôleur européen de la protection des données, il ne s'applique qu'aux données objectives et factuelle pas aux déclarations subjectives qui, par définition, peuvent être erronée d'un point de vue factuel, la CNIL nous assurer que cette interprétation étroite du principe d'exactitude correspondait en tous points sa pratique le droit de rectification n'implique pas d'effacer des données inexactes, il peut être fait droit, par exemple l'en apposant une mention document en ajoutant au dossier des pièces complémentaires comme tous les droits reconnus aux personnes physiques sur leurs données personnelles ce droit, c'est un au décès de l'intéressé et n'est pas transmissible aux héritiers, comme c'était le cas jusqu'en 2004 en revanche s'est mise au point étant faite, la question demeure : faut-il introduire une nouvelle dérogation au droit de rectification au bénéfice des services publics d'archives une telle dérogation pourrait être justifié d'une part par la nécessité de maintenir de maintenir l'intégrité des archives, d'autre part par les règles de communication des archives publiques qui protège dans une certaine mesure, les personnes vivantes contre les atteintes à la vie privée, puisqu'elle prévoit des délais de communication plus ou moins long néanmoins ces délais l'empêche pas que les documents soient communiqués voire largement diffusé avant la mort, désintéressé et c'est bien là notre problème en outre les archives peuvent dans certains cas être communiquée avant l'expiration des délais légaux et l'administration des archives conservent le droit d'ouvrir des fonds d'archives à tout moment avec l'accord de l'administration, elles émanent. La commission des lois, la semaine dernière, estimez légitime qu'une personne vivante ayant connaissance du fait qu'un document d'archives publiques la concernant, contient des informations d'inexactes puisse en obtenir la rectification, il convient d'opérer une juste conciliation entre les objectifs d'intérêt général, poursuivi par les services publics d'archives et la protection des droits des personnes sur leur donner, on ne peut ignorer le préjudice que pourrait causer à ces personnes la publicité donnée à des informations factuellement erronée, j'aimerais mentionner un exemple qui peut peut-être nous aider à réfléchir sur ce sujet délicat en 2013, les ministères de la Défense et de la culture ont demandé à la CNIL, l'autorisation de procéder à la numérisation à l'indexation et la diffusion sur internet des registres matricules du recrutement militaire des soldats ayant participé à la première guerre mondiale, ces registres matricules comprennent entre autres des données sensibles issues du dossier militaire des soldats blessure est un état général Santé Maladie contamination, par conséquent, il avait été prévu d'étendre à tout internaute le droit de demander la rectification des données inexactes, ce qui est exceptionnel des bases de données d'indexation et des registres matricules numérisés, la CNIL avait alors souligné l'intérêt d'une telle disposition relevant qu'aucune analyse quant à l'exactitude des données n'avait été préalablement mené et que les pratiques suivies pour constituer un registre matricule varier d'un bureau de recrutement à un autre bien sûr en 2013 il y avait plus beaucoup de combattants de cette guerre, mais ces soldats auraient-ils voulu je vous pose vraiment la question, ces soldats auraient-ils voulu que des informations fausses les concernant soient diffusées auprès du plus large public, même après leur mort, que dire de leurs enfants ou de leurs petits-enfants qui pouvait voir la mémoire de leur père ou de leur grand-père injustement. Afin d'apaiser ces inquiétudes, je propose par l'demande mon numéro 152 d'expliciter dans la loi que l'exercice du droit de rectification n'implique pas d'effacer les données inexactes mais qu'il peut y être fait droit, soit en apposant une mention rectificative en marge du document, soit en y annexant un document rectificatif plusieurs amendements de nos collègues vise aussi à supprimer le renvoie à un décret en Conseil d'État ajouté par la commission des lois pour tenir compte des observations de la CNIL, en effet, le RGPD prévoit que la loi nationale peut déroger au droit reconnu aux personnes physiques sur leur donner en ce qui concerne les traitements à des fins archiviste hic dans l'intérêt public, mais ces dérogations ne sont permises que sous réserve de garanties appropriées et dans la mesure où ces droits risquerait de rendent impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques de ces traitements, il convient donc de préciser par décret en Conseil d'État, la portée de ces dérogations, les garanties apportées aux personnes concernées et les limitations apportées à la diffusion des données traitées, notamment en ce qui concerne l'indexation de ces données sur les moteurs de recherche je demande donc au nom de la commission que l'amendement numéro 152 soit mis aux voix par priorité. Donc ça au moment venu, on demandera au gouvernement s'il est d'accord et s'il est d'accord, ça vous sera accordée mais. S'il n'est pas d'accord, ça vous sera pas accordé, ce sera un vote du Sénat, il y aura, ça c'est ça sera un vote d'accord, hé bien on continue avec l'amendement 41 Maryse Carrère ou Madame Coste dans le même esprit que notre précédent, maintenant il est défendu très bien à nouveau Monsieur Oui, Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux par Artis 89 le RGPD permet aux traitements à des fins archiviste hic dans l'intérêt public de déroger à certains droits en contrepartie de conditions et garanties appropriées, cette disposition ne concerne que les archives définitives archives historiques et seulement les traitements des services publics d'archives qui ont pour mission de collecter les archives publiques à l'issue de leur durée d'utilité administrative, or la gestion de ces archives est encadré par un ensemble de textes législatifs et réglementaires très dense, plus de 150 disposition dans le code du Patrimoine des dizaines de dispositions inscrites dans d'autres textes, notamment dans les Côtes des relations entre le public et l'administration et plus d'une centaine d'instructions ministérielles toutes les étapes de la chaîne archiviste il trie traitement Conservation et communication sont ainsi juridiquement très encadré, ce corpus législatif et réglementaire, et le respect des normes en matière d'archivage électronique apporte des garanties fortes et suffisante dès lors une nouvelle couche de droit ne ne semble pas nécessaire et apporterait une complexité inutile par ailleurs, le décret d'application de l'article 6 de la loi pour une République numérique dont la parution après avis de la CNIL devrait intervenir prochainement déterminera précisément les conditions de diffusion sur internet, des documents d'archives et de leurs instruments de recherche des dispositions réglementaires supplémentaires sont donc inutiles pour les traitements archiviste mises en oeuvre par les services publics. D'archives, merci Monsieur Mazuz hier sur l'amendement 61, il n'est toujours pas là, amendement 91 du gouvernement Madame la ministre

permettent de déroger à certains droits des personnes concernées, le RGPD n'interdit pas de procéder à des traitements de données archivées à d'autres fins que les fins archiviste dans l'intérêt public, les fins de recherches scientifiques ou historiques ou les fins statistiques néanmoins les traitements en question sont soumis au régime de droit commun du RGPD et de la loi Informatique et libertés, ces traitements ne bénéficient pas des dispositions spécifiques attaché au traitement précités, la nouvelle rédaction de l'année de l'alinéa qui impose certaines conditions spécifiques n'est pas conformes au RGPD le présent amendement comme ceux proposés par plusieurs sénateurs a pour objet de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

mettre un peu d'ordre dans cette discussion puisque Madame Joissains demande que son amendement arrive au vote en prévoit priorité je vais signaler que d'abord. Il faut l'avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, je ne m'oppose pas à la demande de priorité qui a été demandé par Madame la rapporteur je rappelle toutefois que je suis très attaché à ce que l'amendement du gouvernement numéro 90 et les amendements identiques puisse être adopté et donc évidemment, voilà, je voulais juste souligner cela. Madame la Ministre, pour votre information, si ça arrive, en priorité, c'est le si vous dites d'accord, c'est d'accord, mais ça ne remplira pas ce que vous demandez, puisque cet amendement fera sauter le vôtre.

Oui, enfin bon. Eh bien nous, tout le monde a eu toutes les données, donc je vais tout de suite dire avant de passer au vote de l'amendement de Madame Joissains que les amendements qui vont. Tomber automatiquement son 46 rectifier de monsieur passion et les amendements identiques 40 42 53 90 136 et 149 rectifier.

Monsieur le président, je suis favorable à mon amendement et aux amendements identiques, c'est-à-dire mon amendement, c'est le 90 et aux amendements identiques, je suis défavorable aux autres, donc je suis défavorable à l'amendement 152. Oui, j'ai bien vendu par Madame Joissains. Donc, on a l'avis du gouvernement, est ce qu'il y a une explication de vote sur le 1er amendement puisqu'on va commencer les votes de Madame Joissains. Le 152 oui, allez-y monsieur. merci Monsieur le Président, si, si j'ai bien compris la subtile différence et j'ai cru percevoir qu'il y a quelques interrogations dans l'hémicycle, le but poursuivi le même, mais les moyens d'y parvenir sont en revanche très différents et la rapporteure nous propose de rendre possible de conserver manière dérogatoire la conservation des archives mais de rendent possibles des mentions marginales indifférence du gouvernement et des autres amendements des différents groupes qui propose de conserver les archives dans un cadre dérogatoire, moi ce qui me dérange, un petit peu dans la suggestion et même fortement dans assaut d'un proposition de la rapporteure, c'est que c'est c'est postuler adopté serait cet amendement-là c'est postuler que la vérité d'aujourd'hui et celle de demain. Et je ne suis pas certain que ce postulat soit lui-même une vérité. Quand on parle d'histoire, d'esprit critique, d'analyse, je ne pense pas que le législateur soit le mieux placé et des spécialistes qui prennent différentes sources qui les confronte qui les analysent pourquoi autoriser l'inscription sur les archives de la vérité d'aujourd'hui, c'est ainsi que j'entends l'amendement de la rapporteure et ça me dérange très fortement à la différence des autres amendements notamment du gouvernement.

amendements que dans cet hémicycle, nous avons déposé identiquement et qui va dans le sens du rétablissement du du projet de loi, je voudrais dire que ce que nous présente le rapporteur et finalement un commandement qui veut, qui est une demi-mesure, on l'entend bien, vous avez essayé de trouver une forme comme ça de de compromis demi-mesure mais il y a une chose, je vais peut-être un peu basique dans ma réflexion, mais il y a une chose qui ne que vous ne prenez pas en compte et je ne pense pas que ils satisfassent Les les directeurs des services intéressés, c'est de prendre en considération les aspects pratiques du recueil des rectifications à la fois en termes de coûts indirects, mais aussi de tout ce que les de ce que tout ça, de ce que ça va entraîner en terme d'opération et je pense qu'en faisant cela, il faut quand même aussi voir un peu les les incidences que ça, ça peut avoir, donc je pense que nous sommes un certain nombre à à à être d'accord pour hé bien continuer à défendre nos amendements. Alors Monsieur bas. Je vous remercie, Monsieur le Président, je voudrais tenter d'apporter une contribution au débat en vous livrant un éclairage personnel et vraiment personnel parce que je suis passionné par la question des archives et comme ancien président du conseil départemental, je me suis beaucoup impliqué dans ce domaine et pour tout vous dire, le directeur des archives départementales de la Manche n'a pas manqué de m'alerter sur cette question et je comprends sa motivation, il les chartistes, comme beaucoup de nos archiviste, c'est un homme extrêmement cultivé, j'espère que ces compliments iront jusqu'à lui, évidemment, et je vous prie. De m'excuser d'abuser de la prise de parole pour pour les lui adresser mais je trouve ça tout à fait intéressant de se dire que, dans nos archives survive à l'épreuve du temps, de nombreuses inexactitudes qui n'ont jamais été corrigée et qui ont une valeur historique de de très grande importance aussi bien, nous ne pouvons pas nous permettent ici d'adopter une disposition qui effacerait la trace des inexactitudes et empêcherait les historiens de demain de pouvoir exploiter ces Idex attitude pour servir la vérité en quelque sorte, historiques et scientifiques et donc au fond tous les amendements qui seront mis en discussion, je crois, partent de cette idée fondamentale que l'inexactitude a une valeur scientifique et historique au service de la vérité, que devront établir les historiens du futur et là-dessus, pas de débat entre nous, maintenant, comment fait-on, hé bien ce que nous proposons dans l'amendement de la commission il vaut ce qui vaut, nous le pensons qu'il est meilleur que les autres mais chacun des auteurs d'un amendement, le gouvernement le 1er pense aussi que son amendement est meilleur que les autres, alors pourquoi le pensons-nous, pour une raison très simple, c'est que, il trouve une forme de compromis qui consiste à dire la directive le règlement européen, j'ai oublié son nom mais le règlement général pour l'exploitation pour la protection des données, certains l'appellent le RGPD, mais je l'appelle règlement général pour la protection des données, parce que je me dis que tout le monde ne connaît pas le sigle RGPD moi-même j'ai du mal à l'assimiler alors ce règlement général il prévoit effectivement que pour la protection D. D des données on doit corriger les inexactitudes, très bien, mais le le compromis que nous trouvons c'est premièrement les inexactitudes peuvent être corrigés, mais deuxièmement leur trace ne doit pas être effacée, ça c'est simple les inexactitudes peuvent être corrigés, mais simplement quant à la demande de quelqu'un qui est sur une donnée personnelle archivées on où on on est amené à se poser la question d'une inexactitude on met dans la marge que cette inexactitude doit être corrigée, mais on garde la trace de l'inexactitude, c'est pour ça que nous avons pensé que c'était un bon compromis et c'est pour ça que nous vous le présentons en toute bonne foi, en espérant que nos archivistes s'en contenteront. Bien, donc, le débat. Se poursuit puisque Madame Morin-Desailly a demandé la parole. pour avoir été rapporteur de la loi à la dernière loi sur les archives avec mon collègue renégat, René Garrec, je serais plutôt d'avis, j'apporte ses réflexions pour éclairer le débat ne touchez à rien parce que bien entendu il y a ceux RGPD qui nous fait réfléchir sur l'accumulation de données de documents au fil du temps et, au fil d'histoire comment met tout ça en prospectives et s'écrit l'histoire, une histoire des événements, l'histoire de 2 personnages qui ont participé à des événements, mais encore une fois, certains l'ont dit, s'il ne faut pas confondre le rôle de l'historien et de l'archiviste, les archives sont des documents bruts, ce qui compte, on en parlé avec les collègues, c'est leur authenticité après que ces dites d'archives, commente Des Des événements ou fasse des commentaires sur des histoires ou des personnes de leur temps et tiennent des propos exactes ou inexactes, ça fait partie du de commandes archives en tant que telle, en revanche, et Philippe Val a très bien rappelé le rôle de l'historien, ça va être de mettre au regard des unes et des autres archives et de construire l'histoire de décrypter, d'analyser et de mettre en relation en perspective, tout ça, un vrai sujet qui est un rôle très différents, on ne peut réécrire l'histoire, a posteriori que sous le regard de ceux qui en font un décryptage avisé et donc moi je ne serais pas forcément d'avis qu'on touche à quoi que ce soit je vous livre mon sentiment, mais je comprends aussi cette volonté de personnes de vouloir porter voilà à la connaissance générale la vérité, mais la vérité c'est aussi aux historiens de la de la construire et faire la lumière sur sur l'histoire, encore une fois l'les archives sont des documents bruts. Bien la parole à monsieur Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la ministre, chers collègues vont c'est vrai que d'un jour à l'autre, on apprend tous les jours qu'on dit, c'est vrai que notre rapporteur, celui aussi son travail et l'ensemble des collègues de la commission des lois, et le président de la commission des lois, sur un texte qui n'est pas simple faux Hall re re connaître le mérite Laurent revenons tout à fait, c'est vrai, mettre la priorité sur cet amendement, on peut comprendre aussi les attentes et les arguments l'argumentaire aussi qui est fort et et c'est vrai, et le président Philippe Bas, a rappelé le travail j'irai de de celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l'histoire archives locales archives départementales, moi je témoigne modestement, je ne suis pas historien mais je suis géographe donc il y a quand même des Liens avec avec l'histoire et je crois que

dans cette même hémicycle Robert Badinter, nous a expliqué comment il avait sauvé les archives du tribunal de Paris et enfin de la scène à l'époque et comment garde des Sceaux, il avait aussi recherché après une conférence à Vienne, les archives du procès Landru que personne n'avait jamais retrouvé c'est une séance Madame le Garde des Sceaux, que je vous incite à lire, c'est du 8 janvier 2008 comme quoi quelquefois faire 3 mandats d'affilée, ça peut être. Un peu utile parce qu'on a là, on a la même non pas plus mais on a quand même la mémoire, donc ça fait 20 ans que dans cet hémicycle, jour pour jour, on a parlé des archives et je rejoins complètement ce qui est très ce que dit Catherine Morin- Desailly et donc soutenir l'amendement du gouvernement et je vais vous dire pourquoi on parle de on parle de 2 temps différents, le temps de l'des archives est une chose Le Temps de l'histoire en est une autre et moi je suis pas du tout d'accord, parce que les archives, ce n'est pas Wikipédia, monsieur le président de la commission des lois, on ne vient pas apporter une modification ou signaler

parlementaire car je ne l'ai pas lu mais simplement, il me semble absolument évident compte tenu des difficultés de rectification qu'il faut laisser à l'histoire, son rôle et aux archives et aux archivistes le leur et je vous renvoie à ce merveilleux discours de Robert Badinter du 8 janvier 2008 dans cet hémicycle, je crois qu'il a tout dit sur le sujet. C'était il y a 10 ans, 2008. Donc, la parole est à madame Ben Basat. Merci monsieur le président, je me pose la question en tant qu'historien, pour savoir sur la base de quoi vous allez rectifier, c'est ça le problème, ce que vous allez rectifier un nom, bon ça va, bon mais c'est quoi la vérité. Non mais c'est une question naïve mais nous quand nous lisons des archives nous lisons toutes les lignes, nous les commentons de ce qu'il y a pas d'histoire brut l'histoire s'écrit il y a l'histoire, les historiens et ce qu'ils produisent et rectifier au nom de quoi mais quel est ce que votre vérité et plus vrai que la vérité qui sortira de, de l'écriture, mais oui on va, c'est une question que se posent chaque historien lorsqu'il rentre le dans les archives et il se dit est-ce que est-ce que ces archives sont authentiques, en quoi ils sont authentiques, comment je peux les lire, si vous leur donner les clés à partir de votre vérité et vous biaisé un peu l'écriture de l'histoire, me semble-t-il. Alors Monsieur Durand. Merci monsieur le président, oui, moi je, je veux remercier la la la rapporteure pour cette initiative de de compromis qu'elle a fait avec son amendement numéro 152 mais j'en comprends le souhait, c'est-à-dire essayer de trouver quelque chose qui soit équilibré, mais je crois que des sujets des matières sur lesquelles les compromis ne tiennent pas et qu'on finit à avoir une cote mal taillée, et je crois que là on a affaire à une cote mal taillée, on l'a dit la vérité historique et brutes l'histoire c'est le produit d'un regard d'une société à un moment donné, avec sa propre culture, ses propres codes, ses propres références donc essayer d'aller rectifier inscrire en marge ou en annexe une rectification : faut-il revenir sur cette rectification ultérieurement parce que un autre moment, il faudra à nouveau prendre en cours d'autres considérations, ça paraît très compliqué et moi je serais assez favorable à ce qu'on fasse, simple, c'est-à-dire qu'on revienne à la version initiale du texte, on a essayé avec l'article 152 visiblement l'amendement 152 visiblement il fait pas recette il ne satisfera pas les archivistes, donc faisons simple revenons par les arguments les amendements qu'on a, les uns et les autres déposées à la version initiale du texte. Oui, je souscris à ce qui a été dit, parce qu'il ne faut pas confondre la véracité et l'authenticité au niveau des archives, ce que dit Madame Benbassa est intéressant, c'est aux chercheurs et aux historiens, jusqu'à preuve du tout contraire de déterminer par le croisement des sources et l'analyse critique des documents si les faits sont vrais ou pas vrais, et puis il me semble quand même qu'il y a aujourd'hui des textes qui permettent d'entamer des procédures de révision, sans pour autant corriger les originaux et les archives qui sont authentiques, merci. Bien, alors maintenant, madame la rapporteure, vous en profitez pour donner quand même votre avis sur les autres amendements auxquels vous n'avez pas donné encore à votre avis. Merci Monsieur le président. Je Je pense que je, je me suis mal fait comprendre qu'il y a là un vaste malentendu, il ne s'agit pas madame mandat ça de toucher aux archives bien entendu que c'est à l'historien de travailler dessus et que des inexactitudes. Qu'elle recèle, il va pouvoir faire son travail et tiré justement une interprétation de l'histoire, je suis totalement en accord avec ça. Catherine Morin-saillie parlait tout à l'heure du fait que les données étaient parfois subjective et qu'il ne fallait pas y toucher, bien entendu, il y a 2 types de données il y a les données factuelles de type monsieur untel a été jugée telle jour et puis il y a Monsieur X pensée telle ou telle chose de monsieur untel, donc ça ce sont des données subjectives et bien évidemment qu'il ne faut surtout pas toucher à ces données subjectives, il s'agit en l'occurrence simplement lorsqu'il y a des données factuelles qui sont fausses et qui je le rappelle, encore une fois, ne touchent pas des des archives qui, on s'entend, il s'agit d'un droit qui est celui de la personne encore en vie, puisque ce n'est pas un droit transmissible que le droit rectification, hé bien il s'agit pour cette personne et imaginons madame Nathalie Goulet que vous-même vous soyez cité dans un document d'archives qui se retrouvent sur Internet avec quelque chose de faux est ce que vous n'auriez pas le désir parce que ces archives alors que vous êtes encore en vie sont tombés dans les archives publiques de dire : attendez, on garde l'archive, mais moi j'aurais je peux rectifier à côté et rétablir la vérité, et ça je pense que c'est important de pouvoir concilier la vie des archives et la vie de l'individu, je pense véritablement qu'il y a là 2 intérêts majeurs majeurs et que dans la mesure où nous pouvons concilier ses intérêts puisqu'il s'agit juste d'apposer en marge du document voir avec des documents rectificative qui serait à sa suite une vérité purement et simplement factuel qui peut avoir de l'intérêt pour l'honneur des vivants tout de même, nous avons cité tout à l'heure, le problème de de ces messieurs qui était, qui était militaires et leurs familles, oui, non, peut-être pas envie de prendre des choses qui ne sont pas réels, tout simplement, moi je pense qu'il va quand même de la considération que l'on doit à l'individu et nous pouvons tous demain être impacté par une chose de ce type, donc plutôt que d'imaginer que les archives, ce sont des choses, surtout à l'époque d'internet totalement poussiéreuse et qui ne nous concerne pas, finalement, puisque nous ne sommes pas forcément historien tous ici autant que nous sommes, hé bien je dis moi qu'il faut concilier ces 2 intérêts, il y a des archives publiques qui concernent des individus envie le droit de rectification concerne uniquement les individus qui sont en vie et il me semble que ce droit-là est tout aussi important que l'autre, dans la mesure, et c'est là où je reprends ce que disait Catherine Morin-de saillies dans la mesure où il ne s'agit pas du tout de rectifier des données subjectives, mais uniquement les données factuelles qui peuvent. Encore une fois la Madame, la rapporteur. Là je j'ai laissé j'ai laissé une minute de plus à votre réponse parce que je considère vous empiéter sur les autres réponses que vous devez apporter mais il il faut maintenant passer au vote. Alors, ben écoutez, moi j'ai maintenir cet amendement parce que je pense qu'il est une bonne conciliation entre le vivant et les archives publiques et je pense que l'étain il négocie Very. Tables ment l'existence des de droits, donc à partir de là je je me, je ne me sens pas de le retirer, honnêtement, parce que je pense qu'il est vraiment une très belle conciliation après ben évidemment je ne peux or qu'un avis de retrait par rapport aux autres amendements mais je laisse mes collègues décidé. Bien, madame la milice me demande un petit mot, allez-y. Merci Monsieur le Président, et pardonnez-moi de reprendre la parole, c'est simplement pour réagir à ce que vient de la démonstration que vient de faire Madame Joissains et je pense que ça démontre tracions si on n'est pas tout à fait exact parce que ce soit un document et sur Internet, auquel cas il est vivant, ce n'est pas une archive et si les vivants, bien sûr, dans ce cadre-là, on peut opérer la rectification nous c'est tout à fait possible, en revanche, si c'est une archive, le document n'est pas communicable, il n'est pas communicables et donc s'il n'est pas communicable, il faut qu'il reste en l'état, je rappelle que, il n'est pas connue mini-câble entre 50 et 100 20 ans, tout dépend des situations, donc à ce moment-là, personne n'y a accès pendant ce délai-là et au bout de 120 ans ou de 50 ans, les historiens feront leur travail comme j'ai eu l'occasion de le faire moi-même sur des archives 2777 et où j'ai eu repérer des inexactitudes que j'ai eu l'occasion de soulever, mais je faisais un travail d'historien du droit, non pas de l'Aveyron, sur le conseil de chancellerie. Alors c'est la toute dernière intervention avant ce vote de l'amendement de Madame Joissains, monsieur le président de la commission. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie, c'est l'intervention de Madame le Ministre, qui me force à reprendre la parole madame le ministre, on numérise des archives et ensuite on les met sur internet, elle comporte des INEC cette tude qui mettent en cause des personnes vivantes veulent que soient corrigées sanisettes ces inexactitudes, on doit leur permettre de le faire à condition. De ne pas détruire l'archive d'origine et donc le problème se pose véritablement. Bien, alors on passe au vote de l'amendement 152 qui a été demandé par la rapporteure en priorité. Et je vous ai dit les conséquences de tous les amendements derrière qui tomberait donc qui est pour.

qui est contre Il est rejeté par adopter, donc maintenant nous passons à l'amendement 46 rectifier qu'a défendu monsieur alors lui il fait tomber tout. La première série. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, plus la 2ème série des amendements, s'il est adopté. Qui est pour.

non, non, non, attendez, on ne va pas, on va pas recommencer l'amendement maintenant qui va être mis au vote. Fait tomber tous les amendements de la discussion commune qui suivent voilà donc monsieur si vous avez le droit à une explication de vote allez-y si vous le souhaitez. ai une question de procédure, si cet amendement est retiré, il est retiré au profit d'un amendement singulier où nous procédons vote sur l'ensemble des autres amendements. On continue par ordre l'amendement suivant les amendements identiques les votent ensemble et les amendements, discussions communes seulement on les votes séparément, il y a 2 séries d'amendements identiques. La sagesse voudrait que soit retiré au profit de celui du gouvernement, ce qui est légitime et peut-être que cela inspirera

dans lequel est aussi celui du gouvernement, mais ils sont identiques à tous les intervenants de qui, qui ont défendu leurs amendements, donc il est pour.

91 135 donc aussi à l'intérieur, celui du gouvernement sont identiques, qui est pour. Qui est contraint. Qui s'abstient non. Ils sont à adopter : voilà, nous sommes sortis de cette discussion commune. Les amendements adoptés, nous rentrons dans 2 amendements identiques le 92, madame la ministre. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise à rétablir la dérogation au droit de rectification des données à caractère personnel pour les archives définitives comme de d'autres amendements le proposer également cette dérogation, je le rappelle, elle est permise par l'article 89 du RGPD elle était inscrite dans le projet de loi initial et dans son avis sur le projet de loi, la CNIL n'a pas émis de réserves sur ce sujet, il me semble opportun de rappeler que l'article 12 du projet de loi ne vise que les archives définitives comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ou les archives historiques et non les archives courantes ou les archives intermédiaires parfois appelée archives vivantes dont nous avons parlé tout à l'heure qui reste elle soumise bien évidemment au droit de rectification, mais à l'issue de leur durée d'utilité administrative les archives qui sont sélectionnés pour être conservés par un service public d'archives qu'il s'agisse des archives nationales, régionales, départementales communales ne doivent plus être modifiés, c'est l'un des grands principes de l'archiviste hic qui garantit des sources intègre, authentique et non dénaturée qui sont nécessaires, bien évidemment, à tout travail d'historien qui se pencheront donc plus tard sur ces documents, modifier des archives historiques, sous prétexte de rectifier une donnée personnelle reviendrait en réalité à portait atteinte à porter atteinte à l'intégrité original avec un risque de falsification et d'atteinte à son caractère authentique ou bien à altérer un travail futur de recherche, la commission des lois à modifier la rédaction de l'article 36 de la loi Informatique et libertés en prévoyant que les traitements archiviste peuvent déroger à une partie des droits des personnes prévues par le RGPD, mais elle a omis d'inclure le droit rectification dans la liste, ces dérogations l'objet de cet amendement, qui rejoint donc ceux proposés par d'autres sénateurs et de rétablir cette dérogation. Merci madame la ministre, il y avait un amendement identique 144 qui n'est pas défendu puisque monsieur patients seul signataire n'est pas là. Il est signé que par lui et pas par son groupe, donc l'avis de la Commission sur cet amendement du gouvernement. Défavorable, défavorable, nous passons au vote donc. Un avis défavorable à la commission et amendement du gouvernement qui est pour. Qui est contre Il y a un doute, peut-être que les mains doivent se lever plus franchement, donc qui est pour. qui est contre Il était adopté. Donc, nous passons à l'amendement 27 rectifiait terre. Savary à la parole. un alinéa, le but, l'objet de l'amendement, c'est disposer du résultat d'un traitement donné à finalistes et statistiques actuellement ne permet pas d'identifier les personnes dont les données ont servi à la production du des résultats, bien entendu, par conséquent, en absence de dérogations particulières, le responsable du traitement ne peut plus informer directement les personnes concernées de leurs droits, notamment de leur droit de rectification qui permet d'assurer la qualité de la production statistique ni prendre l'initiative de les informer directement de leurs droits d'accéder aux résultats statistiques pourtant prévue au Code des relations entre le public et l'administration le présent amendement vise à préciser les moyens dont peut disposer le responsable d'un traitement de données à finalité statistique pour permettre aux personnes concernées d'exercer effectivement leurs droits, notamment celui d'accéder à l'information statistique, il contribue à produire l'amendement permet ainsi d'assumer une meilleure cohérence dans les faits, avec les dispositions du code des relations entre le public et l'administration merci. Merci l'avis de la commission Madame la rapporteure. La commission demande l'avis du gouvernement. Eh bien, Madame la Ministre à vous. Monsieur le président, c'est un avis défavorable que j'aimais à cet amendement qui vise à permettre donc la conservation données personnelles non nécessaire à un traitement dont la finalité est la production d'une information anonyme, il est donc au contraire, me semble-t-il, au respect du principe de nécessité et de minimisation des données de l'article 5,1 du RGPD la conservation des données personnelles en marge de traitement ayant pour finalité la production de statistiques anonymes aux seules fins de respecter le droit d'information des personnes concernées est également en contradiction avec l'article 11 du RGPD j'émet donc un avis défavorable à cet amendement. Bien, donc un avis, la commission a demandé l'avis du gouvernement est-ce que maintenant elle a un avis puisque le gouvernement a donné le sien. Défavorable, défavorable, donc 2 avis défavorables qui est pour.

Il s'agit de l'amendement de coordination Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, après l'article 12 il y a un amendement de monsieur Loïc Hervé. 80 rectifier. Oui merci monsieur le président, conformément au code du Patrimoine, le service public d'archives d'une collectivité peut mutualiser la conservation d'archives numériques avec un autre service public d'archives, en pratique, cette possibilité ne concerne pas exclusivement les EPCI a fait ce qui était propre, le sens de cet amendement, c'est d'adapter la rédaction de l'article susvisés afin d'étende son Champ d'application à d'autres regroupements qui interviennent également dans le même domaine, donc il s'agit de syndicats mixtes informatique ou de G IP. Merci l'avis de la commission Madame la rapporteure avis favorable, avis du gouvernement, Madame la Ministre. Défavorable, monsieur le président, il me semble que c'est un cavalier législatif en se oui, mais je trouve que, nous trouvons je trouve que ça n'a pas un rapport immédiat avec la question des données personnelles, puisque vous votre amendement vise à modifier les conditions de mutualisation de l'archivage des documents électroniques public qu'ils contiennent, tout le monde et données personnelles, je l'analyse comme un cavalier législatif j'émet donc un avis défavorable.

qui est pour. Qui s'abstient, il est adopté, nous passons à l'article 13 avec un amendement 12 rectifier Madame Delmont poulies et là vous. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'objet de cet amendement vise à circonscrire le traitement des données de santé par les organismes complémentaires aux seules fins de remboursement des soins, l'encadrement de la protection des données de santé souffrait jusqu'ici d'un relatif vide juridique aussi le législateur européen a tenu à les doter d'une définition précise à l'article 4 du RGPD nous savons tous que toutes les informations concernant un patient sont enregistrées puis stockées dans une base appelée Sunny IRAM chaque année pas moins de 1,2 milliard de feuilles de soins 500 millions d'actes médicaux et 11 millions de séjours hospitaliers y transitent, faisant de cette base un véritable Jackpot pour les organismes qui accéderont car c'est l'une des plus grandes bases médico-administratives au monde qui comprend en réalité 2 catégories de données, les données agrégées traité afin d'obtenir des informations anonymes, ces jeux de données sont rendus disponibles par l'assurance maladie, mais également les données à caractère personnel dites sensibles et nominative, quand on peut avoir accès à ces 2 types de données, même partiellement la faille du principe général d'anonymisation des données de santé réside dans le fait qu'on peut en croisant les informations ré-identifier une personne, or le texte que nous étudions aujourd'hui prévoit d'ouvrir aux organismes complémentaires privés un accès automatique aux données de santé à caractère personnel issu de la facturation des soins sans avoir à recueillir à chaque fois leur accord préalable, il existe déjà certains garde-fous dans notre droit qui nous protège des dérives qui pourraient découler d'un traitement des données par ces organismes et plus particulièrement sur les majorations, qui pourrait être appliquée sur les contrats en fonction de l'état de santé et des données de santé évolutive cependant l'amendement que je vous propose mes chers collègues, vise à renforcer ses garde-fous afin d'empêcher tout contournement de la loi par une interdiction explicite de fixation des prix des assurances ainsi que l'utilisation de ces données à des fins de choix thérapeutiques ou médical, oui, car il s'agit bien d'un risque d'une exploitation mercantile des données de santé éléments fondamentaux, clé de voûte de la protection de la vie privée, reconnue comme un principe fondamental du droit, c'est de cela dont il est question, rien de plus, rien de moins, notre système de protection sociale et précieux et rare, nous devons en prévenir les défaillances et non amortir sa chute, je vous remercie. Merci, avis de la commission Madame la rapporteure. Avis favorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Avis défavorable, monsieur le président, pour 2 raisons il nous semble qu'en 1er lieu cet amendement n'a pas sa place à l'alinéa 9 de l'article 13 qui vise uniquement à exclure certains traitements du Champ d'application du chapitre 9 de la loi qui est relatif donc au traitement mis en oeuvre aux fins d'assurer le service des prestations ou le contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que la prise en charge de prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire donc 1er Première Première éléments, il nous semble que cet amendement n'a pas sa place, les à 9 et en second lieu, il nous semble également qu'il existe déjà des garde-fous qui permettent d'éviter les risques invoqués quant au libre choix par le patient de son médecin et de ses choix thérapeutique médicaux des dispositions législatives du code de la santé du code de la Sécurité sociale protège ses droits des patients, je ne vous les cite pas, mais s'il y en a plusieurs, et s'agissant de la sélection des risques, il y a également d'autres dispositions qui permettent d'éviter ces dérives, je pense notamment à des dispositions des des assurances et de la Mutualité, notamment en matière de conditions d'exclusion et de modulation des cotisations encadrée donc pour ces raisons, j'émets un avis défavorable à l'amendement. Bien, donc il y a un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement Monsieur Savary. Oui, Madame la Ministre, moi je, je, j'ai cosigné cet amendement en tant que médecin, parce que je pense que véritablement, il va falloir aller plus loin dans ce qui, en ce qui concerne ce ce traitement des données personnelles, on peut retrouver, notamment pour des maladies particulières, par le biais du Smirat mot par le biais derrière de la part complémentaire qui est remboursé par la mutuelle ou pour par tout autre organisme assurantielle ou de prévoyance, on peut retrouver les malades, on le sait, ça a déjà été évoqué et on voit bien que les constructions de réseau qui amène derrière, peut-être sans vouloir préjuger de quoi que ce soit une Tina à Bakou peuvent se constituer autour d'un certain nombre de données et que derrière, selon le nombre de spécialistes médicaux, paramédicaux et d'ailleurs, que vous avez consulté, on peut retrouver des pathologies et dans certains cas identifié les personnes qui ont porté ces pathologies, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne prendra jamais suffisamment de précautions en ce qui concerne ces données-là parce qu'on sait très bien que derrière, ça peut être la porte ouverte à un certain nombre de dispositifs bancaire ou autres qui irait à l'encontre des intérêts du patient, donc je pense que véritablement on ne mettra jamais assez de garde-fous en ce qui concerne la production de ces données, notamment sur les choix thérapeutiques et médicaux, c'est la raison pour laquelle je voudrais remercier la Commission pour avoir donné un avis favorable, je pense que ce sera une Pierre supplémentaire pour une garantie le respect en tout cas de la confidentialité, en ce qui concerne les patients. Merci. On passe au vote. Donc je rappelle l'avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Cet amendement vise à intégrer dans la loi une obligation de langage clair facilement accessibles, lorsque l'administration s'adresse à un mineur âgé de 15 ans ou plus, il est essentiel qu'un mineur, choisissant d'échanger seul avec l'administration soit en mesure d'avoir un échange franc accessibles et compréhensibles. Cet abonnement qui lisent poser aux responsables de traitement de données de santé de dispenser dans un langage clair et facilement accessibles les informations données un mineur exerçant seul ses droits et satisfait le RGPD prévoit déjà de façon générale, d'informer de façon concise transparente, compréhensible et aisément accessible en des termes clairs et simples, les personnes exerçant leur droit, il craint en outre une obligation, c'est là où ça concerne le texte d'adapter toute information destinée spécifiquement à l'enfant. Bien, madame la Ministre votre avis. Même fiche souhaite le retrait ou elle n'favorable. Quand donc la commission et le gouvernement dit satisfait en demandant un retrait, vous dites quoi, monsieur. Bien, eu égard aux explications qui ont été demandé je retire amendement. Il est retiré ensuite amendement numéro 49. Messieurs de belles années Patriat c'est vous devez le nez. Oui, merci Monsieur le président, il s'agit d'une précision rédactionnelle puisque les conditions légales du consentement sont définies dans le règlement, comme dans la directive, comme la la manifestation de volonté spécifique éclairé et univoque et donc il conviendrait d'ajouter : article 42 après les mots, le consentement et qui est C'est une demande de retrait car les conditions de recueil du consentement sont déjà intégralement régit la manière générale et transversal par le règlement général pour la protection des données à l'article 7 et le règlement étant d'application directe, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il est non seulement inutile mais interdit d'introduire dans le droit national des dispositions redondantes divergentes. Madame la ministre, votre avis. c'est un avis favorable que je donne à cet amendement, puisque il me semble, pour être très bref, que le président le présent amendement qui rétablit le VISA de l'ensemble des conditions du consentement peut être soutenu, je crois que c'est une précision utile. Bien, donc il y a un avis défavorable de la commission, un avis favorable du gouvernement qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, il est rejeté amendement du gouvernement Madame la milice numéro 117. Mesdames et messieurs les sénateurs par cet amendement, le gouvernement propose d'instituer un comité de dite du système national des données de santé et CNDS qui est chargé de réaliser de faire réaliser des audits sur l'ensemble des systèmes portant sur des données qui sont issus du SNE DS ou bien qui composent le DS dans le respect des missions et des pouvoirs de la CNIL l'USN DS qui a été créé par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé regroupe, vous le savez, les principales bases de données de santé publique qui existe, le SNE DS vise donc à améliorer les connaissances sur la prise en charge médicale il leur gisement du Champ des recherches, des études et évaluations dans le domaine de la santé, les systèmes qui porte sur les données issues du SNE DS ou qui composent le SNS représente à ce jour près de 300 bases en l'état actuel de la législation, la seule autorité de contrôle de ses bases, c'est la CNIL au regard des enjeux de sécurité qui pèse sur ces données, l'objectif du présent amendement et donc de développer une politique d'audits piloté par l'État, en complément des pouvoirs de la CNIL, et notamment au en amont, permettant ainsi de sécuriser le processus de mise à disposition des données de santé : la mise en place d'une politique de dites propres au traitement réalisé avec des données du SNE DS participent, me semble-t-il directement de la crédibilité de l'ensemble du dispositif ces opérations d'audits ne sont que la juste contrepartie de l'ouverture de l'accès à des données sensibles, elles doivent permettre de garantir le bon usage et la sécurité de ces données, en vérifiant notamment que la réglementation est respectée que la finalité des traitements et conforme à ce qui a été annoncé et que le référentiel de sécurité est appliquée pour ce faire, dans le cadre de la gouvernance du SNE DS le comité stratégique données de santé a donc décidé la création d'un comité de dites pilotée par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères sociaux et qui est chargé d'établir un programme d'audits et d'en suivre l'exécution. Oui, madame la rapporteure votre avis. Le présent amendement crée un comité d'audit du système national des données de santé et autorisent en cas d'urgence, le directeur de la CNAM à suspendre temporairement l'accès au DS dans la mesure où les compétences et les prérogatives de la CNIL sont intégralement préservés le renforcement de la sécurité par ce dispositif me semble une très bonne chose, sur la forme, en revanche, vous me perdrez toutefois de regretter que le gouvernement ne découvrent cette excellente idée devant la 2ème assemblée saisie et au stade des amendements de séance simplement j'aurais aimé pouvoir solliciter l'avis de nos collègues de la commission des affaires sociales, mais ce sera évidemment une sagesse favorable. Bien donc sagesse favorable sur un amendement du gouvernement de la part de la Commission, oui Madame Goulet. Goulet. Explications de vote Monsieur le le président, Madame le ministre, moi je trouve que c'est, c'est un très bon amendement parce qu'un audit de plus chaque fois qu'on demande des rapports, on nous les refuse, c'est on va quand même pas refuser à un rapport et un audit proposé par le gouvernement, ce serait, ce serait quand même un peu, un peu malvenu, je voudrais vous poser une question : le ministre parce que l'intitulé et le et le thème même de votre amendement me fait penser à un amendement que j'avais déposée durant l'Plfss, qui concernait un auditeur, contrôle de l'INSEE, vous savez qu'on a à peu près un 1000000 800 1000 faux numéro digne c'est qui sont un sésame pays moi pour autant de prestations sociales et donc je voulais simplement Madame le ministre, vous, vous proposez d'avoir le même type de comité déontologique et le même type d'audits organisée par le gouvernement auprès de île c'est parce que c'est à peu près 40 milliards de fraude sociale et je pense que ce serait une excellente idée d'appliquer la même chose : c'est une, c'est une association d'idées que je fais en soutenant évidemment votre amendement 117 mais je pense qu'on aurait grand intérêt à multiplier ce type d'expérience pour d'autres bases de données et notamment lycée qui est la base de départ d'un certain nombre de prestations. Bien donc de un avis de sagesse positive qui est pour. Qui est contre qui s'abstient cet amendement du gouvernement est adopté un autre amendement du gouvernement, le numéro 93 Madame la Ministre. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, le gouvernement souhaite répondre à un besoin exprimé par les établissements de santé toujours dans leur pratique du codage et leur permettent d'avoir recours à des sociétés prestataires pour traiter les données, les données de santé nécessaires à la prise en charge des patients cet amendement fait suite à un courrier récent de la présidente de la CNIL à ma collègue Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé qui a soulevé un risque juridique, faute de base légale pour permettre à certains professionnels d'accéder aux données de santé des patients le codage est en effet nécessaire au financement de ces établissements par la tarification à l'activité, la fameuse T2A cette tarification impose à chaque établissement de santé concernés de rendre compte de son activité par une remontée de donner quantifier et standardiser relatives à la prise en charge des patients, c'est l'objet du programme de médicalisation des systèmes d'information PMSI, cet amendement vise donc d'une part à permettre aux établissements de santé, de faire appel en toute sécurité juridique au regard du secret médical, à des prestataires de codage des actes de soins dont les établissements ont réellement besoin et d'autre part à permettre aux commissaires aux comptes d'exercer pleinement leur mission en leur permettant de procéder à des vérifications sur un dossier individuel l'amendement proposé renvoie à un décret le soin de préciser les conditions réglementaires dans lesquelles s'est prêté prestataires extérieurs pourront accéder aux dossiers médicaux des patients, il permettra ainsi de sécuriser le recours à ces prestataires extérieurs pour le codage ou le dites des données PMSI en fixant un cadre juridique qui permet de garantir la protection des données de santé à caractère personnel des patients concernés. Merci l'avis de la commission Madame la rapporteur. Le présent amendement propose un dispositif qui facilitent et sécurisent le recours aux prestataires extérieurs pour les opérations de codage ou d'audit des établissements de santé, soumis à la tarification à l'activité, il s'agit d'un sujet très technique et l'a priori, nous y sommes favorables mais la présentation tardive de cet amendement en séance permet tout de même pas une expertise approfondie d'un sujet qui aurait bien mérité de consulter nos collègues de la commission des affaires sociales sagesse favorable. Bien sagesse favorable amendement du gouvernement qui est pour, ah pardon Monsieur Savary veut la parole. Oui, oui. Effectivement, je pense que c'est très particulier, c'est un sujet bien précis que ce clonage, on y travaille d'ailleurs à la commission des affaires sociales, dans un certain nombre de de domaines et ça montre bien qu'il y a des dispositions à prendre sur la protection des données, ça rejoint le l'amendement de le tout-à-l'heure auquel vous aviez donné un avis défavorable, madame la ministre, c'est dommage parce que véritablement il y a des enjeux derrière et en discuter avec ma collègue tout à l'heure, il y a par exemple le droit à l'oubli, pour lequel on s'est battus et qui restent encore pas forcément appliquer en ce qui concerne les personnes qui ont des pathologies et qui dit derrière quand ils veulent construire un projet, des difficultés pour avoir un prêt bancaire, ou en tout cas, quand ils en noir, ils ont une une un sur un intérêt qui est quand même parfois inacceptable puisque il y a bien entendu des guérisons et on ne doit pas porter toute sa vie, quand même, les séquelles d'un d'un accident intervenu à un certain moment, c'est la raison pour laquelle, moi je pense qu'il aurait fallu véritablement qu'il y a un avis, ça mérite une discussion approfondie de la commission des affaires sociales et je regrette effectivement que ce en tant que vice-président et d'ailleurs de la commission des affaires sociales, je regrette véritablement qu'il n'ait pas été discutée pour avis auprès de cette commission. Oui, Madame le Ministre. qui nous a alerté sur cette difficulté et cette lettre, nous l'avons reçu fin janvier 2018, c'est la raison pour laquelle, nous vous proposons cet amendement maintenant seulement, je ne méconnais pas évidemment les propositions que vous faites à cet égard. Monsieur le président, bas. Oui, je voudrais simplement présidé préciser à mon collègue Savary je voudrais préciser à mon collègue Savary, que nous avons proposé à la commission des affaires sociales, soit de lui déléguer cet article soit qu'elle s'en saisisse pour avis et c'est la commission des affaires sociales qui n'a pas souhaité le faire, je tenais à le dire souhaite, je souhaite naturellement que entre Commission, nous ayons les rapports de travail les plus coopératifs. Très bien, alors qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, nous allons passer au vote de l'article 13 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, je mais on voit aussi l'article 13 bis qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il est adopté. Nous arrivons à un article additionnel après l'article 13 bis avec un amendement à nouveau du gouvernement, le numéro 94 Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018 rond comme vous le savez puisque nous en parlons depuis hier avec la logique des formalités préalables les hypothèses dans lesquelles une autorisation préalable de la CNIL est requise, est requise, sont désormais résiduel est limitée aux traitements les plus sensibles, tels que les fichiers dits de souveraineté ou se comportant des données biométriques sous génétique dans un contexte qui est marqué notamment par des attentats très douloureux comme ceux commis par Mohamed Meira contre les militaires marquée également par un risque sécuritaire accrue, le ministère de la Défense a souhaité renforcer leur sécurité, en encadrant les conditions dans lesquelles les traitements de données à caractère personnel pouvait pouvait renseigner la qualité de militaire et certaines informations ayant trait à leur vie privée, le dispositif mis en oeuvre par l'article 117 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le Crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit ainsi un régime d'autorisation auprès de la CNIL pour mettre en oeuvre un fichier dont la finalité la finalité est fondée sur la qualité de militaire des personnes qui y figurent, ce dispositif prévoit également la réalisation d'une enquête administrative sur la personne responsable du traitement ainsi que sur toutes celles qui peuvent accéder aux données comportant la qualité de militaire, enfin des prescriptions techniques peuvent être imposées aux opérateurs privés concernés par le dispositif, telles que le renforcement de la sécurité des outils informatiques utilisés dans un souci d'allégement des formalités préalables et des sujétions imposées aux opérateurs privés, le présent amendement propose de refondre ce dispositif conformément à l'article 5 points du RGPD, le responsable d'un traitement ne pourra conserver la mention de la qualité de militaire des personnes dont les données sont traitées que si celle-ci est strictement nécessaire à l'une des filatures, des finalités du traitement, une campagne de sensibilisation des opérateurs privés sera à ce titre, réalisé par le ministère des Armées pour les traitements dont l'une des filles ladite et requiert absolument la mention de qualité de militaire, les responsables de traitement seront uniquement tenu d'informer le ministre compétent de leur mise en oeuvre et ils ne seront plus soumis à un régime d'autorisation ou de déclaration auprès de la CNIL en outre et à la différence du dispositif actuel, l'obligation d'information ne pèsera pas sur les collectivités territoriales et leurs regroupement pas davantage que sur les associations à but non lucratif, par ailleurs, le ministère des Armées pourra, le cas échéant, décidé de s'assurer de la sécurité des traitements en cause en procédant à une enquête administrative sur les personnes qui acceptent données personnelles des militaires, sans que cette enquête ne soit toutefois une obligation, ce projet d'article entend ainsi concilier l'impératif de sécurité des militaires qui a prévalu à la mise en oeuvre de ce dispositif et l'objectif d'allégement des obligations pesant sur les opérateurs privés. Merci l'avis de la commission madame la rapporteur. Cet amendement répond à un objectif parfaitement légitime qui vise à refondre le régime d'autorisation des fichiers mentionnant la qualité de mythe militaires pour être plus efficace, mais je me permet néanmoins de mettre en garde le gouvernement contre le risque des législations précipité cet amendement, qui est présenté par le gouvernement pour la première fois en séance publique dans la 2ème assemblée saisie vise à réécrire le cadre légal de ces fichiers, qui lui-même résulte d'un amendement déposé tardivement en séance publique lors de l'examen parlementaire au Sénat de la loi du 3 juin 2016, j'espère que cette fois, le régime a été davantage penser qu'en 2016 et qui ne présentera bien sûr pas tous les inconvénients que vous présentez pour présenter le précédent alors s'il est parfait, on va dire : avis favorable.

Merci Monsieur le Président Madame la présidente, madame la Ministre, cette intervention pour inciter mes collègues à vaincre le la réticence la répugnance même que provoque évidemment un amendement déposé aussi tardivement par le gouvernement et pour les inciter à voter pour en considération du fond et des enjeux pour les armées mais aussi pour les opérateurs privés, il s'agit de recalibrer un dispositif protecteurs de l'identité des militaires certes bien inspiré, mais ma foi mal dosé en l'état, c'est un marteau pilon pour écraser une mouche la DRS dès et le service de renseignement interne du ministère des Armées seraient obligés de faire 300000 le criblage par an, cela fait peser une charge disproportionnée également sur les acteurs économiques et sur la CNIL, le gouvernement propose de remplacer ce système par un autre mieux proportionnée qui restera crédible et efficace pour la protection des militaires, donc le maintien de la mention de militaires que si c'est indispensable, une enquête est possible mais non obligatoires, donc moi je pense qu'il faut voter pour cet amendement. oui Madame Boulet. le personnel pénitentiaire alors mais est ma question était la suivante est-ce que ce cette excellente disposition ne concerne que les militaires, est ce que vous avez l'intention de détendre ça aux gendarmes, aux policiers, peut-être que ce serait une une bonne idée, alors évidemment l'amendement n'a pas été sous-amendé mais vous avez un ensemble de forces de de police et de sécurité qui mériterait bien cette, cette mesure de protection voilà mais c'est un amendement que naturellement je soutiendrai. Bien à vif, pardon monsieur Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, bon c'est vrai que cet amendement présenté par Madame la Garde des Sceaux et bon, une explication aussi particulièrement importante pédagogique et c'est vrai qu'il complète les dix des dispositions au niveau du code de la défense, compte tenu, je dirais de l'objet de ce Tom Hand mon et surtout dans un contexte très particulier, très compliqué pour les militaires et, naturellement, la lutte contre le terrorisme et on associe aussi l'ensemble des forces de sécurité intérieure, police nationale Gendarmerie nationale militaire et seuls ceux aussi qui oeuvrent au quotidien pour la défense Des personnes et des biens en ajoutant aussi même l'est et les sapeurs-pompiers, c'est aussi un tout ce travail collectif là au niveau du col de la défense pour le ajout, bon j'irai aussi dans le sens de soutenir cet amendement du gouvernement, je dirais qu'il vise aussi à protéger aussi l'ensemble des forces de sécurité et les militaires, en particulier, je vous remercie. Merci donc avis favorable de la commission, un amendement du gouvernement qui est pour.

alors le 1er malgré plusieurs lignes de signataires n'ait pas soutenu, puisqu'aucun des signataires n'est dans l'hémicycle, donc on passe au 68 rectifier Madame Ben Basat. Monsieur le président, mes chers collègues, selon l'article 7 de la loi numéro 78 17 du 16 du 6 janvier 60 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement des données à caractère personnel pour être licite doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions énumérées par la loi, l'objet de notre amendement similaire à celui qui vient d'être défendus par nos collègues qui n'était pas là est alors de préciser la notion de consentement nous le plus long pour ce faire, les préconisations de la CNIL et du G29, groupe de travail Arctique 29 sur la protection des données, et propose donc que soit précisé dans la loi que le consentement est une démarche active de l'utilisateur explicite et de préférence écrite qui doit être libre spécifique à informer, cela implique notamment que son consentement ne soit pas exigé en contrepartie d'un bien ou d'un service merci. Merci avides de non on passe au 2ème rang en discussion commune Madame Carrère. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la question du consentement à la collecte de données personnelles est un sujet fondamental qui va probablement s'accroître avec la multiplication des utilisations faite de ces données une fois collectées jusqu'à présent, en effet, la méfiance de nos concitoyens, c'est essentiellement porté sur les fichiers constitués par les pouvoirs publics et notamment les fiches et les la prise de conscience de la valeur financière que représente la masse des données personnelles progressivement accumulées dans le secteur privé alimente des revendications destiné à permettre aux individus de monnayer la commercialisation de leurs données personnelles, cette revendication qui peut apparaître légitime remet ce matin cependant une question : le financement des sites internet gratuit qui se rémunèrent souvent par la publicité ciblée à partir des données personnelles collectées sur ces sites, où par ailleurs en quelque sorte les consommateurs de sites Internet sont déjà rémunérés pour le transfert de données personnelles par la consommation gratuite de service qui ont des coûts de maintenance et de main d'oeuvre ces sites souligne d'ailleurs souvent l'attachement des citoyens européens à la gratuité, il serait 80 nous paraît il nous apparaît important de réfléchir désappris à l'accompagnement vers un nouveau mode de financement des services consommateurs de données par ce qui soient plus respectueux de la notion juridique de consentement, aujourd'hui elle est réduite au rôle de simple formalité impérative pour l'accès à un service dans cette perspective, cet amendement vise à instaurer un vice du consentement, un cas de l'existence d'une exigence d'autorisation d'utilisation de ses données personnelles en contrepartie d'un bien ou d'un service à moins évidemment que le traitement faisant l'objet du consentement ne soit indispensable à la fourniture de ce bien ou de ce service. Merci à vie, madame la rapporteure sur ces 2 amendements. enfin les prix, les 6 2 amendements tant compléter la loi Informatique et libertés a en vue de préciser les conditions de validité de rucks de recueil du consentement, mais le nouveau règlement général de protection des données apportent désormais une définition très précise du consentement et détaille en outre au sein d'un article spécifique les conditions applicables à la validité de son recueil comme le rappelait encore récemment la Commission européenne dans une communication dédiée à l'entrée en vigueur du règlement selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il n'est pas seulement inutile mais bel et bien interdit de reproduire le contenu d'un règlement européen dans le droit national. Madame la Ministre, vos avis. Même avis, Monsieur le Président. Bien donc. Demande de retrait, que faites-vous madame Ben Basat Maryse Carrère, vous retirez Madame ben ça non, donc Madame Benbassa maintient son amendement qui est pour.

Après l'article 14 à un amendement de Madame Carrère le 38 rectifier. destinée à mieux protéger le consentement des personnes à l'utilisation de leurs données à des fins commerciales comme je viens de le dire, cette réflexion doit se mener de Pair avec celle sur le financement des services en ligne proposés aujourd'hui gratuitement en apparence, en l'occurrence, il s'agit d'imposer le recueil du consentement au moment d'une cession de données personnelles à des fins d'utilisation commerciale. Madame la rapporteure merci. Cet amendement introduit des concepts et des interdictions, qui ne sont pas ceux prévus par le règlement qui régit déjà précisément les conditions de traitement fondé sur le consentement et encadre de multiples garantit les aventures le retraitement ultérieur, respect des finalités exercice des droits, droits, sommes obligés de nous y tenir, demande de retrait. Bien demande de retrait, Madame la Ministre, même ma fille, monsieur le Président Madame Carrère vous retirer

Allez-y absolument ce président Madame la ministre, même le rapporteur, cet amendement est tout à fait particulier, sans revenir sur la décision de la commission de maintenir l'âge du consentement à 16 ans, cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de consentement conjoints prévus dans le RGPD, alors title 8, ce traitement n'est licite que si, dans la mesure où le consentement, les données autorisés par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, en effet, le RGPD est très floue en la matière : son article 8 disposant que le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier en pareil cas, que le consentement, les données autorisés par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponible que s'édifie la notion d'effort raisonnables: comment évaluer les moyens technologiquement disponible qui ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des entreprises au même moment la loi américaine la Loire Copa et paradoxalement beaucoup plus précises et protectrice en matière de consentement parental sans faire peser un fardeau normatif trop lourd Cholet responsable de traitement, la procédure de consentement conjoint devraient

de la Commission nationale de l'informatique et des libertés devra préciser les conditions dans lesquelles s'exerce ce consentement conjoint information à communiquer procédures à suivre pour obtenir l'effacement des données et enfin il prévoit que le responsable de traitement efface l'ensemble des données personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint s'il le dit consentement n'est pas donné dans un délai de 15 jours les données personnelles à la fois des parents et des mineurs pourront être recueillis lors de cette procédure que l'entreprise d'aucune raison de conserver si ce consentement n'est pas, il fit les données. La vie de la commission Madame la rapporteur. Cet amendement est en partie satisfait par le règlement, dont je rappelle qu'il fixe par défaut, l'âge de consentement des mineurs à 16 ans, et il n'est donc interdit par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union peine de recopier ces dispositions dans le droit national, je vous demanderai Madame la ministre. On est bien d'accord, c'est sur les 3 amendements, Oui, monsieur le président, c'est un avis défavorable que jamais cet amendement comme l'a dit Madame la rapporteure, la marge de manoeuvre de l'article 8 points du règlement permet aux États-membres savons prévoir par la loi un âge inférieur etc ne permet cependant pas de préciser les conditions de recueil de ce consentement, comme le précise l'objet de cet amendement, l'obligation présente à l'article 8,2 et celle d'un effort raisonnable, ce qui implique une obligation de moyens, précisée par un décret comme cela est suggéré les conditions applicables à ce consentement pourrait pourrait remettre en cause plusieurs objectifs du règlement de 2016 et notamment la question de l'harmonisation et de la responsabilisation par ailleurs le décret en Conseil d'État n'apparaît pas être l'outil le plus adapté, les services de la société de l'information concerne évoluent très rapidement, alors que l'outil proposé reste relativement rigides et ce, alors même que les autorités de protection données qui sont réunis au sein du G29, ont précisé les conditions ne se concentrant dans un avis récent qui plus évolutif, une nouvelle version de cet avis devrait d'ailleurs être publiée prochainement à la suite de la consultation publique a été menée par ses autorités, par ailleurs, l'amendement proposant l'effacement des données à caractère personnel si le consentement n'est pas donné dans un délai de 15 jours, il me semble que ce délai n'apparaît pas souhaitable en effet si par exemple le consentement n'est pas autorisé, il n'y a aucune utilité à conserver les données plus longtemps que nécessaire et en ce sens, le G29 rappelle l'application de l'article 5,1 avec ce principe de mutualisation des données dans le cas de la mise en oeuvre du RGPD pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable. Donc c'est avis défavorable sur les 3. Donc : demande de retrait sur les trois par Madame la rapporteure et avis défavorable de Madame la Ministre.

de créer un droit de la propriété intellectuelle sur les écrits publics en ligne sur un blog sur un réseau social média d'expression moderne, il convient de reconnaître que le Net et les réseaux sociaux sont aujourd'hui un foyer de création artistique et intellectuelle, cet amendement entend reconnaître cette création numérique est accordé aux citoyens un droit d'exploitation des données numériques au-delà de la création de données personnelles cet amendement crée un droit moral sur les données non coordonnées historique de l'obligation légale à ses héritiers ou à des tiers, afin d'encourager une gestion prudente des données personnelles, il est en effet pas normal que ces données soient aujourd'hui exploité sans vergogne, alors que la grande majorité des utilisateurs n'a pas connaissance de ces bases de données produites et abandonnée à des opérateurs extérieurs. Merci à vie de madame la rapporteure. Oui, le droit de la propriété intellectuelle qui attache des droits patrimoniaux et moraux créations originales de l'esprit ne paraît pas être l'outil adapté à pour régir justement les les données personnelles et j'ai aussi un doute sur le caractère normatif de de de cette proclamation, c'est un avis de retrait. Donc, retrait, Madame la Ministre. Monsieur le président, Monsieur le Sénateur, le gouvernement est défavorable, comme à l'Assemblée nationale, d'ailleurs à cet amendement qui a pour effet de conduire à une patrimoniale à une patrimonial il importe de rappeler, je crois que le droit d'auteur et le droit moral qui lui est attachée, ne s'applique qu'aux Oeuvres de l'esprit, notamment aux livres auto-visuel ou sculptures turque créée par les auteurs de simples données personnelles qui ne résulte donc pas d'un acte de création non, me semble-t-il, pas vocation à être protégé par le droit d'auteur, l'extension du droit d'auteur aux données personnelles l'insertion des données personnelles dans le Champ de protection du droit d'auteur aurait en effet pour conséquence de consacrer au profit des personnes concernées, un véritable monopole d'exploitation sur ces données qui interfèrent avec le cadre fixé par la loi de 1978 donc, de façon générale la la patrimonial disent Sion des données personnelles constituent bien sûr un sujet extrêmement complexe qui n'est pas tranchée complètement aujourd'hui en l'état du droit, il n'existe pas de droit de propriété de l'individu sur ses données personnelles et le le RGPD ne l'a d'ailleurs pas consacré au niveau européen des réflexions très approfondies ont déjà été conduites sur ce sujet, et notamment le Conseil d'État, il a consacré une analyse extrêmement intéressante et approfondie dans son étude annuelle de 2014 sur le numérique et les droits fondamentaux, il a jugé préférable d'écarter la reconnaissance d'un droit de propriété de l'individu sur ces données et consacré à la place un droit à je le cite : l'autodétermination informationnelle qui est entendu comme la liberté de l'individu, de décider comment ces données personnelles peuvent être utilisés, ce droit a d'ailleurs été développé par la cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui a consacré un tels concepts en 1983 tendance, je cite la cour à garantir en principe la capacité de l'individu, a décidé de la communication et de l'utilisation de ces données à caractère personnel cette conception a été reprise au niveau national dans la loi pour une République numérique et il n'est aujourd'hui pas envisager d'aller plus loin, pas dans le cas du présent projet de loi, je sais que certains considèrent que reconnaître un droit de propriété sur ces données seraient plus favorables aux citoyens car il permettrait de mieux les associer à la création des richesses produites par l'exploitation de leurs données personnelles, il s'agirait également d'accompagner peut-être une réalité qui est que nos données, nous le savons, sont déjà obligés de commerce mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent avant de s'engager sur cette voie, comme l'a rappelé le Conseil d'État une untel rééquilibrage serait largement illusoire, comment fixer le prix d'une donnée alors que ce sont souvent les croisements de très grandes bases de données qui leur confère de la valeur en permettant par exemple de créer des ciblage publicitaire très précis : comment assurer le respect d'telle droit à l'échelle européenne ou internationale comment articuler ce droit avec les restrictions au droit, protection des données, etc, il existe déjà un certain nombre de normes qui protège l'individu contre une exploitation abusive de leurs données personnelles, l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement européen et la directive que nous transpose 11 aujourd'hui dans le présent projet de loi ainsi que diverses législations sectorielles propres par exemple à la protection des bases de données en matière de droits de la propriété intellectuelle permettent de converger sur ce point de vue, il me paraît donc plus sage de de conserver ce cadre juridique plutôt que de s'engager sur la voie d'une patrimonial disent Sion des données personnelles. Oui, Monsieur le Président, naturellement, cela ne me satisfait pas totalement mais les explications qui m'ont été donnés l'invite à retirer cet amendement. Très bien. Il est retiré, donc on vote sur l'article 14 inquiets pour. Qui est compte qui s'abstient. article 14 amendement numéro 95 du gouvernement. Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mesdames et messieurs, c'est tellement de m'95 vise à maintenir dans sa rédaction actuelle alinéa 1er de l'article 10 de la loi dite CNIL matériellement le Champ de la rédaction issue de la commission et celui du droit actuel, nous le considérons comme identiques et nous sommes préférable de s'en tenir plutôt au droit en vigueur qu'il y a au moins 2 avantages, le 1er c'est que c'est le droit actuellement pratiqués est connu, et le 2ème, c'est qu'il est plus explicite que la proposition de l'votre rédaction parce qu'il ne procède pas un renvoi au règlement et vise directement les traitement automatisé de données à caractère personnel prohibé, c'est-à-dire pour les rappeler les traitements destinés à évaluer certains aspects de sa Pernel considérant que le droit actuel est plus performant aujourd'hui que la par opposition que vous seriez amené à faire. Bien, madame la rapporteure votre avis. Il nous semblait qu'que la définition à la commission était plus complète puisque, à la place de une appréciation sur le comportement d'une personne vous renvoyons justement au profilage à la définition du profilage qui consiste à partir de faits passés relatifs à une personne évalue la probabilité de faits passés, présents ou futurs, la concernant, qu'elle est comme une infraction bon sagesse. Bien avis de sagesse de la commission avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui s'abstient, Qui s'abstient, il est adopté. 2 amendements en discussion commune 1er du gouvernement numéro 96 Madame la Ministre. monsieur le président. Madame le rapporteur alors en préambule, le gouvernement se doit de noter la convergence de vues sur le fond avec Madame le rapporteur, vous avez écrit dans votre rapport, on ne saurait admettre que l'administration se défausse de ses responsabilités sur la machine en jouant de la complexité technique et et de la réputation d'infaillibilité des automates pour masquer ses propres choix, hé bien je partage tout à fait cette analyse, c'est bien cela qui fait du tort en définitive à la dématérialisation et à la modernisation de nos modes d'action qui la caricature malheureusement si cette convergence visible dans votre rapport semble cette cette convergence qui était visible dans l'analyse du rapport semble s'être perdu dans le texte, finalement adopté par la commission des lois qui nous semblent obscurcir et limiter considérablement le Champ d'application et sur lequel il se doit donc de revenir le présent amendement il rétablit globalement le texte dans sa version issue de l'Assemblée nationale l'équilibre qui avait été trouvé, il s'agissait de réellement permettre le recours à des décisions administratives prises sur le fondement d'un traitement algorithmique, tout en offrant les garanties nécessaires pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes des usagers concernés en 1er lieu il est important que figure explicitement dans le texte de la loi Informatique et Libertés, les garanties prévues, permettez-moi de revenir dessus, sur ces trois transparence intervention humaine et maîtrise. Transparence, l'usager est informer systématiquement lorsqu'une décision est prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, il peut demander des informations supplémentaires, très détaillé, deuxièmement, il s'agit de l'intervention humaine à travers le droit de recours qui est permis déjà aujourd'hui et enfin de la maîtrise du traitement et cette garantie, elle doit être explicitée et la CNIL il a particulièrement insisté sur ce point dans son avis, le lien entre la maîtrise et la transparence à travers l'explique habilité du traitement et on en reviendra, on y reviendra plus tard sur plusieurs amendements est important pour l'économie globale du dispositif, à notre sens, l'obligation de maîtrise constitue une intervention humaine à priori dans le cas de l'élaboration du traitement algorithmique lui-même, c'est donc la garantie que propose le gouvernement, contre le risque lié à l'essor de l'Intelligence artificielle et des algorithmes, que l'on appelle auto-apprenants et des traitements dits de boîtes noires, alors le gouvernement vous propose d'affirmer ses garanties qui sont selon nous suffisante, plutôt que de restreindre draps strict drastiquement le Champ d'application de ces usages. Oui, madame la rapporteure votre avis. La commission des lois a estimé que les garanties apportées par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les décisions prises par l'administration sur le fondement d'allégories tu n'étaient pas suffisantes, sans méconnaître les bénéfices liés à l'usage d'algorithme par l'administration, la Commission a voulu se prémunir d'un triple risque hein, une décision automatisée risquent d'être aveugle à des circonstances de l'espèce qui mériteraient d'être prises en compte, parce que l'algorithme n'a pas été programmé pour le faire, le recours aux algorithmes donc être réservé à des cas qui n'appellent aucun pouvoir d'appréciation : le 2ème risque lié à l'essor de l'Intelligence artificielle et que des décisions administratives individuelles soient prises, sans que personne ne sache suivant quels critères l'algorithme ayant déterminé lui-même les critères à appliquer leur pondération, c'est ce qu'on appelle le phénomène des boîtes noires, le 3ème risque que la programmation des algorithmes destiné à prendre des décisions individuelles n'aboutissent à contourner les règles de fond et de forme qui encadre l'exercice du pouvoir réglementaire ainsi dans la procédure, dite Admission post-bac, les candidatures des lycéens dans les licences universitaires étaient classés suivant des critères reposant sur une base légale fragile qui n'avait jamais été explicité dans un texte réglementaire et qui n'est même n'était même pas rendu public, on ne saurait admettent que l'administration se défausse, c'est ce que vous disiez en répétant les arguments de la commission se défausse ainsi de ses responsabilités sur la machine, un jour, la complicité technique et la réputation d'infaillibilité des automates pour masquer ses propres choix, la commission des lois a donc choisi de n'autoriser les décisions administratives individuelles prises sur le fondement d'un traitement automatisé de données personnelles que lorsque ce traitement a pour objet d'appliquer strictement les dispositions légales ou réglementaires à des faits dans la matérialité la qualification juridique ont été établies sur un autre fondement qu'un traitement automatisé, cela rend inutile la précision apportée par l'assemblée, selon laquelle le responsable de traitement s'assure de la maîtrise du traitement algorithmique et ses évolutions afin de pouvoir expliquer d'État et sous une forme intelligible à la personne concernée, la manière dont le traitement a été mis en oeuvre à son égard : pourquoi, d'une part parce que l'algorithme ne pourra pas évoluer, ce ne sera pas une boîte noire et il se rapproche la pour appliquer strictement le droit, c'est une de nos exigences principales d'autre part parce que le code des relations entre le public et l'administration garantit déjà tout la possibilité de se voir communiquer les règles et les principales caractéristiques de mise en oeuvre d'un algorithme lorsque celui-ci a servi à prendre une décision à son égard, nous retrouvons ce problème je crois dans les amendements à venir enfin contrairement à ce qu'indique l'objet de l'amendement gouvernemental, il paraît tout à fait nécessaire d'inscrire dans la loi que la Gorrite doit avoir pour objet d'appliquer strictement les dispositions légales du réglementaire, il existe en effet toutes sortes de décisions administratives individuelles dont le sens n'est pas déterminé par le cadre législatif ou réglementaire, ce sont les décisions pour lesquels l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation, or nous refusons absolument que de telles décisions soient prises sur le fondement d'un algorithme, ce qui reviendrait d'ailleurs pour l'administration à renoncer à son pouvoir d'appréciation au cas par cas.

Qui est contre. Qui sapiens il est rejeté un amendement dit d'ailleurs c'était en discussion commune mais comme on a fait le vote différemment, on continue, amendement 138 de madame Sylvie Robert. je, je vais aller vite puisque cet amendement reprend en partie et les garanties apportées par le paragraphe 3 de l'article 22 du règlement en matière de protection des droits et des libertés, de l'individu et notre amendes prévoir que dans le cadre des décisions administratives individuelles prises sur le fondement d'un algorithme, l'intéressé puisse exprimer son point de vue et surtout contesté la décision qui en résultent, en fait c'est un renforcement du droit recours je voudrais en profiter, monsieur le président, rapidement, puisque nous sommes sur un article, je voudrais féliciter la rapporteur pour la réécriture de ce de de cet article qui, de mon point de vue apporte beaucoup plus de garanties en la matière, la question des des algorithmes, on le sait, soulève et de plus en plus, de nombreuses questions aujourd'hui et et et je ne souhaitais pas même si on pourra y revenir que elle soit évacuée comme cela,

puisque Parcoursup est quand même un algorithme, d'ailleurs, il se compose de 2 algorithmes central et un appareil un appariement avec des algorithmes locaux et je pense qu'on peut avoir un débat sur cette question à la fois de transparence et et du coup d'incidence sur à la fois cet appariement et je dirais l'opacité qui qui règne autour de cet algorithme jouera terminait par dire que on on se souvient, puisqu'on parle de 2 cas concrets de la question d'APB, ce qui avait fait défaut dans APB c'était justement que l'opacité, ne permettait plus la confiance et je crois que cette question de confiance est extrêmement importante, quand on parle d'algorithmes et et je trouve que, en tout cas la réécriture que vous avez fait madame rapporteur de Séraphin de cet article 14 qu'on essaie d'améliorer et sur lesquels nous allons apporter des amendements et fort bien aujourd'hui. Merci donc avis de la Commission sur cet amendement Santropol. Eh bien. Avis favorable de la commission et. Le gouvernement dit quoi, monsieur le Ministre. Encore une fois, si le gouvernement partage bien sûr l'objectif de cet amendement et je le répète, qui est de s'assurer que la personne concernée par la décision puisse faire valoir son point de vue et bénéficie d'un plein droit de recours et vous avez rappelé votre regard général cet article 14 que nous partageons aussi sur la nécessité la plus absolue de transparence et le gouvernement est défavorable à votre amendement car nous pensons que les autres mesures permettent d'appliquer toute l'ambition par ailleurs.

notre Haute assemblée avait considéré que les algorithmes le co-devait être dissociée de la décision prise par l'administration, la ministre s'était engagée sur ce principe, nous avait donné des garanties et on s'est aperçu que dans les décrets, une autre voie réglementaire a été a été prise, qui considèrent que le résultat de l'algorithme est partie prenante de la décision du jury qui est couvert par le secret des délibérations, ce qui en droit n'est pas recevable puisqu'il s'agit réellement d'un traitement automatisé qui est préalable au débat de des enseignants sur sur les dossiers, donc l'article 14, telle que il est proposé aujourd'hui vient combler un vide juridique, de façon tout à fait pertinente je le soutiendrais volontiers. Bien donc nous passons au vote, il a un avis favorable de la commission, un avis défavorable. Du gouvernement Madame Morin-Desailly pour explication de vote. Oui, je voulais juste apporter un complément d'information à notre débat puisque, on évoque la loi orientation résulte des étudiants que nous avons voté il y a quelques semaines ici dans l'hémicycle, je me fais un petit peu aussi le porte-parole du rapporteur Jacques Grosperrin avec lequel on a, on a discuté ces derniers jours sur ces questions de transparence des algorithmes, il est vrai qu'au moment des débats, ce dernier était très sensible à l'idée de la publication des algorithmes locaux pour que en effet on ne retourne pas dans un système de de boîtes noires telles que APB avait fini par être appréhendé, dans le dispositif APP, on avait l'impression que toute décision humaine d'ailleurs avait totalement disparu et que finalement on s'en remettait complètement au résultat produit pour la machine, bon je crois que l'état d'esprit de la loi Orientation et réussite des étudiants n'est pas n'est pour dire honnêtement les choses débattu de l'idée que, comment dirais-je, les inscriptions se faisait bien sûr de manière automatisée avec un certain nombre de de critères voilà qui sont établis, mais que le résultat, c'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec notre collègue Ouzoulias, le résultat ne devait être qu'une aide qu'une aide et non pas conditionné totalement et directement et inéluctablement la la décision je rappelle quand même que que il y a un comité pédagogique qui doit quand même examiné les choses et je rappellerai aussi que le Sénat a voulu dans dans sa sagesse instauré bien sûr un comité déontologique qui puisse bien entendu être garant un comité éthique et scientifique, plus précisément, qui a vocation à prévenir tout risque lié à de, de, de, de, de transparence, mais ce que je veux dire à c'est complètement, c'est que la part humaine dans le cas des décisions qui sont prises dans un cadre pédagogique, le secret des délibérations aussi d'une instance qui se réunit et tout à fait légitime, donc je souscris tout à fait au travail fait par Madame Joissains qui est un excellent travail et qui justement pose les conditions que nous-mêmes, nous avions établi apporter ce type de précision et dire aussi que le le texte a été voté à l'époque, en l'état, avec cet amendement du gouvernement, on est aussi dans une année de transition où les universités vont expérimenter, en quelque sorte le le le dispositif qu'il faudra être attentif aussi aux remontées qui vont venir du terrain pour ajuster au mieux le processus d'orientation des élèves vers leur parcours de de de réussite que ils sont là dans une phase où ils vont rentrer dans la phase où ils terminent leur vie entre le 15 et le et le transport, terme 30 mars donc, le processus est enclenché, donc je me demande madame le rapporteur si la disposition proposée, qui est un renforcement de de cette obligation de transparence, ce qui est tout à fait légitime mériterait pas d'être appliquée voilà, à partir du moment où le processus est déjà pour cette année, en tout cas, terminé. Bien, il y a un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour. qui est contre qui s'abstient c'est un amendement 138 adopté. Donc, nous passons à 2 amendements identiques le 97 du gouvernement. Monsieur le président, madame la rapporteure avant d'aborder le l'amendement 97, je voudrais simplement que l'on est tous en tête l'idée que nous allons bien discuter de ce sujet de l'application de la loi Where dans le cas de l'amendement 99 sur lequel je prendrai le temps temps d'expliciter la position du gouvernement de la détailler de vous rassurer sur le nombre des éléments parce que sur ce sujet, nous partageons et la même ambition et je crois que je serais de jusqu'en mesure de vous apporter de nombreuses informations actualisées alors sur l'amendement 97 je voudrais aussi en profiter pour faire un un petit commentaire plus général sur l'utilisation des Data Science de sciences de la donner au son administration dans le cas de la modernisation de l'action publique, nous souhaitons que les datations se répandre dans l'administration française et que les opérations d'enquête ou de contrôle puisse s'appuyer plus souvent sur des analyses de données à la fois pour optimiser l'activité des services d'enquête dont les ressources notamment humaines sont toujours trop limité mais les traitements sur lesquels ils peuvent s'appuyer doivent demeurer exactement cela, des outils d'aide à la décision, rien de plus, rien de moins, c'est bien cette situation qui prévaut aujourd'hui dans l'appareil d'État, des outils d'aide à la décision basé sur les sciences de la donner, y compris au sein de l'administration fiscale. En outre, cet alinéa, il nous sommes contraires au règlement puisque dans c'est le cas de cette année n'a aucune garantie n'est prévu pour que ces actes alors qu'ils affectent significativement les personnes ne sont pas ne ne reçoivent aucune garantie si je sur ces garanties, il y a d'abord le droit au recours à faire valoir son point de vue qui n'existe pas dans le cas telle qu'il est rapporté dans cette écriture mais il n'y a pas non plus dans ce cas de mention dans l'acte alertant la personne sur le recours un algorithme pour ces raisons, nous proposons, c'est un nom. Bien amendement présenté par Monsieur Durand identique, il est défendu et donc avis de la Commission sur ces 2 amendements identiques. Un simple acte d'enquête ou de contrôle peut-être intrusif, même si la Commission l'avait décidé différemment la réflexion sur les algorithmes et vraiment loin d'être abouti, nous ne savons pas encore très clairement dans quelle mesure nous pouvons nous y fiez quel biais, ils peuvent comporter quel discrimination et peuvent engendrer, quelle est la bonne manière de les contrôler, raison pour laquelle nous avons pris certaines mesures que nous détaillons peu à peu, il serait bon d'ailleurs que le gouvernement ne fasse part de son appréciation sur l'idée de créer une commission consultative, voire une autorité administrative spécialement chargé du contrôle des algorithmes. Attendons d'y voir plus clair, je pense qu'il convient de faire preuve de prudence et à titre personnel, de l'avis favorable à ces amendements. Bien, donc avis favorable aux amendements du gouvernement et de Monsieur Durand qui sont identiques, qui est pour.

Nous allons à présent passer à 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune d'abord le 98, soutenu par le gouvernement, monsieur le Ministre. Monsieur le président, Mesdames, le rapporteur monsieur le président de la commission des lois, mesdames et messieurs les sénateurs, alors cet amendement 98 qui vise à supprimer la 8 de l'Arctique, qui prévoit la nuit la nullité des décisions administratives individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique ne comprenant pas la mention d'information de l'usager mentions obligatoires si le gouvernement partage pleinement, et je le répète encore une fois, je le répète très souvent pleinement l'objectif de faire appliquer l'article L 311 3 1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'est pas favorable à ce que l'absence de mention dans la décision conduise immédiatement à la nullité de cette dernière, ce qui serait, selon nous, complètement disproportionnée et nous sommes d'une part que ce de point doit être laissée à l'appréciation du juge administratif avec l'application de la jurisprudence d'Anthony en la matière qui n'est pas univoque, il note d'autre part qu'il n'existe pas de précédent de ce type en matière d'obligation d'Editis qu'en effet aujourd'hui l'autre mention obligatoire dans les décisions administratives concernant la mention des voix et délais de recours de la décision, l'absence de C. mention n'entraîne pas la nullité des décisions mais la simple non oppose habilité des délais de recours, la décision, elle reste valide. Concrètement que signifierait la nullité de la décision, dans des cas très pratique pour les Français, si je reçois mon avis d'imposition, sans mention et ce que je peux refuser de payer l'impôt si je reçois la décision que je peux recevoir le RSA sans mention quelles en seraient les conséquences, alors je veux le redire, simplement pour que la position du gouvernement soit très simple, la mention, elle est bien obligatoire, le droit existantes dans le droit existant et nous la ferons respecter et nous la faisons respecter. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, je Monsieur le Ministre, mes chers collègues, que nous avons tous conscience dégaine administratif a tirer de l'utilisation des nouveaux outils technologiques comme les algorithmes lors de l'examen de la loi pour une République numérique, le groupe RDSE avait cependant déjà pointé les limites de l'utilisation d'algorithmes pour la transparence des décisions individuelles prises sur ce fondement, mes collègues avait alors proposé et obtenu que les caractéristiques de ces algorithmes puissent être communiquées aux personnes intéressées qui en faisaient la demande, comme l'a souligné l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, c'est moins le logiciel d'admission post-bac que les dispositions juridiques et les choix politiques sur le fondement desquels il a été programmé qui ont conduit au bug largement commentée, beaucoup considèrent que la résistance des ministères, a communiqué les codes sources de tels algorithme contribue à accroître les suspicions qui existe à leur encontre en cas de généralisation de traitement automatisé similaire, il est à craindre que les fondements effectif les décisions administratives deviennent moins accessible et moins intelligible si ses codes sources ne sont pas communiqués, c'est pourquoi nous souhaitons que ces caractéristiques techniques soient systématiquement publiés afin que chacun puisse prendre connaissance des critères effectivement retenu lobes l'élaboration de telles décisions individuelles dès lors que ces algorithmes n'ont pas vocation à se substituer totalement l'appréciation des agents administratifs chargés de préparer les décisions concernés, il n'y a pas de raison vous de vouloir s'opposer à leur libre communication a l'air de la transparence, il serait invraisemblable de pouvoir maintenir de l'opacité sur ces questions. Merci monsieur le président, il s'inscrit dans le droit fil de ce qui vient d'être présentée par notre collègue Carrère, l'article 311 tiré 3 attiré 1 du code des relations dans le public, administration dans sa rédaction actuelle prévoit que les informations concernant le fonctionnement de l'algorithme sont communiquées l'par l'administration à l'intéressé, s'il en fait la demande, nous proposons d'inverser le principe dès lors que les algorithmes sont partout qu'ils seront encore plus présents dans les années à venir, que la transmission à l'intéressé soit systématique et que l'intéressé n'est plus à en faire la demande, donc c'est l'objet de cet amendement, qui permettrait d'assurer l'information des administrés sur le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, de communiquer, elle assure l'administrer la nature des données traitées leurs sources, les paramètres de traitement éventuellement leur pondération les conditions d'application de de de cet article sera fixé par décret en Conseil d'État. Merci, cher collègue, je vais demander l'avis de la commission pour cette série d'amendements.

de déclarer des droits si le citoyen n'en est pas informé et si finalement ces droits-là restent lettre morte, la loi pour une République numérique qui est qui a été promulguée en octobre 2016 a prévu que les décisions individuelles fondées sur un traitement algorithmique devrait comporter une mention en ce sens. L'administration doit appliquer la loi, tout simplement, alors après bon juge peut vous parler de la jurisprudence Anthony mais au-delà de ça, dans la pratique, puisque vous y faisiez allusion dans la pratique ça ça nécessitera simplement de renvoyer la même décision, le même courrier avec la mention que ce que cela occasionnera je pense que c'est pas forcément plus mal de temps à autre, pour que les pratiques se mettent en place, pas de sonner, un petit peu l'alarme tout simplement ensuite concernant l'amendement de de Madame Carrère, je dirais que la proposition est satisfaite, mais je dirais sagesse sagesse pour ma part, je voterai pour. Idem du reste, pour l'amendement numéro 134 rectifier. Merci madame le rapporteur, quel est l'avis du gouvernement pour 145 et 134 rectifier. Monsieur le Président Madame la rapporteure insulter certains je voulais entrer d'abord sur le 134 rectifier le gouvernement est défavorable à cet amendement il a déjà eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale, mais permettez-moi de exposés puisque ça a été l'objet de nombreuses discussions depuis tout à l'heure à nouveau l'équilibre que nous avions trouvé en matière d'information sur les algorithmes et cet équilibre telle qu'il avait été trouvé, il me semble bon d'abord les administrations sont et vous avez rappelé, texte qui a permis son tout d'abord soumise à une obligation générale de publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmique utilisés dans l'accomplissement de leur mission lorsqu'ils font des décisions individuelles, c'est donc un 1er niveau d'information à priori pour tous les usagers et à tout moment et ce sera une obligation généralisée à compter d'octobre 2 1000 18 premières étape 2ème il y a ensuite une information systématique de chaque intéressé concernés en cas de décision, la personne est informé à chaque fois de la mise en eau du traitement algorithmique par une mission d'une mention bien visible dans la décision, vous venez de l'Euro défendent je rappelle cette obligation-là l'élément sur lequel nous nous opposons, c'est celui de la conséquence de l'absence de cette mention, mais cette mention est obligatoire et solidaire d'une indications qui est en charge de le faire respecter, et donc c'est le cas, ce sera de plus en plus le cas et celles qui n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui le feront de plus en plus la nullité ne peut pas être une sanction la nullité une sanction que nous considérons comme étant non proportionnel. Cette mention, elle va et elle fait déjà, elle précise la finalité poursuivie par l'algorithme et elle rappelle le droit de la personne d'obtenir communication des règles du traitement et de leur application dans son cas particulier, ainsi que sur les modalités d'exercice de son droit à la communication et à la saisie 3ème étape si la personne en fait la demande, elle obtient donc beaucoup plus information ces informations qui sont précisés au niveau réglementaire, elles sont au nombre de 4 : le le degré le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, de les données traitées et leurs sources, ainsi que les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondérations appliquées à la situation de l'intéressé et quatrièmement les opérations qui ont été effectués par le traitement cette information là elle est individualisé, elle est très détaillé, elle comprend l'intégralité des données ayant servi à faire fonctionner l'algorithme toutes ces caractéristiques, c'est ça qui fait l'intérêt du dispositif mais elles en font également pour l'instant, un dispositif qui n'est pas automatiser able ou généralisable et qui exigent un traitement au cas par cas, donc une charge réelle pour les services aujourd'hui, ce sont bien des être s'humains, des agents publics qu'ils prennent le temps de faire ses réponses personnalisées en réunissant toutes ces informations, alors s'il fallait prévoir une information systématique des personnes comme le propose cet amendement, il faudrait mettre en place un mécanisme automatisé et donc la conséquence, ce serait de dégrader le niveau d'information qui serait donnée, alors il me semble qu'il y a aujourd'hui un bon équilibre entre des vecteurs d'information systématique et la possibilité d'obtenir sur demande des informations beaucoup plus détaillé par exemple, lorsque la décision est défavorable, dans ce cas, je veux en savoir plus, ou en cas de questionnement sur les motivations, la garantie de transparence doit notamment se lire en lien avec les garanties liées au recours prévues par le règlement dans le considérant 71, enfin, je veux revenir sur le code source le code source des des algorithmes ayant des conséquences sociales, sanitaires ou économiques sera également mis à la disposition du public, ce qui permettra une complet trop de validité de l'Administration puisque des personnes pour et de la personne de la société, expert de la société civile pour l'analyser en détail voir rejouer des signes de situations rejouer des scénarios et vérifier que la procédure s'est correctement déroulé concernant l'amendement 145. Dans la continuité du 134 je voudrais revenir sur quelques éléments sur la question de la nullité en cas d'absence de mention, nous en avons parlé mais s'agissant du reste de l'amendement, il est déjà très largement, voire complètement satisfait par le droit, en vertu de l'article L 312 3 du code des relations entre public et l'administration, les administrations devront et je l'ai rappelé dans les différents grades devront a pu compter d'octobre 2018 publiée en ligne accessible au grand public, toutes les règles définissant les principaux traitements algorithmique utilisé pour toutes ces raisons, le gouvernement est défavorable.

votre analyse, je crois qu'il satisfait une des car une des interrogations que nous avons évoqués à l'instant, reprenons l'exemple de ce qui se passe avec la loi Orientation et réussite des étudiants y à Parcoursup qui est soumis au contrôle que vous avez indiqué les dossiers arrivent dans les universités, ils sont traités par des algorithmes locaux qui permettent un pré-tri automatisé, ensuite ils sont transmis au jury qui décide sur un examen pédagogique des dossiers la Reuss, il la recevabilité du dossier, j'aimerais savoir, je crois que vous avez répondu favorablement, si les algorithmes mis au point par les universités pour faire le tri des dossiers qui leur écrivent par le pied de Parcoursup seront soumis aux mêmes conditions évoquées dans l'article 14 je crois que vous avez dit oui est ce que vous nous confirmez. c'est oui donc. ça vous engage Monsieur le Ministre. Merci, cher collègue Madame Goulet pour explication de vote. Oui, Monsieur le président, Monsieur Madame le Ministre, mais mes chers collègues, moi je vais soutenir les positions de la commission parce qu'une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance est ce que vous connaissez un proverbe normand, ce que vous connaissez monsieur le ministre, tout ça par coeur. Mais il y a pas encore tellement longtemps, notre ministre de la Défense parlait d'algorithmes quand on lui demandait des détails, on n'était pas très bien sûr qu'il avait tout compris et nous d'ailleurs et et vous serez peut-être au banc demain. Sur l'excellent texte sur la transposition du code financier sur les services de paiement dans le marché intérieur, il faudrait nous faire une version pour les nuls pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit, tant le texte qui nous est proposé et abscons, donc moi je pense que les explications que vous allez donner aux contribuables, les explications que vous allez donner dans l'exemple qui est pris dans l'excellent rapport de notre commission sur un établissement de crédit qui souhaite confier à un automate, le soin d'évaluer la solvabilité des emprunteurs, je pense que toutes les éléments que vous allez devoir donner pour justifier du détail de la procédure et de l'algorithme et les explications qui seront donnés, ce serait bien ou Poussier nous donner un exemple de de la façon dont ce sera expliqué parce que moi, voyez-vous, je doute sur non pas sur la qualité de l'explication, mais sur le le l'entendement Cora le le citoyen lambda des explications que vous allez lui donner sur une procédure qui est somme toute un peu nouvelle et qui, en tous les cas, utilisent des procédés qui sont parfois totalement étranger soit au contribuable soit au demandeurs d'un crédit et encore plus aux étudiants qui ont été visés par la procédure dont on parle tout à l'heure, donc moi je crois que plus nous donneront des garanties de d'une loi claire et des sanctions importantes puisque la nullité, finalement ça obligera l'administration à être intelligible et je pense que c'est pas une mauvaise disposition. Merci, cher collègue Monsieur de Bellmer pour explication de vote. très merci monsieur le président, Mesdames ce ministe, chers collègues, très très brièvement, j'entends les doutes sur un sujet aussi techniques, j'entends aussi un ministre qui, à la différence de celui des armées est un expert sur le sujet et démontre les choses de manière pragmatique, Claire et presque intelligible pour les non-initiés je parle a-t-il personnel mais plutôt plutôt enclin à lui faire confiance, alors peut-être que cette inclinaison n'est pas pleinement partagée dans l'hémicycle et dans ce cas, quand on n'a pas cette inclinaison à la confiance, ce qui est intéressant c'est peut-être de regarder les ceux qui sont directement concernés, vive vive les choses et on a fait le lien souvent tout au long de cet article avec l'amendement 99 qui arrive, qui évoquait tout à l'heure avec une vraie connaissance Catherine Morin- Desailly, la conférence des présidents d'université. Confirme en pratique ce que nous dit le ministre et attendra de nous que espère de nous que nous adoptions, le futur amendement 99 et donc je me dis : si le ministre est un discours que sur un certain nombre de sujets, ceux qui vivent l'utilisation de ces outils, confirme ce que dit le ministre, pourquoi prendre un risque quand le ministre nous dit qu'il y en a.

j'ai trouvé que le le ministre était plus que presque intelligible, il était tout à fait intelligible et que c'était très très solide et très argumentée, moi ce qui me ce qui m'inquiète quand même, en dernière analyse, c'est que nous disons, il faut qu'il y ait une information systématique des administrés et vous nous dites en décrivant un parcours du combattant extrêmement ardue escarpé, il y aura un recours de 1er niveau puis le 2ème niveau puis 3ème niveau et à la fin des fins, ils auront accès à toutes les informations utiles et nécessaires, je trouve que, entre quelque chose qui est systématique, est ce que vous nous avez décrit il y a quand même un monde et puis dernier sujet vous vous objecter à un argument de principe l'accès systématique à une information, un argument de moyens en disant : on ne peut pas le faire, c'est pas possible ça demande trop de temps de travail, donc je pour toutes ces raisons, parce que je reprendrais la formule normande de notre collègue, je resterai sur cette Merci, cher collègue plus décidé de demandes d'explications de vote, je mets aux voix l'amendement 98 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, je mais aux voix l'amendement 145. Avec un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il est adopté et fait tomber le suivant: 134 rectifier, je mets au moins l'article. 99 à. Oui, le fameux amendement 99. Du du gouvernement. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président Madame la rapporteur Monsieur le président de la commission des lois, mesdames et messieurs, si vous me permettez, je prendrai un peu de temps pour être précis, complet, car je crois que dans cet article, c'est peut-être l'amendement qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui présente amendement il preuve de rétablir une disposition de la loi du 8 mars 2018 relatives à l'orientation et à la réussite des étudiants supprimée par la commission des lois, avant toute chose, vous l'avez rappelé Madame la présidente, cette loi, elle est entrée en vigueur il y a tout juste 2 semaines après avoir été adopté par le Sénat en février dernier, modifié le droit applicable à ce stade de la procédure Parcoursup suscite déjà et nous sommes regardés une très vive inquiétude dans les établissements d'enseignement supérieur qui devront commencer à examiner les voeux des lycéens de plusieurs millions de lycéens dans une dizaine de jours. La commission des lois, considère que cette disposition qui protège le secret des délibérations des équipes pédagogiques, chargée de l'examen des candidatures ouvrirait la voie à la lumière de l'article 14 du présent projet de loi à une généralisation du traitement algorithmique pour produire les décisions d'affectation, sans aucune intervention humaine je voudrais donc rappeler qu'la télévision la vision et la philosophie du gouvernement dans tout le cadre de la refondation de l'accès au 1er cycle pour maître et pour mettre et pourrait l'expliquer Pour mettre un terme à l'opacité qui entoure et le fonctionnement de la plateforme APB que nous reconnaissons tous puisque ça a même été un élément que nous avons signalé dès notre arrivée au pouvoir, le gouvernement articuler la procédure d'inscription licence autour de 2 exigences fondamentales de l'humain, remettre de l'humain dans la procédure d'affectation en écartant toute prise de décision sur le seul fondement d'un algorithme c'est bien le 1er pilier de ce projet, le 2ème, c'est celui de garantir la transparence de la procédure d'affectation, autant au niveau national qu'au niveau local et je vais être très précis, d'abord sur la transparence, les nouvelles dispositions de l'article L 612 3 du code de l'éducation, qui sont issus de cette loi garantit cette transparence qu'il s'agisse du fonctionnement de la plateforme Parcoursup en général ou de la procédure du traitement des dossiers de candidature dans les établissements, les critères d'examen des voeux son public : la loi instaure un critère général la cohérence entre le profil du candidat et les caractéristiques de formation alors alors conformément aux alinéas 2 et 3 du I de l'article 612 3 toutes les informations relatives aux éléments pris en compte pour l'examen des dossiers dans les 13000 formations qui sont inscrites, dont Parcoursup chacune sont mis à la disposition des lycéens sur la plateforme, les critères d'examens ne sont pas les seuls éléments rendus publics le de de l'article prévoit que la transparence s'applique également aux traitements automatisés, cela concerne également le code source de l'outil d'aide à la décision proposée aux formation par le ministère pour les assister dans l'examen des voeux pour le redire ça veut dire qu'il n'y a pas de boîte noire, à la fois transparence sur les critères transparence sur les traitements, ouverture du code source de l'algorithme national et pour le dire très précisément, ouverture du code source de l'outil d'aide aux établissements, mais c'est pas fini,

qui exclut toute prise de décision automatisée, c'est pour ça que vous me permettrez de nuancer la présentation que vous avez pu faire de la procédure telle qu'elle a lieu dans les établissements, aujourd'hui, le décret d'application de la loi, il instaure pour chaque formation, une commission d'examen des voeux principalement composé d'enseignants chargés d'examiner de classer les dossiers, comme son nom l'indique, l'outil d'aide à la décision et je l'ai rappelé tout à l'heure, dont le code sera publié n'est qu'un appui proposé à la Commission d'examen, la Commission peut décider de ne pas l'utiliser du tout, et certaines ont décidé de ne pas l'utiliser du tout si la commission souhaite l'utiliser, alors elle doit paramétrer l'outil en fonction des éléments d'appréciation pédagogique qu'peut-elle seule déterminé en superviser le fonctionnement et ont validé le résultat, il s'agit bien d'un outil à l'amende, la commission ce paramétrage il consiste pour l'essentiel à une précision, une hiérarchisation et une pondération des critères qui ont été portés à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Donc, je le répète, transparence de ces critères, sur la plateforme et ensuite, un comité qui lui-même pourra apporter une hiérarchisation des précisions une pondération des critères seule cette commission d'examen des voeux est compétente pour décider des réponses qui seront apportées aux candidats ainsi la manière dont l'outil d'aide à la décision est utilisé est indissociable de la délibération elles-mêmes mais il ne s'y substitue pas et c'est ça qui était un élément essentiel de précision, le Module en lui-même ne peut fonder la décision de l'établissement, celle-ci ne peut pas découler, celle-ci ne peut découler que des délibérations de cette commission chaque dossier, il a été rappelé, doit être examiné, c'est l'esprit même de tout le projet chaque dossier individuel est examiné par la commission, c'est pour ça veut dire que le gouvernement a mobilisé une aide spéciale de près de 10 millions d'euros auprès des établissements pour qu'il puisse s'assurer de cette évaluation de chacun des dossiers qui est présenté. Enfin, la disposition nous souhaitons rétablir, elle permet d'ancrer dans la loi, le rôle des équipes pédagogiques et de protéger le contenu de leurs délibérations, concrètement, il s'agit de garantir à chaque candidat et je vais être très précis, je vais l'illustre à chaque candidat un accès individuel aux informations émotif qui justifie la décision prise par l'établissement jusqu'à présent, aujourd'hui, la loi de 79 relatives à la motivation des décisions administratives n'imposait pas aux équipes pédagogiques de motiver leurs notes et leurs décisions, la disposition adoptée en février dernier par le Sénat et donc une avancée majeure en faveur de la transparence, elle permet à chaque étudiant à titre individuel d'obtenir tous les éléments qui ont justifié localement la décision de l'établissement, ça va, si on les lustres jusqu'au rang qu'il a obtenu dans le cadre de la décision de cette commission, ça va même jusqu'au niveau d'appréciation qui été porté par la Commission sur chacun des critères qui a été utilisée pour l'évaluation des admissions alors l'application des dispositions droit commun, elle conduirait à rendre publics tous les éléments d'appréciation retenu par les équipes pédagogiques, lesquels sont en principe couvert par le principe du secret des délibérations, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, une telle remise en cause, elle est excessive et l'elle crée une absence de protection dans les délibérations de ces équipes pédagogiques qui, par crainte de recours contentieux serait conduite soit renoncer au Module d'aide à la décision souhaite à y recourir, mais de façon mécanique, sans l'orienter dans le sens d'une véritable démarche pédagogique, si on veut respecter cet équilibre entre la capacité de la souveraineté d'une commission, l'utilisation d'outils modernes d'aide à la décision, le rétablissement de cette attaque est la seule solution pour le faire mais en vue de se prémunir contre d'éventuelles dérives, la loi du 8 mars a par ailleurs institué un comité d'éthique et scientifique qui a vocation à prévenir ce type de risque et à garantir une intervention humaine systématique dans le traitement des dossiers et un haut niveau de protection des candidats, le Sénat a consacré l'existence de ce comité dans la loi, de manière à lui conférer pérennité et indépendance Frédérique Vidal, ministre en charge de l'enseignement supérieur, se tient à votre disposition et elle nous regarde et à la disposition des commissions des lois et de la culture afin de rendre compte du traitement des voeux et au sein de ces formations, je propose par conséquent de rétablir cette disposition en adoptant l'amendement du gouvernement et j'espère que j'aurai été particulièrement précis, nous l'avons voulu cette réponse très complète et nous l'avons travaillé avec tout le gouvernement, pourquoi vous la présenté aujourd'hui. Merci monsieur le ministre, quelle est la vie de Madame, le rapporteur de la commission. d'abord je dois dire que si le dépôt de cet amendement, permis le déblocage de 10 millions d'euros en direction des établissements supérieurs et en renfort, nous en sommes déjà très heureux, ensuite il s'agit ici de la nouvelle procédure d'affectation des bacheliers dans l'enseignement supérieur de Parcoursup on se souvient du scandale provoqué par la précédente procédure dite Admission post-bac, qui utilisait est à la fois des algorithmes de classement des candidatures, notamment dans les filières non sélectives en tension et un algorithme d'appariement les paramètres utilisés par les algorithmes de classement reposer sur une base légale qui était extrêmement fragile et jusqu'à l'an dernier il n'avait été ni explicité dans un texte réglementaire ni publiée, sous quelque forme que ce soit la communication du ministère était même vraiment délibérément trompeuses à ce sujet, je crois que c'est aujourd'hui reconnue par tous, c'est pour ça qu'on n'hésite pas à présent de sites, a tiré la sonnette d'alarme en temps et en heure, dont Parcoursup il ne sera plus fait appel à un algorithme d'appariement du même type que dans Admission post-bac, reconnaît volontiers, en revanche, les formations devront examiner reclassé un nombre de dossiers beaucoup plus élevé que précédemment et auront pour ce faire, recours à des algorithmes de classement or lors de l'examen du projet de loi relatif à l'orientation à la réussite des étudiants le 7 février dernier, le gouvernement a fait adopter un amendement de dernier dernière minute déposé en séance publique, sans que la commission de la culture et plus en faire un examen approfondi qui exonère ses algorithme de classement des obligations de transparence par le code des relations entre le public et l'administration, le rapporteur de la commission de la culture, Jacques Grosperrin avait au contraire déposé un amendement imposant dans tous les cas, la publication des règles de l'agglo, RIM et des principales caractéristiques de sa mise en oeuvre, la commission des lois a choisi de revenir sur cette première entorses aux règles de transparence définies par la loi pour une République numérique écartons d'emblée l'un des griefs avancés par le gouvernement, la suppression du dernier alinéa du I de l'article 612 3 du code de l'éducation ne prive nullement de base légale, les délibérations des équipes pédagogiques, nous voulons bien faire crédit au gouvernement, qu'aucun dossier ne sera acceptée ou rejetée sans examen sur le simple fondement du résultat, produit par la grume de classement, toutefois, la loi n'empêche pas cette dérive, le critère la cohérence entre le profil du candidat, ils attendent la formation demandée, reconnaissez-le tout de même extrêmement large sinon vague si tous les dossiers doivent être réexaminés par les équipes pédagogiques : pourquoi les prix ordonnancer au moyen d'algorithme de classement, il y a tout lieu de craindre que l'examen humain ne soit au mieux que superficielle homme a minima pour certains dossiers très bien ou très mal passé, dès lors nous paraît légitime que les bacheliers puisse savoir quels critères de classement leur ont été appliquées par voie d'algorithmes conformément au droit commun, toutefois je peux entendre ce qui me remonte depuis quelques jours aussi au niveau des des présidents d'établissements, je vous entends de la crainte que les établissements d'enseignement supérieur ne soient déstabilisés au cours de la première année d'application de Parcoursup alors qu'ils l'ont été sur le système Admission post-bac, il y a tout de même très peu de temps, l'application des règles de transparence, de droit commun, a attiré l'attention sur l'usage fait par les établissements d'algorithme de classement sur les différences entre les résultats produits par un algorithme et le classement issu des délibérations des équipes pédagogiques et pourrait évidemment encourager les recours, dans ces conditions, les enseignants chercheurs seraient encore plus réticents qui ne le sont déjà, face à la nouvelle procédure je crois nécessaire mais, chers collègues, que le Sénat réaffirme une position de principe à ce sujet, il n'y a aucune raison pour que les garanties de transparence offerte à l'ensemble des administrés ne s'applique pas à l'accès à l'université d'autant plus qu'il y a aussi une vertu pédagogique à cela, un étudiant qui aura échoué à l'entrée dans un établissement supérieur d'enseignement supérieur, une année, a besoin de connaître ces critères ne serait-ce que pour mieux se préparer à à l'année d'après, en revanche, par souci de pragmatisme mais si mes collègues en sont d'accord, je prends l'engagement au nom de la commission des lois de rechercher un terrain de compromis en commission mixte paritaire, de manière à reporter au 1er janvier 2019, l'entrée en vigueur du 3 de l'article 14 cela obligera le gouvernement revenir sur le sujet en vue de la rentrée 2019 mais laissera tout de même une année d'apaisement aux établissements supérieurs voilà, d'autre part, il nous paraît important d'énoncer clairement dans le code de l'éducation que les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ne peuvent être prises sur le fondement exclusif d'un algorithme.

Bien la rapporteure nous a déjà un peu interpellé sur son amendement, c'est aussi la raison pour laquelle je je je souhaite lui répondre mais plus généralement sur sur ce qu'on vient d'entendre, je dois vous avouer que mais avec mes collègues nous avions été extrêmement frustré de ce qui s'était passé à la fin de l'examen du du projet de loi sur l'orientation et la réussite des étudiants, puisque la question du secret des délibérations et cet amendement, qui était arrivé beaucoup trop tard et que madame la présidente, nous n'avions pas plus verrez véritablement regardez en en commission nous avait laissés sur notre faim car nous considérions en plus de l'urgence à Metz ce nouveau Parcoursup et c'est une nouvelle je dirais politique d'orientation des étudiants en plus de l'urgence des financements et de tout le contexte qui avait prévalu à l'examen de ce projet de loi qu'il y avait là un angle mort qui nous laisser vraiment sur notre faim et et je suis très heureux aujourd'hui, je vous le dis, et que nous puissions à la faveur de ce texte remettre, au moins, ce débat et à la faveur de de l'amendement du gouvernement que non, bien sûr, vous imaginez, nous ne partageons pas le contenu mais au moins la la la réflexion de la rapporteure, nous puissions de nouveau en parler, je serais très pref pour dire que je peux tout à fait entendre que, vu l'urgence, ce soit difficile effectivement que dans 15 jours, enfin, c'est à la fin du mois de mars,

entre guillemets, aux établissements, le traitement des dossiers pour classer classer les candidats et ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais nous le savons tous quand nous regardons dans nos universités, c'est que, forcément, elles vont mettre en place ce qu'on appelle des algorithmes maison, j'appelle ça maison forcément en fonction du nombre de, de, de, de dossiers parce que ça va être extrêmement difficile et c'est extrêmement difficile, on le voit aujourd'hui de le faire, donc si nous avons l'engagement comme la rapporteure l'dit que cette question de la transparence. à laquelle vous êtes attaché, forcément parce que ça participe à la fois de la confiance dans cet outil, mais aussi la confiance plus plus général que doivent avoir et que devraient avoir nos concitoyens dans la question des des algorithmes si ces principes-là si nous avons l'assurance que ces principes sont bien maintenues et seront inscrits dans la loi, avec effectivement un compromis en CMP qui permettrait au moins sur Parcoursup de lait, de les, de les mettre en oeuvre que à la début de l'année 2019, je pense que nous serons

qui dans le contexte à parasiter un peu la vision qu'on en avait aujourd'hui. Oui. Merci, cher collègue, vu les demandes d'explications de vote, qui reste je vais suspendre maintenant la séance. Il y a trop de demandes d'explications de vote, je vais être obligé de suspendre et nous reprendront à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte à 21 heures 35 pardon,